La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Pendant la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres. Mes chers collègues. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes retransmis sur Public Sénat sur notre site internet. Et chacun sera attentif. Au respect du temps de parole et du respect des uns et des autres. Je vais donner immédiatement la parole à notre collègue Cyrille va pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Monsieur Monsieur le président, madame, la Première ministre, mes chers collègues. Ce 8 juin l'horreur absolue, a frappé la paisible ville d'Annecy sur les berges du lac un assaillant a attaqué à l'arme blanche quatre très jeunes enfants de 22 à 36 mois de on vit leurs pronostics vitaux engagés et 2 adultes ont été également gravement blessés. Cet acte et de lors de l'indicible on protège un enfant on le console on l'éduque mais jamais au grand jamais, on ne le poignard dans sa poussette. Collectivement le coeur des Français s'est brisé pour les victimes et leurs parents mais aussi pour les passants traumatisés. Je le réitère notre entière et soutien. Car si l'inquiétude concernant l'état de santé des blessés s'est dissipé, le chemin de la guérison, tant physique que psychique sera encore long. Je tiens également à rendre hommage au préfet à nos forces de l'ordre et de sécurité civile aux soignants et aurait euros du quotidien comme on rit pour leur bravoure leur formidable mobilisation a sans aucun doute permis d'éviter un bilan encore plus lourd. J'ai pu voir leur choc et leur effroi face à la cruauté d'une telle attaque. Mais cela ne les a pas empêchés d'être admirable je souhaite aussi témoigner ma reconnaissance aux élus locaux pour leur réactivité en particulier au maire d'Annecy, François Astorg élu signifier mon soutien en face aux attaques indignes dont il fait l'objet. Enfin, madame, la Première ministre. Nous vous sommes reconnaissants ainsi qu'au président de la République et au ministre de l'Intérieur de vous êtes rendue rapidement sur place pour signifier le soutien de l'ensemble de la nation. Si l'heure est aujourd'hui au recueillement et s'il nous faut éviter les polémiques. Plusieurs zones d'ombres demeurent. Je ne doute pas que l'enquête en cours viendra nous éclairer sur le parcours de l'assaillant ni migratoire comme psychiatrique mais les premiers éléments qui nous sont parvenues interroges il pas en particulier que les délais de traitement de sa demande d'asile ont été particulièrement long alors qu'elle était manifestement irrecevable. Le système Eurodac permettait pourtant de vérifier qu'il avait déjà obtenu le statut de réfugié en Suède. Comment expliquez-vous donc la décision de refus ne lui a été signifié que 6 mois après le dépôt de sa demande en outre à la charte des droits fondamentaux de l'UE prévoit qu'il est possible d'accorder la liberté de circulation aux ressortissants de pays tiers résidant sur le territoire d'un État membre. Il s'agit bien d'une faculté, laissée à la discrétion des États et non pas d'une obligation. Je souhaiterais donc savoir si vous comptez restantes suédois qui lui permettait de séjourner en France sans VISA pour une durée de 3 mois, je vous remercie. je vous remercie. La parole est à madame la Première ministre madame, la Première ministre avait la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Cyril va vous l'avez rappelé jeudi dernier dans la matinée, un homme a attaqué de très jeunes enfants dans un parc à Annecy. Il n'y a rien de plus lâche de plus choquant de plus monstrueux que de s'en prendre à l'innocence de s'en prendre à de jeunes enfants. 4 enfants et 2 adultes ont été grièvement blessées dans cette attaque. Je me suis immédiatement rendue sur place avec le ministre de l'Intérieur et le président lui-même a été aux côtés des familles, en soutien à tous les intervenants dès le lendemain, au nom du gouvernement et comme vous Monsieur sénateur. Je veux dire mais pensez à toutes les victimes. Ma solidarité à leurs familles et à leurs proches et dire mon soutien aux habitants et aux familles d'Annecy profondément choqué par cette attaque. Je veux aussi remercier et rendre hommage avec vous aux forces de l'ordre qui sont intervenues extrêmement rapidement, ainsi qu'aux secours aux soignants aux citoyens dont l'action a permis de sauver les victimes et d'éviter l'irréparable. Monsieur le sénateur Pell va comme vous et comme tous les Français. Je souhaite que l'lumière lumière soit faite. Sur les circonstances exactes de cet effroyable attaque. Une enquête est en cours. Elle permettra d'éclairer les faits et les parcours et les motivations de l'auteur. En attendant les conclusions de cette enquête. L'heure est à la dignité. L'heure est au recueillement. L'heure est au soutien des victimes de leur famille et des habitants d'Annecy et je peux vous assurer que de notre côté, le gouvernement reste mobilisés plus que jamais pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci la parole. Est à notre collègue Loïc Hervé, pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président. Il faisait beau ce jeudi matin au bord du lac sur le Pâquier à Annecy. Tout à coup dans le square au pied du pont des amours qui enjambe le canal du passé. Un assaillant armé d'un couteau allait venir poignardé plusieurs petits-enfants jusque dans leur poussette avant de s'en prendre à des personnes âgées. Nous devons 1er témoin d'avoir ralenti l'agresseur puis à la chaîne exceptionnelle des forces de l'ordre, secouristes et soignants d'être intervenu avec une rapidité exceptionnelle qui a permis de sauver la vie de toutes les victimes. Notre reconnaissance aujourd'hui à leur égard est immense. Depuis cet événement tragique, la ville et toute la Haute-Savoie sont sous le choc. La venue des plus hautes autorités de l'État dont la vôtre le jour même madame, la Première ministre et le Rassemblement citoyen de dimanche ont été des occasions de témoigner notre unité est aussi notre solidarité avec les familles. Et si quelques polémiques à ses veines ont été balayés et c'est tant mieux. Des questions lourdes restent posées et attendent des réponses courageuses madame, la Première ministre. Celles-ci sont à mes yeux de 2 ordres, l'application des règles du droit d'asile et la psychiatrie. Premièrement, si le fonctionnement de l'espace Schengen fixe des règles européennes de liberté de circulation, il n'existe pas en soi de liberté d'établissement. L'auteur des faits semblerait avoir choisi de résider dans les rues d'Annecy. Depuis 7 mois. Deuxièmement, l'état de la psychiatrie hospitalière Haute-Savoie est catastrophique des services ont été fermés à l'hôpital de Thonon pour être transféré à l'hôpital de La Roche-sur-Foron où un tiers des lits sont fermés par manque de personnel dans ces conditions, comment imaginer une politique de prévention digne de ce nom. Comment aller vers les populations de 102.000 fissile fixe souvent étrangers de plus en plus nombreux qui sont dans des situations de véritables marginalité madame, la Première ministre en parallèle avec l'enquête judiciaire en cours. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les décisions préventives que le gouvernement entend prendre pour qu'un tel. Ne se reproduise jamais. Madame, la Première ministre pour répondre. À notre collègue. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président le riz Loïc Hervé, alors vous avez raison de le dire hein. Le drame survenu à Annecy jeudi dernier est un choc terrible pour tous nos concitoyens. À l'heure actuelle, les 6 blessés dont 4 jeunes enfants sont hors de danger. J'ai à nouveau une pensée pour eux, pour leurs familles et leurs proches. Et nous le devons cette bonne issue finalement en tout cas d'avoir évité le pire à l'action des forces de l'ordre des secours des soignants et des citoyens. À nouveau, avec vous, je veux leur rendre hommage. Monsieur le sénateur. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit, elle permettra de tirer les conclusions sur le profil l'état psychiatrique le parcours et les intentions de l'assaillant et je veux le redire hein. Nous avons naturellement interroger tous les services de renseignement des autres pays européens. Nous avons naturellement interroger les autorités judiciaires et aucun signalement. N'avait été connu. S'agissant de cet agresseur et aucun signalement psychiatrique n'avait été fait préalablement. En parallèle, et indépendamment de l'enquête et du drame. Notre mobilisation continue avec le goût un gouvernement avec tous les élus qui, comme vous, Monsieur le Sénateur veulent agir pour la sécurité de nos, de nos concitoyens et qui veulent veiller au respect de nos frontières et peut être pour répondre à la question précédente, je, je pense en effet que ce genre de demandes d'asile. Émanant d'une personne qui a déjà le statut de réfugié dans un autre État-membre doit pouvoir être traitées plus rapidement et nous allons également examiner ce point au-delà des démarches importante et des des avancées que nous portons au niveau européen et qui ont notamment pu se traduire lors du dernier conseil des ministres de l'intérieur par la définition d'une procédure de demande d'asile obligatoire aux frontières de l'Europe qui je pense répond à notre attente et répond à l'attente de beaucoup d'États membres européens. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 30 juin prochain, une nouvelle étape va être franchie dans la libéralisation du secteur de l'énergie, avec la suppression le suppression des tarifs réglementés du gaz et la fin du bouclier tarifaire dès le lendemain de vers 6 millions de foyers vont devoir passer d'un contrat fixe et réguler à une offre de marché c'est une folie dans la période de crise énergétique. Vous avez une vision erronée des cours du gaz sur le marché mondial. Car la stabilité que nous observons depuis le début de l'année 2023 n'est qu'une accalmie, les prix restent hauts et risque d'augmenter à nouveau dès cet hiver dans un contexte de concurrence mondiale pour la livraison du gaz qatari et du GNL américain et de reprise économique de l'industrie chinoise. Pourtant, souvenez-vous, la concurrence devait faire baisser les prix. Le résultat, rien que pour le gars c'est plus de 90% sur les tarifs en une décennie, et depuis la crise énergétique. C'est un bond de plus de 50%. Plus personne ne croit en votre fable car pour les usagers, nos entreprises et nos collectivités. C'est le raquette au profit des acteurs alternatifs et des traders qui gonflent leurs dividendes grâce au marché européen de l'énergie. Dans ce contexte, notre groupe a déposé une proposition de loi pour prolonger les tarifs réglementés du ventre du gars. Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à prolonger les tarifs réglementés ou allez-vous laisser de 6 millions de foyers être livré au marché et s'enfoncer dans la précarité énergétique.

C'est pas une fable, c'est une réalité que je vais vous raconter une histoire qui fait que depuis un peu plus d'un an. Les ménages français sont protégés contre la hausse des prix du gaz et le TRV n'a rien à voir dans l'affaire. La réalité c'est que TRV ou pas. Si le gouvernement n'avait pas mis en place un bouclier tarifaire les hausses des tarifs auraient été exceptionnel, je le répète TRV ou pas. Vous savez très bien ce qui se passe au 1er juillet, Monsieur le Sénateur. Le TRV en est terminée, conformément à une loi votée par les 2 chambres de l'Assemblée et promulguée en 2019, elle va se traduire par, en fait, aucun changement pour la plupart des 2 millions et quelques ménages que vous mentionnez puisque par défaut, ils passeront sur le tarif 10 passerelle d'Engie et pour les autres qui ont décidé de changer de fournisseur. J'imagine que s'ils le font, c'est parce qu'ils considéreront que le nouveau fournisseur et meilleur marché, ils auront peut-être même des baisses de prix. Au total, vous le voyez bien on est en train de protéger les ménages français par le bouclier tarifaire. Le prix du gaz, vous le savez, aujourd'hui il est revenu à ses plus bas qui prévalait même avant la crise et avant la guerre en Ukraine et ça il faut le reconnaître aujourd'hui que le marché européen, nous y aide évidemment le marché européen, vous savez il faut il faut le changer. Nous le faisons en profondeur, notamment sur la fixation des prix de l'électricité mais, aujourd'hui, ne fait pas peur à des ménages qui, je le répète au 1er juillet ne verront rien si ce n'est peut-être pour certains d'entre eux, une baisse de tarifs. Si. Merci monsieur le président. Jusqu'à quand. Monsieur le Ministre, nous allons respecter des règles européennes que plus personne ne respecte mise à part nous, les Portugais, les espagnols ont obtenu une dérogation. Les Allemands viennent aujourd'hui même d'annoncer un plan de 50 milliards d'euros pour subventionner et notamment sur le prix du tarif du gaz et nous on reste pieds et poings liés à ces règles que plus personne ne respecte et qui mettent à bas nos collectivités nos entreprises et surtout les usagers il urgent, créer un grand service public de l'énergie avec un monopole public et si vous le faites pas, nous le ferons à votre place. à votre place. Président François Patriat pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. De parole, monsieur le président. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues. Comment évoquer les problèmes de l'enfance sont à mon tour. Évoquer mais aussi les drames terribles arrivé récemment dans plusieurs villes de notre de notre pays. Acte ont Dieu acte monstrueux que nous condamnons tous avec fermeté et nos pensées avec les vôtres vont à la fois aux victimes, aux familles, aux cités et à leurs proches. Sans faire le lien bien évidemment. Médias je voudrais madame, la Première ministre vous interroger sur le problème de l'enfance en associant à ma question. Mon ami Xavier, Xavier Iacovelli particulièrement impliqué dans ce domaine. Vous avez annoncé il y a quelques jours mais c'est vrai que c'était occultée par les événements dramatiques que nous connaissons. Vous avez à l'issue du conseil national de la refondation évoqué la création d'un service national de la petite enfance, de façon à assurer un meilleur accueil pour les enfants en bas âge de notre pays. Cela répond en effet à une. Un engagement pris à multiples reprises par le président de la République et que vous avez tenu. En effet aujourd'hui recrutement insuffisant. Disparités régionales. Insuffisance et inégalités sociales importantes. Il est aujourd'hui indispensable de revaloriser le métier d'accueil véritable pilier de notre politique familiale mais aussi véritable pilier pour abreuver un accès et à qui table à l'emploi et au travail aujourd'hui. Donc c'est une Pierre supplémentaire dans la politique qui mène au point d'emploi aujourd'hui dans notre pays et le gouvernement tient à le faire avancer. Ce fonds est doté aujourd'hui d'un.

ce fond, mes chers collègues. Et donc doté d'un milliard et demi d'euros en projeté sur 5 ans, ce qui fait 5 milliards et demi et sept et ces 5 milliards et demi seront ancrés par l'État annoncé, vous avez annoncé Madame la bonne la ministre que ce en répondant en cela aux acteurs de terrain. Ce serait les communes qui seraient de demain les autorités organisatrices. Il y a donc 2 choses qui intéressent notre assemblée aujourd'hui la petite enfance et d'autre part, les communes concernées. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ce service public de l'enfance. Nous. Madame, la Première Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, monsieur le président, François Patriat. Assurer l'accueil de la petite enfance, c'est construire l'avenir de notre pays et montrer le modèle de société que nous voulons. Car en améliorant l'accueil des jeunes enfants. Nous répondons à une des premières préoccupations des parents. Nous avançons pour l'égalité entre les femmes et les hommes et nous levons un des freins majeurs à l'emploi. Depuis 6 ans nous avons avancé mais aujourd'hui encore les parents vivent trop souvent un parcours d'obstacles pour obtenir une place d'accueil, de fortes inégalités sociales persistent et au total le nombre de places restent insuffisants. C'est pourquoi conformément aux engagements du président de la République. J'ai annoncé un plan ambitieux avec le ministre des solidarités, Jean-Christophe Combe, pour lancer un véritable service public de la petite enfance, créer 200.000 places d'accueil supplémentaires d'ici 2030. Et garantir à tous les parents. Une réponse pour leurs enfants. Notre objectif est d'abord de permettre une meilleure coordination entre les acteurs en confortant les maires dans leur mission en tant que autorité organisatrice de l'offre d'accueil je connais l'engagement des maires et je veux le saluer ainsi le projet de loi pour le plein emploi qui portera les mesures législatives correspondante prévoit que les offres d'accueil comme les besoins des parents sont recensés à l'échelle de la commune. Il prévoit également que les grandes communes élabore des schémas stratégique pour définir une trajectoire de développement de l'offre adaptée aux besoins des des familles et je sais, Monsieur le Président Patriat que votre groupe, il est particulièrement attentif. Ensuite nous allons augmenter considérablement les moyens dédiés à la petite enfance. Conformément à ce que nous avons prévu dans notre trajectoire budgétaire. Nous allons investir plus de 5 milliards d'euros supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Il s'agit d'accompagner à la fois les investissements des collectivités mais aussi comme elle le souhaite, le fonctionnement pour ces nouvelles places de crèches. Nous voulons également faciliter la vie des parents oeuvrer à l'attractivité des métiers et améliorer la formation et je veux ici, rendre hommage à tous les professionnels de la petite enfance, enfin nous allons renforcer la confiance dans le système d'accueil, notamment en renforçant les dispositifs de contrôle et j'ai confié la présidente du conseil départemental du Maine-et-Loire. Florence Dabin une mission pour identifier des solutions rapides et efficaces pour prévenir la maltraitance. Monsieur le Président Patriat avec le service public de la petite enfance. Nous garantissons l'accès à une solution d'accueil pour tous. Nous agissons pour le plein emploi en levant une barrière au retour au travail. Nous oeuvrons pour l'égalité des chances et l'égalité entre les femmes et des hommes, ce sont des objectifs que nous partageons, j'imagine, tout ce que vous partagez tous sur ces bancs et avec la mobilisation de tous les acteurs et les élus nous réussirons. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Isabelle briquet pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci monsieur le président, ma question à laquelle j'associe ma collègue ma collègue Marie-Arlette Carlotti s'adresse à Madame, la ministre des Affaires étrangères. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine et que les populations civiles continuent d'y vivre sous les bombardements incessants. Nous nous interrogeons sur la stratégie du gouvernement en ce qui concerne l'accompagnement à la nécessaire reconstruction de ce pays ami. Ces derniers mois, les bombardements russes ont ont en effet particulièrement cibler les infrastructures civiles. Le barrage de Kakhovka et malheureusement le dernier exemple en date. Ces bombardements désorganisent le pays affilié affectent le quotidien de millions d'Ukrainiens. Amoindrissent leurs conditions de résistance et soulève la question de la reconstruction. Si le gouvernement français a apporté un soutien financier à l'Ukraine. Il n'a pas précisé sa stratégie en matière d'accompagnement des autorités dans le rétablissement des services essentiels à la vie quotidienne de la population. Quel secteur allons-nous prioriser avec quels moyens dans quel cadre. Certains pays de l'Union européenne sont d'ores et déjà présents pour appuyer pour appuyer les les efforts du gouvernement ukrainien dans de nombreux secteurs d'activité. La France n'est pas pour l'instant au rendez vous. Pourtant des opérateurs nationaux notamment privé se sont dits prêts à s'engager en faveur de ce pays allié à condition que la zone rouge soit au moins partiellement levé, cela rendrait possible leur action dans un contexte relativement moins incertain. Elles sont envisagées et sous quel délai. Au au-delà nous voudrions également savoir quel est le mandat donné aux opérateurs publics comme expertise France ou l'AfD. Afin qu'une action concertée soit réellement possible. Madame la Ministre, la France doit être aujourd'hui et surtout demain, aux côtés du peuple ukrainien. Je vous remercie. On vous réponde la parole état. Madame le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, madame Colonna. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice. L'Ukraine ne sera pas vaincu. Elle se relèvera et lorsqu'elle aura surmonté cette épreuve elle sera unie et pleinement ancrée dans la famille européenne. C'est notre conviction et nous y travaillons d'ores et déjà. En complément de l'aide d'urgence, imposé par la guerre que cette aide soit militaire, on en parle souvent au civil notamment aux moments les plus difficiles de l'hiver, nous ont aidé à la résilience du peuple ukrainien. Ou que ce soit évidemment une aide humanitaire comme nous n'avons encore montré ces derniers jours, après le sabotage du barrage en envoyant déjà 10 tonnes de matériel et nous travaillons d'ores et déjà à l'après. C'est la raison pour laquelle nous avons nommé en mars et la France était le 1er pays du G7 à le faire. Un envoyé spécial chargé de la reconstruction. Il s'agit de Pierre Heilbronn d'une excellente qualité. Il travaille en lien avec les Ukrainiens pour identifier leurs besoins prioritaires et avec les bailleurs internationaux pour construire les financements. La France met aussi en place des mesures concrètes pour les entreprises françaises qui souhaiteraient s'engager en Ukraine, elles sont nombreuses. La conférence qui s'est tenue le 13 décembre dernier à Bercy, il a montré et nous réfléchissons, je peux vous le dire, madame la sénatrice aux règles de sécurité, sachant que l'Ukraine est pour l'heure un pays en guerre. Je participerai enfin le 21 juin à Londres, à une conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine et j'annoncerai notamment de nouveaux financements pour la reconstruction des infrastructures civiles critiques celle dont vous parlez, celle qui sont attaqués, jour après jour Vous le voyez, madame la sénatrice. Il n'est pas trop tôt pour s'occuper de l'après-et c'est ce que nous faisons et nous le faisons depuis des mois déjà. Je vous remercie. La parole est à notre collègue il a une Pentel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Madame, la Première Ministre Mesdames et messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8 septembre 2024. Il s'agit d'un rendez-vous très attendu par nos concitoyens. Grever une dimension populaire et multiculturelle. Le 23 mai dernier, vous avez signé un protocole de sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Cela représente au total une mobilisation de 35.000 membres des forces de l'ordre, gendarmes, policiers et agents du ministère des Armées, auxquels s'ajouteront des agents de sécurité privés privée pardon et ceux de la ville de Paris. Aussi, vous avez annoncé le déploiement de 2800 agents supplémentaires d'ici d'ouverture des Jeux. Il ne fait aucun doute que ces décisions sont le fruit d'une évaluation détaillée des besoins d'une manifestation de cette envergure. Or, Monsieur le Ministre force est de constater que l'on voit poindre dans nos territoires ruraux la probabilité d'une réquisition des agents des services de sécurité publique qui exerce quotidiennement dans nos brigades de gendarmeries et commissariats de police. La conséquence indésirable qui se profile, c'est l'impossibilité en terme d'effectifs d'assurer un appui pour la protection des événements sociaux, culturels et sportifs d'un aux régions et d'un provoqué l'annulation. En effet, bon nombre d'associations n'ont pas les moyens financiers d'engager des sociétés de sécurité privées et les petites communes ne disposent pas de policiers municipaux. Ainsi, avant que la flamme olympique ne gagne Paris plus de 60 départements devraient être traversée. Or, vous conviendrez que cela ne servirait à rien si une partie des Français étaient privés d'un été festif en 2024. En conclusion que prévoyez-vous pour garantir l'équilibre territorial des effectifs des services de sécurité publique sur la période des Jeux, notamment dans les territoires ruraux. Les renforts estivaux seront-ils maintenus et les Psig ne vont-ils pas être déplacés. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est à madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Madame, Sonia Backès ce vous avez la parole madame la Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Pentel. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Vous le savez, sont un événement planétaire qui nécessitera une mobilisation totale et sans précédent de nos forces de sécurité, Gérald Darmanin a eu l'occasion de le dire devant vous l'engagement du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer ne pourrait être que total pour garantir la sécurisation optimale de l'événement mais aussi pour garantir et assurer la sécurité de nos concitoyens dans les territoires. Les forces de sécurité intérieure seront en première ligne, vous l'avez dit, chaque jour près de 35.000 à 35.000 agents des forces de sécurité intérieure seront mobilisés. La réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale forte de 31.000 femmes et hommes, et les réserves des écoles de police et de gendarmerie seront également mobilisés. La décision a été prise de suspendre le temps des Jeux la distinction entre zones de compétence, police et gendarmerie, cela permettra une organisation par mission plus adapté à la situation. L'engagement des personnels de sécurité privée des agents des polices municipales et des militaires des forces armées sera nécessaire pour parfaire le dispositif global. Bien sûr, nous pourrons compter sur l'appui de l'ensemble des technologies de sécurité de renseignement autorisé par la loi sur l'ensemble du territoire national. Les forces de sécurité seront mobilisés pour garantir la sécurité quotidienne des Français. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Vous le savez, a demandé aux préfets de mettre en oeuvre des plans zéro délinquance, vous le voyez, madame la sénatrice, tout est fait pour anticiper et préparer au mieux cet événement majeur pour la France sans mettre en difficulté les territoires. Vous savez, pouvoir compter sur la mobilisation entière des femmes et des hommes de la gendarmerie et de la police nationale, nos forces de sécurité seront n'en doutons pas à la hauteur, je vous remercie. La parole est maintenant au président Guillaume Gontard. Pour le groupe. Écologiste solidarité et. Merci, merci monsieur le président, madame, la Première ministre. Jeudi dernier l'horreur a frappé à Annecy et a étreint le coeur du pays tout entier, 7 personnes dont 4 enfants ont été victimes d'une sauvagerie aussi absurde qu'incompréhensible. À toutes les victimes à leurs parents à leur famille, à leurs proches à la ville d'Annecy meurtri à son maire François Astorg gars la France sidérée. Les écologistes, apportent leur soutien. Le pire de l'humanité côtoie souvent le meilleur nous admirons l'héroïsme des passants qui ont tenté de s'interposer, celui d'Henri, qui a mis assaillants en fuite. Nous saluons le professionnalisme des forces de l'ordre qui ont un interpellé rapidement l'individu le sang froid de celles et ceux qui ont prodigué attend les premiers soins. Nous remercions les médecins qui ont travaillé sans relâche grâce au bouclier inestimable que représente le services publics encore pire a été évité. Madame, la Première ministre, alors que les vautours avaient quitté leur nid plus vite qu'à le coutume vous avez avec la droiture que vous nous connaissons appeler chacun à la dignité. Nous saluons ce propos, nous le faisons nôtre. Face à l'horreur, le plus grand danger qui guette le corps social c'est la désunion face à la folie. La colère et la haine émotion compréhensible sont néanmoins parfaitement vaine la haine néonazis qui s'est déversée en toute impunité dans les rues d'Annecy appel la condamnation la plus ferme de tous les républicains. La haine raciste qui se déchaîne contre le maire d'Annecy, appelle le soutien sans faille de toute la classe politique. Nous appelons chacun et chacune à ne pas céder aux sirènes de de la démagogie a ignoré les solutions toutes faites aussi inepte qu'injuste la haine la peur et le rejet de l'autre, ne pas nous protégerons jamais nos enfants. Bien au contraire, c'est la justice, la bienveillance l'inclusion, la solidarité, la prise en charge de la matinée de maladie mentale. Tous ceux qui luttent contre la misère et l'isolement tout ce qui renforce la communauté humaine qui protégera la nation et ses enfants. Madame, la Première ministre, comment comptez-vous agir pour assurer la tenue de cette ligne de dignité. Merci. On vous la parole est à madame la Première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le président Gontard. Vous avez rappelé les faits et le drame qui a touché Annecy jeudi dernier et profondément marqué notre communauté nationale. Qu'il me soit permis à nouveau de dire mon soutien aux victimes ma solidarité envers les familles, les proches et les Annéciens. Qu'il me soit permis encore car nous ne le faisons jamais assez de rendre hommage à la police nationale à la police municipale. Au secours aux soignants et aux citoyens qui ont permis de stopper rapidement ce drame et de sauver les victimes. Alors qu'il est. Leurs jours ne sont plus en danger. Monsieur le Président Ganta Gontard. L'enquête fera la lumière sur les circonstances précises de ce qui s'est passé. Il ne m'appartient pas d'en anticiper les conclusions. Certains ont tenté de qualifier les faits et leur et, leur hauteur alors même que nous ne connaissions pas son identité que certaines victimes étaient entre la vie et la mort. Face à un tel drame. Il n'y a pas place pour des polémiques politiciennes. Soyez sûr, monsieur le président que je refuserai toujours les accusations hâtives et les tentatives de récupération, elles ne sont pas dignes du drame que nous avons. Alors Alors avec le ministre de l'Intérieur avec les forces de sécurité intérieure. Nous sommes mobilisés. Nous sommes au travail pour protéger les Français. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Daniel chassa pour le groupe les indépendants. Le but et territoires monsieur. Monsieur le président, madame de mise la chanter, chers collègues. Le président de la République veut renforcer la souveraineté de la France. Quant à la production de médicaments, c'est bien. Il faut aussi améliorer les conditions de travail des infirmières libérales. Je viens de rencontrer en Corrèze, les représentants d'un collectif de 340 infirmière tous les jours de la semaine le week-end et jours fériés. Ces professionnels passionnés par leur métier se rendent au domicile des personnes dépendantes et pour des soins chroniques. Pilier du maintien à domicile. Elles sont pourtant maltraités au niveau de leurs revenus. L'indemnité forfaitaire de déplacement et passé deux euros 30 à 2 euros 50 en 2000. Lancent l'indemnité kilométrique de 0 35 à 0 50 en 2009, les actes médicaux infirmiers de 3 euros à trois

Un exemple, une personne de 93 ans dépendante mais non d'un continent est classé BSA, il existe 3 passages à domicile matin toilette lourde midi des médicaments le soir pour la toilette, l'infirmière d'apercevoir. 36 euros percevez avec les AIS aujourd'hui elle ne peut facturer que le PS BSA trois euros, 13 euros. Certaines infirmières sont obligés de refuser des soins. Beaucoup d'actes sont hors nomenclature Madame le Ministre faut conserver les infirmières elles sont les collaboratrices indispensable des médecins. Elles sont les fantassins du maintien à domicile, pourtant elles n'ont bénéficié d'aucune revalorisation depuis 2011. Comment allez-vous prendre en compte leurs légitimes revendications. Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée. Chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé Madame Firmin Le Bodo. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Chassaing. Vous avez raison, Monsieur le Sénateur, de souligner l'importance et le rôle primordial des infirmiers et infirmières libéraux dans notre système de santé. Il s'agit de la première première professions de santé libérales en France métropolitaine. Elle est également la plus présente en zone rurale et dans les petites agglomérations. François Braun et moi-même ne cessons de le réaffirmer le gouvernement soutient l'application essentielle des infirmières libérales auprès des patients. À ce titre, nous accordons bien entendu une importance prioritaire au sujet de leur rémunération. D'une part parce qu'il est important de reconnaître financièrement l'étendue des services de santé qu'ils assurent, d'autre part parce que comme l'ensemble de nos concitoyens. Ces idées elles sont touchés par les tensions sur le pouvoir d'achat qui parcourt l'ensemble des secteurs économiques face à cette situation, nous avons souhaité que les partenaires conventionnels puisse ouvrir des négociations rapides et ciblées pour que les idées, elle puisse bénéficier d'un rapide soutien à leur activité de soins. Ces discussions se sont ouvertes avec l'assurance maladie, les échanges de la semaine dernière se sont bien déroulées et devrait nous l'espérons aboutir rapidement à un accord, nous ne pouvons que nous en féliciter sur le sujet du BSI je connais également les les débats qui traversent la procession de la profession sur le déploiement des bilans de soins infirmiers. J'ai l'occasion de prendre une tournée avec une infirmière libérale et nous en avons échangé largement si les déploiements de ce ben ici a été décalé je veux vous assurer sur ce point, cette réforme du mode de financement des actes infirmiers demeure pertinente et nous souhaitons la poursuivre rapidement. Il s'agit en effet d'un outil pertinent et efficace dont les infirmiers, ce sont des ordres d'ores et déjà saisi. Enfin la meilleure reconnaissance des idées, elle passe aussi par une meilleure connaissance de leur compétence et de leur expertise l'ouverture d'un nouveau Champ d'exercice autonomes en exercice coordonné pour la prise en charge des plaies, le droit de prescription d'administration de l'ensemble des vaccins ou encore l'expérimentation de la réalisation de certificat de décès. Enfin dans le cadre de l'examen de la PPL Valletoux le gouvernement soutiendra l'amendement permettant de créer le statut d'infirmier référent. C'est aussi ce que nous faisons dans avec l'ambitieux chantier de refondation du métier d'infirmier que nous avons ouvert le 26 mai dernier. Monsieur. Si Madame la Ministre d'écouter ces professionnels, elles font un travail formidable pour le maintien à domicile. La parole est à notre collègue Laurence Garnier pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur Merci monsieur le président, ma question s'adresse à la Première ministre. Madame, la Première ministre dimanche dernier des délinquants des soulèvements de la Terre ont violé des propriétés privées. Détruit des outils de travail saccager les cultures des maraîchers nantais. Ils ont arraché des cultures expérimentales. Économes en eau qui avait précisément pour vocation de préparer la transition écologique du maraîchage. Sur le site. Et c'est encore plus grave. Il y avait des élus de la République. Présent. En écharpe tricolore aux côtés de ces délinquants. Ils sont la honte de notre République. Le Le 25 mai à Brévin, il défilait la main sur le coeur contre les violences d'extrême droite. Le 11 juin à Pont Saint Martin il soutenait les violences des éco-terroristes d'extrême gauche, madame, la Première ministre. Vous êtes la garante de l'ordre public et vous avez les moyens d'agir. Les conseils des ministres se succèdent et la dissolution promise. Des soulèvements de la Terre n'est toujours pas prononcé. C'est pour quand. Vous devez aussi agir à l'encontre des élus présents et demander à votre ministre de l'Intérieur de les suspendre de leurs fonctions comme il autorise le code général des collectivités territoriales. L'écologie est en train de devenir le totem d'immunité d'une extrême gauche qui appelle de ses voeux la zadisation de notre pays. Madame la ministre. Vous avez cédé. À notre dame des Landes ne cédait plus face au totalitarisme Vert. Vert. Répondent. La parole est au ministre délégué. Chargé du renouveau démocratique porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les. Les sénateurs, madame la sénatrice Laurence Garnier, merci pour votre question évidemment. Le constat que vous faites. Il est partagé, très largement, au-delà d'ailleurs des clivages politiques quand on veut militer. Quand on veut militer pour le climat, on n'arrache pas des salades, on arrive pas du muguet, quand on veut militer pour la terre on ne harcèle pas et on n'humilie pas les agriculteurs qui nous nourrissent et qui font vivre à la terre. Et quand on prétend porter une cause sociale écologique humaniste. On s'en prend pas aux gens encore moins aux forces de l'ordre, on n'organise pas des manifestations interdites. C'est une évidence que vous rappelez, et c'est d'ailleurs pour cela que je peux vous confirmer que nous. Le gouvernement a la ferme intention la Première ministre à la ferme intention de pouvoir présenter en conseil des ministres le dossier de dissolution de soulèvements de la Terre. Le dossier est en cours de constitution, de manière à être absolument impeccable comme vous pouvez vous pouvez l'imaginer après vous m'interrogez, vous interrogez le gouvernement sur la présence d'élus, il y a quelque chose qui ne va pas. Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas un élu de la République, quel que soit son mandat, quelle que soit son parti n'a pas participé à une manifestation lorsqu'elle est interdite par la préfecture. C'est la base. C'est la base. Un élu de la République n'a pas participé. Par sa présence et donc a cautionné par sa présence des exactions qui sont réalisés en l'occurrence contre des agriculteurs tout en prétendant les défend lorsqu'ils sont dans leur territoire, leur circonscription, ça aussi c'est la base, madame la sénatrice et nous sommes pleinement d'accord enfin quand on porte une écharpe tricolore. Quand on est porteur de la confiance de ses concitoyens quand on est porteur d'un mandat qu'il soit local ou qu'il soit national, on doit tout simplement être à la hauteur de la confiance qui nous a été conféré la hauteur du drapeau tricolore que 12 arborant je vous remercie. La parole est à notre collègue. Lui va. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le ministre du Travail, l'Observatoire des inégalités, vient de sortir à un dernier rapport et il est parfaitement documentée Prouve, s'il le fallait, avec des arguments extrêmement sérieux que la fracture sociale continue à se creuser. Dans ce pays, les ouvriers et les employés qui représentent 20%. Des Français ne voient pas leurs conditions de vie s'améliorer et pire encore, ne voit pas ne des perspectives d'avenir pour leurs enfants et ils prennent de plein fouet la réforme des retraites qui les pénalisera à eux en premier, nous n'y reviendrons pas. Nous voyons arriver là-dessus. Le projet de loi plein emploi. Alors certes dans ce projet de loi il y était question nous avions entendu parler. De travail obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Cette mesure ne figure plus dans le projet de loi, d'abord elle était complètement incongrue et ensuite elle était de toute façon. façon. Impossible à mettre en oeuvre. Il n'empêche, il n'empêche que nous pensons très fortement que ce projet de loi servira à stigmatiser les plus pauvres d'entre nous il jettera l'opprobre, une fois de plus sur les plus propres pauvres d'entre nous parce que il est simpliste de penser que on pourra mettre à l'emploi des gens qui en sont aujourd'hui le plus éloigné, parce que ce qui reste aujourd'hui au RSA sont ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Donc Monsieur le Ministre, moi je vous demande simplement quelles mesures vous allez prendre dans les mois qui viennent pour enfin prendre en compte et cette question de la fracture sociale, sans pour autant toujours stigmatiser les plus pauvres. vous répondre. La parole est au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, monsieur Dussopt. Vous. M'interrogez Madame la sénatrice sur la fracture sociale et sur les difficultés qui peuvent survenir. Je crois qu'une des causes de la fracture sociale, c'est la précarité, le maintient dans la précarité, c'est l'exclusion et le maintien dans l'exclusion. Lorsque nous regardons les faits qui sont là aussi très bien documenté. Je pense à un rapport de la Cour des comptes de demi-début 2022. Que dit ce que dit ce rapport au sujet des allocataires du RSA. Il dit que, en moyenne 7 ans cette année complète. Après une première inscription RSA 42% des bénéficiaires sont toujours inscrits au RSA, soit de manière continue, soit de manière récurrente et il dit que seulement 33% de ces mêmes inscrits ont retrouvé un emploi souvent un emploi d'ailleurs qui ne se caractérise pas par la stabilité et c'est un euphémisme. Je crois que nous avons à agir parce que ce chiffre 4. 4 allocataires sur 10 qui s'étend après sont encore RSA ça vient, si il y a une forme d'échec collectif Échec sur des questions de formation, nous y répondons avec le pic, cela prend du temps, mais c'est efficace. Échec aussi sur notre capacité à accompagner lorsque l'on regarde la création du RMI en 1988 la loi disait que 20% des fonds devait être consacrée à l'insertion et 80% l'allocation. Aujourd'hui nous sommes à moins de 10% pour l'insertion, c'est aussi une explication que faire le gouvernement c'est investir de manière massive dans cet accompagnement. C'est ce que préconise le rapport que m'a remis le haut-commissaire au mois d'avril et ce que nous voulons faire, c'est réformer l'accompagnement des allocataires du RSA le réformer, comment d'abord en mettant des moyens, je l'ai dit en ayant un diagnostic social et professionnel et un suivi social et professionnel du château aujourd'hui presque un allocataire sur 5 17 pour % ne n'a ni suivi social ni suivi professionnel et en élaborant avec eux en application de la loi, non pas de la nouvelle loi mais lois de 88, un contrat d'engagement réciproque prévoyant des activités d'insertion, de formation d'accompagnement. Nous ne parlons pas de bénévolat obligatoire ni travail gratuit mais d'accompagnement est ce que nous y arriverons surtout peut être pas mais le pire, ce serait renoncer ça serait renoncer parce qu'il y a 9.950.000 foyers qui aujourd'hui ne pas que du RSA et ça, ça n'est pas une situation acceptable. C'est cela qui qui nourrit la fracture sociale que vous dénoncez. Monsieur le Ministre, je partage ce que vous venez de dire, une fois n'est pas coutume, parce que le rapport de la de la de la de la Cour des comptes est parfaitement explicite et nous savons que la dans une dans une mesure assez importante l'inclusion ne fonctionnait pas, dans votre projet de loi dans le zéro, l'occasion de discuter. J'ai vu certaines mesures dont je ne comprends pas bien l'utilité, je n'ai pas vu de moyens supplémentaires et je crains qu'on ne confie l'insertion des bénéficiaires du RSA à des personnes qui ne le connaissent pas parfaitement qu'ils ne connaissent pas suffisamment, c'est public. La parole est à d'autres collègues qui luttent Tabarot pour le groupe Les Républicains, vous avez là. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les lois de l'homme et climat et résilience ont engagé la mise en place progressive de ZFE. L'objectif est d'éviter 7000 décès par an directement liés aux oxydes d'azote qui proviennent majoritairement du transport routier. Mais comme vous le savez, un grand nombre de nos concitoyens vivent très mal. Ces différentes mesures. Cette mauvaise perception est confirmée par une consultation sénatoriale où sur plus de 50.000 réponses, 86% sont défavorables ou très défavorables aux ZFE nos concitoyens voudrait bien mais ne peuvent pas quelquefois se séparer de leur automobile, faute de moyens pour le faire ou de transports en commun adaptés. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité après une cinquantaine d'audition présenté un rapport d'information que j'espère réalistes concrets et de bon sens. Au terme de ce travail, nous vous adressons un certain nombre de recommandations, en réponse aux inquiétudes de nos concitoyens mais an parfois colère et Roger dans le contexte que nous connaissons de baisse de pouvoir d'achat. Aussi, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt à renforcer les dispositifs d'accompagnement pour les ménages modestes et ce résident loin des ZFE avec le prêt à taux zéro ou le leasing social, d'offre en transports communs et assouplir le calendrier de restriction de circulation comme le Sénat le préconise, êtes-vous prêt à rendre ce dispositif plus lisible et à engager une réelle planification de plus long terme pour éviter d'envoyer 13 millions d'automobiles à la casse dans moins de 2 ans. Êtes-vous prêt tout simplement à réconcilier, qualité de l'air et acceptabilité sociale si ce n'est pas le cas Monsieur le Ministre, j'ai peur que les tensions sociales que les gouvernements ont connu avec la hausse du coût du carburant les limitation à 80 km/h ou la taxe carbone ne soit que le hors-d'Oeuvres de ce qui ce qui vous attend demain. On vous répond. La parole est au ministre de la transition écologique et de la cohésion des. Monsieur le Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le. Sénateur Tabarot avant toute chose, je suis prêt à vous recevoir avec le président Longeau pour que vous puissiez me donner. Le caractère complet de ce rapport, dont je salue l'existence et la temporalité. J'avais eu l'occasion il y a quelques semaines ici même de vous dire que le 10 juillet. Je ne crois pas avoir donné le jour mais qu'au début du mois de juillet. France urbaine. Et les élus qui sont d'ores et déjà concernés par une partie de ces ZFE. À commencer par le président Moudenc et par la vice-, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg Anne-Marie Jean vont remettre un rapport sur, d'après eux, tout ce qui ne va pas tout ce qu'il faut améliorer et la manière de rendre plus facile plus acceptable plus soutenable. L'ensemble du dispositif. J'ai lu. Dans quelques bribes de presse des idées qui me semblent pertinentes qui me semble pouvoir aller dans le bon sens et j'en profite. Peut être pour amener tout de suite un ou 2 éléments d'apaisement. Rien dans la loi rien. Ne prévoient pour le gouvernement d'aller un jour imaginer interdire les critères de. Pour les Crit'Air 3 il n'y a que les agglomérations qui serait en dépassement de seuil qui seraient concernés. Le chiffre d'agglomérations susceptibles de se retrouver dans cette situation et à l'heure actuelle de 5. Et la loi prévoit que une partie des 43 agglomérations concernées. Pourront bénéficier d'exonérations compte de leur qualité de l'air et nous sommes sur le point de publier ses chiffres qui va concerner de nombreuses agglomérations de plus de 150.000 habitants dans le pays. Je vous rejoins sur beaucoup de points. D'abord si nous avions. Posé la question aux Français ce que vous êtes pour que on diminue le nombre de décès des particules fines du dioxyde d'azote ou de l'espérance de vie. 100% des gens auraient dit, oui. Pour autant, c'est pas parce qu'un objectif et noble que les moyens qui permettent de. De l'atteindre. Ne doivent pas être regardée de façon fine vous évoquiez y compris dans votre rapport avec la pollution de l'air ne se limite pas à la question du transport routier et qu'il faut qu'on ait une approche globale. Notre vision, les simple protéger la France, la santé de nos concitoyens. Faire en sorte d'avoir une, une réforme qui soit concrète qui assouplissent le dispositif des ZFE en préservant l'essentiel mais en évitant les crispations qui pourrait être généré par une application aveugle. La parole est à notre collègue daphné Ract-Madoux pour le groupe de l'Union centriste. J'ai bien conscience en posant cette question, qu'elle n'intègre pâle la totalité du territoire national. Ni qu'elle concerne la totalité des Français. Mais que voulez-vous. Elle appelle une question, une réponse nationale. Elle concerne la ratification. Par la France d'un accord européen. Portant sur la durée de travail au télétravail des travailleurs frontaliers, accord qui comme vous le savez. permettra dès le 1er juillet prochain avec l'autorisation de l'employeur de passer de 25% à 49% la durée de travail télétravail être télétravaillé en maintenant c'est ça l'avantage. Le régime de couverture sociale. Dans mon département. Un beau département, celui de la Moselle. Que je vous invite à visiter toutes et tous. 100.000. Plus de 100.000. Travailleurs frontaliers parce je dirais essaie de passer la frontière. Avec tant de difficultés, puisque toutes les voies routières, autoroutières sont saturés et les bus et les trains sont tous bondés. Et voyez-vous cette. Avancée européenne. Pour régler non seulement le volet social mais aussi le volet environnemental et à améliorer sensiblement enfin la moins pénible. La qualité de vie de ses habitants. Mais pour que cette avancée ne soit pas fictive mais qu'elle devienne réel, encore faut-il que la France comme l'a fait l'Allemagne et le. Et la Belgique ratifie cet accord. La question est simple, monsieur le Ministre quand allez-vous ratifier cet accord et. Le ratifierait vous. Merci beaucoup. Pour vous répondre. La parole est au ministre du Travail. L'emploi monsieur Dussopt. Merci monsieur le président, monsieur le sénateur, vous vous m'interrogez effectivement sur. La signature possible par la France de l'accord multilatéral consacré au télétravail en rappelant l'application de la loi telle qu'elle est prévue aujourd'hui puisqu'en application du règlement européen dit de coordination des régimes de Sécurité sociale règlement 883 les travailleurs qui télétravail actuellement plus d'un jour par semaine dans leur état de résidence voient leur législation sociale basculer

pour augmenter le nombre de jours de télétravail possible sans qu'il y ait bascule dans la législation sociale de l'État de résidence et avec maintien dans la législation sociale de l'État, où est située l'employeur. Cette période de flexibilité a permis de neutraliser les effets sociaux du télétravail pour accompagner nos compatriotes frontaliers face à cette situation, où la crise a amené un délai plus long très sensible du télétravail. Nous avons voulu tous les États travailler pour intégrer plus durablement ces changements et une commission administrative pour la coordination des régimes de Sécurité sociale a été créé et a mis en place une période de flexibilité jusqu'au 30 juin de cette année, les États membres de travail et de ses de ce travail du groupe ad-hoc est sorti un accord multilatéral qui a déjà reçu l'agrément d'un certain nombre d'États membres et d'État frontaliers. nous sommes en train de regarder aujourd'hui quelles sont les conséquences exactes de cet accord multilatéral. Vous l'avez évoqué sous l'angle de la facilité de vie pour nos compatriotes transfrontaliers qui pourraient ainsi travailler à leur domicile plus facilement. Il faut aussi que nous puissions mesurer les effets en termes de recettes de cotisations sociales d'externalités sur les bassins d'emploi de dépenses d'indemnisation chômage mais aussi de recrutement dans les bassins concernés. Nous le faisons et je le précise, en lien avec un autre débat qui anime le Conseil des ministres européens du travail qui concernent la révision de la totalité du règlement 883 qui ne porte pas uniquement sur le télétravail, mais bien sur l'ensemble de la coordination de la sécurité sociale dans les tout prochains jours sur l'autorité de madame, la Première ministre nous arrêterons de notre position définitive en tenant compte de l'ensemble de ces paramètres. Mais aujourd'hui le texte auquel nous avons participé, est encore à l'instruction de service. Merci la parole est à notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe Les Républicains. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre la semaine dernière sur le site gouvernemental, je veux aider Point gouv Point FR plateforme publique de l'engagement, on pouvait découvrir une jeune fille voilée qui a subrepticement été remplacé 3 jours plus tard par une autre jeune fille à la tête. Découverte. Alors ma question est simple, Madame la Ministre comment nous faire croire que le gouvernement lutte contre les abayas lorsqu'il affiche ouvertement sur un site gouvernemental. Une jeune fille voilée sous le drapeau français et donc, plus globalement, quelle est la ligne du gouvernement en matière de lutte contre l'inquiétante offensives islamistes dans notre pays. Pour vous répondre. La parole est à madame Sonia Backès secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, pardon. Il ne m'appartient pas de de commenter l'exemple que vous avez pris, mais nous ne sommes pas naïfs. La République, l'école de la République en particulier est en ce moment la cible d'organisations islamistes qui via les réseaux sociaux organisent des, des attaques contre la loi de 2004. Depuis la rentrée scolaire 2022. Les services de renseignements qui sont en lien constant avec les responsables des communautés éducative documente une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école. Nous suivons cette évolution en lien étroit avec le ministre de l'éducation nationale et ses services comme vous, nous avons entendu les demandes légitimes des enseignants et des chefs d'établissements de disposer de consignes claires. Nous leur devons cette clarté. Je me permets de vous rappeler Madame la sénatrice. La loi de 2004 qui interdit explicitement le port de tout vêtement ostentatoires en milieu scolaire public en application du principe de laïcité. Pour le dire plus clairement et dans la droite ligne des propos que j'avais tenu en octobre dernier, les abayas et les qamis constituent des vêtements religieux par destination dès lors que la finalité qui s'attachent à leur port ne fait aucun doute et qu'elle constitue une tentative de contournement manifeste de la loi de 2004. Dès lors, les chefs d'établissements concernés sont fondés à prendre des sanctions contre les élèves. À l'origine à l'origine de tels comportements et à leur interdire l'accès à leur établissement. Cette ligne et celle du gouvernement. Je rappelle qu'elle avait été indiqué dans une instruction aux préfets envoyé par Gérald Darmanin et moi-même le 17 octobre dernier. Je le dis clairement, madame la sénatrice, la loi de 2004 est une loi protectrice et une loi d'émancipation et nous devons veiller à sa stricte application sans naïveté et sans complaisance. Je ne suis pas certaine Madame la Ministre que les Français soient rassurés et convaincus par vos propos j'ai posé quelques questions, comment expliquez-vous qu'une conférence à la Sorbonne sur l'entrisme des Frères musulmans initialement reporté ce soit tenu sous haute protection, sans le soutien de la ministre concerné. Comment expliquez-vous le silence il l'inaction du ministère de l'Éducation nationale pour faire en sorte que le collège de Conflans où enseignait Samuel Paty porte son nom. Comment expliquez-vous l'ambiguïté du discours gouvernemental autour de l'abaya et vous m'avez pas rassuré fruit du wahhabisme de l'Islam le plus rigoriste prônée en prônée en Arabie Saoudite, que l'on voit prospérer de manière inquiétante dans nos collèges et de lycées. Comment expliquez-vous le silence du ministère à l'égalité femme sur tous ces sujets. Alors que de plus en plus de petites filles sont voilées dans notre pays. Petite fille auxquels on inculque l'idée que leur corps est sale et un pur et doit être caché du regard de des hommes. N'y a-t-il pas des mots que tout le monde connaît et capable de comprendre dès son plus en 2, son plus jeune âge les mots non est interdit. Alors pourquoi ne jamais les utiliser afin de préserver l'unité de la nation et de la communauté nationale. Ne pas répondre à toutes ces questions avec clarté, ne pas choisir ses permettent l'offensive islamiste de continuer à progresser. Vous en êtes et vous en serez redevable devant les Français. si la parole est à notre collègue. Gilbert Luc de ménage pour le groupe socialiste. L'écologiste et républicain. Merci, monsieur le Président Madame la Ministre poêle en téflon textiles industriels emballages alimentaires, les milliers de qui fasse sont partout dans notre quotidien. Malheureusement ces molécules quasiment indestructible sont également présentes dans les rivières l'eau de pluie, les sols, l'alimentation et le lait maternel et ton face au poison du siècle. Je viens de la région la plus exposée à ces polluants éternels après les recommandations émises par l'ARS de ne pas consommer des poissons pêchés dans le Rhône, puis les oeufs et la et les volailles. Voilà qu'un documentaire révèle l'imprégnation extrêmement élevé des riverains de l'usine Arkema cette fois plus que la moyenne des français. Une plainte a d'ailleurs été déposée le 25 mai par un collectif d'associations et de citoyens, les habitants comme les élus sont à juste titre, très inquiets, car les effets nocifs et toxiques de certaines substances sont désormais reconnus. Selon le dernier rapport de l'Inspection générale de l'environnement, la France ne réglemente aucun puis face. Le constat est sévère pour notre pays. Le gouvernement a annoncé un plan d'action pour 3 ans où aucune norme concernant les rejets industriels n'est proposé. L'urgence est pourtant réelle aussi Madame la Ministre comment votre gouvernement compte-t-il accompagner les collectivités touchées par ces problèmes. Qui paiera la dépollution des sites contaminés et à quand une vaste étude d'imprégnation sur les populations locales. On vous répond de la parole est à la ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé que vous avez la parole. Merci monsieur le président, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur de Villeneuve mieux prendre en compte les effets et maîtriser les risques pour l'environnement. La santé liés à l'usage des P. face les polyfluoroalkylées. Répond à une préoccupation forte et légitime de nos concitoyens. Vous l'avez dit, c'est un enjeu de santé publique essentielle est une priorité de notre action sur laquelle le gouvernement est pleinement mobilisée au niveau national et européen, sur laquelle nous devons une transparence complète sur les informations dont nous disposons. Avec Christophe Béchu. Nous avons souhaité renforcer notre ambition collective sur ce sujet dans le cadre d'un plan d'action lancée en janvier dernier. Ce sont des actions concrètes en matière de maîtrise des rejets industriels et de connaissance des contaminations environnementales. La priorité, c'est de l'amélioration de la connaissance des rejets ainsi que de l'imprégnation des milieux pour réduire l'Exposition des populations. À ce titre, l'analyse des effluents industriels fortement susceptibles de contenir des PFAS fait actuellement l'objet d'un projet d'arrêté ministériel ouvert à consultation du public. Ce projet d'arrêté vise environ 5000 installations industrielles sur l'ensemble du territoire français couvrant la quasi-intégralité des sites pouvant produire utiliser ou rejeter des L'objectif c'est de mieux surveiller et engagé en conséquence des actions de réduction des émissions. J'ajoute que la directive européenne eau potable rend obligatoire à partir de 2026, le contrôle sanitaire des face dans l'eau, nous avons souhaité anticiper cette exigence et rendre ce contrôle applicable dès janvier dernier pour mieux surveiller la présence de ces polluants dans les eaux. Concernant la situation de Pierre-Bénite en lien avec le préfet nous avons prescrit à l'entreprise Arkema la réduction par paliers, puis l'âge l'arrêt des rejets en paix face sur le site de Pierre-Bénite d'ici fin 2024. Par ailleurs, à la suite de la première campagne des mesures dans l'environnement réalisée par Arkema conformément aux arrêtés préfectoraux du 1er juillet 2022. Des mesures supplémentaires de paix face dans les sols et dans les végétaux ont été demandés à l'exploitant autour de leurs installations et à leurs frais. Afin d'avoir une meilleure connaissance des risques sanitaires enseigne a été saisi en novembre dernier, des éléments de réponse sont attendus fin d'année. En complément, Santé publique France va déployer le futur programme national de bio-surveillance Alban qui s'installera s'intéressera particulièrement à cette Exposition hop merci Monsieur. Le président ma. Merci de votre réponse. J'entends bien surveillée, c'est bien, agir c'est mieux et il me semble que si des démarches ont lancé au niveau européen, on n'est pas obligé d'attendre la fin de ces démarches au niveau européen, je prendrai le Danemark Le Danemark. Interdit certains pères face depuis 2020 il y a me semble-t-il, au-delà de la surveillance des mesures coercitives à prendre. Merci. La parole est à d'notre collègue Bruno Sido. Pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre vous vanter les mérites de l'apprentissage et vous avez raison. À ce titre vous inciter les collectivités territoriales à recruter plus de jeunes et à les former mais sans moyens financiers de la part de l'État, elles ne pourront pas y parvenir. En effet, depuis la loi du 6 août 2019, le Centre national de la fonction publique territoriale. Et les représentants des employeurs territoriaux cherche un accord de financement pérenne. Nouveau système de financement que nous avons voté dans le lot finances pour 2022 prévoit une taxe d'apprentissage de 0,1% pour les employeurs territoriaux en contrepartie de quoi l'État et France compétences finance à hauteur de 15 millions d'euros chacun et le Cnfpt à hauteur de 13 millions et après avoir menacé de vous retirer sous la pression des employeurs locaux. Vous avez accepté de maintenir pour 3 années supplémentaires. La contribution de l'État aux frais de formation des apprentis en collectivité mais voilà que par une circulaire du 10 mai dernier vous actez unilatéralement le désengagement de France compétences dès 2024, passant de 15 millions en 2023, 5 millions en 2025 avant extinction complète de la participation. Une réelle dynamique s'est engagé pour l'apprentissage, passant de 8000 contrats en 2020 à 12.000 en 2022 et pour 2023 18.000. On atteint les 18.000 ce qui représente un engagement financier de plus de 160 millions d'euros. Ce n'est pas tenable financièrement alors même que les recettes perçues sont de 75 millions d'euros par le Cnfpt il manque près de 87 millions d'euros dans la même circulaire du 10 mai dernier, vous demandez aux employeurs locaux de faire plus tout en vous désengageant alors madame, la Première ministre, que comptez-vous faire pour pérenniser le développement de l'apprentissage dans les collectivités. Oh vous répondent, la parole est à la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales. Madame la Ministre, devait la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Sido l'encouragement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales est au coeur de nos priorités pour 2 raisons. Il permet aux collectivités d'attirer des jeunes talents et il permet aux jeunes de se confronter à une palette de métiers au service de l'intérêt général dans les territoires pour leur permettre d'acquérir de solides compétences c'est un tremplin pour l'emploi. Une chance pour les collectivités. Cet effort passe par un maintien de notre engagement financier dans les collectivités territoriales dans les années à venir, à hauteur de 15 millions d'euros pour les apprentis recrutés en 2023 en 2024 et en 2025 comme cela a été pris précédemment prévus pour 2022 comme vous l'avez indiqué la Première ministre, il a inscrit dans sa circulaire du 10 mars 2023 relative au renforcement du recrutement d'apprentis dans la fonction publique afin d'atteindre l'objectif fixé par le président de la République de recrutement d'un million d'apprentis d'ici la fin du quinquennat. Ces 12.000 apprentis en 2022 et probablement moins autant. Qui rejoindront nos collectivités locales en 2023, cet engagement de l'État à hauteur de 45 millions d'euros sur 3 ans permettra de développer le recrutement d'apprentis dans nos collectivités territoriales, nous sommes d'ailleurs sur le point de finaliser la convention qui lie l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale. Nous devons également lever les blocages statutaires qui empêche les collectivités qui le souhaitent de recruter durablement leurs apprentis, nous voulons faire de l'apprentissage, une voie de recrutement pérenne pour les collectivités locales car nous voulons éviter qu'elle se sépare des apprentis au bout de deux ans, c'est l'un des axes du chantier. Parcours rémunération menée par Stanislas Guerini Ministre de la Transformation et de la fonction publique qui permettra de faire de l'apprentissage, une voie de prérecrutement une réelle modalités de recrutement dans la fonction publique territoriale. Je vous remercie. madame la Ministre vous souvent se dit à l'apprentissage dans le privé avec de l'argent public à hauteur de 6 milliards d'euros par an. Un apprenti de public est-il à ce point moins méritants qui ne nécessite n'hésite pas le même effort national en termes budgétaires est une énième façon de faire peser sur les collectivités territoriales, une charge de plus. Merci. La parole est à notre collègue daphné Ract-Madoux pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le président, madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de la transformation et de la fonction publique. Vous venez d'annoncer une augmentation du point d'indice de la fonction publique de 1,5% applicable au 1er juillet prochain ainsi que des mesures complémentaires prime facultative, augmentation du nombre de points. Pour les agents de catégorie B et C, en 2024. Dans le contexte de forte inflation que nous connaissons, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cette augmentation constituera un coup de pouce dont les agents publics ont le plus grand besoin pour soutenir leur pouvoir d'achat. Cette annonce intervient cependant à une époque de l'année où les Budgets des communes ont déjà été voté des Budgets déjà contraint et avec parfois des augmentations d'impôts décidées pour faire face et continuer d'investir. Certaines communes n'ont eu communication de la part de leur fournisseur d'énergie du montant de leur facture d'électricité du premier trimestre qu'après le vote de leur budget avec parfois des augmentations substantielles dans mon département, même avec les boucliers tarifaires, elles peuvent être de l'Ordre de 40%. En un mot, nos villes et nos villages surtout non plus ni marge budgétaire ni perspective. Dans ces conditions, on le sait sans Z, c'est l'équilibre des Budgets qui est remis en cause et va compromettre leur investissement et leur projet. Faute de moyens d'amorce de ces projets. Les collectivités de mots ne pourront prétendre aux aides DETR déciles fonds verts ou autres subventions, les élus ont le sentiment qu'on reprend, d'un côté ce que l'on donne de l'autre. Monsieur le ministre, ma question est donc simple, l'augmentation du point d'indice de la fonction publique étant une décision d'État, l'état va-t-il compenser comme cela a été fait, même partiellement dans la loi de finances rectificative en août 2022. Enfin, comment avez-vous et allez-vous consulter les associations d'élus, ces élus qui sont encore et toujours en première ligne dans nos territoires. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Ract-Madoux. Vous poser plusieurs questions. Est ce que nous avons concerté avec les associations d'élus. La réponse est oui. Je les ai réuni, le 23 mai dernier. Je les ai réunis à nouveau avec ma collègue Dominique Faure, le 12 juin, avant de recevoir les organisations syndicales et de procéder à un certain nombre d'annonces. Une question, c'est ce que nous avons tenu compte de ce que nous on dit les associés de ce genre d'élus et la réponse à nouveau c'est oui. Elles nous ont dit 3 choses. Le 23 mai. Hein. Que l'effort hein. DCR c'est-à-dire contraints, pour les collectivités, soit le plus modérée possible Que nous concentrions nos efforts sur les plus bas salaires. Vous le savez la fonction publique territoriale, c'est trois quarts de catégorie C trois que cet effort indiciaire puisse être lissée dans le temps et précisément les annonces que j'ai au nom du gouvernement avec l'arbitrage après un ministre est plus porté répondre à ces 3 points. L'année dernière c'était trois et demi, pour 100 d'augmentation du point d'indice en cours d'année, un et demi. Vous l'avez mentionné. De nous utilisons l'enveloppe budgétaire de façon très différente pour la concentrer sur les plus bas salaires. C'est précisément ce que nous demandaient les associations d'élus cet effort budgétaire. Oui, il sera lissé dans le temps puisque une partie de l'effort porte sur 2023 c'est l'augmentation du point d'indice, l'autre partie, c'est la distribution de points indifférencié à toute la gris interviendra en janvier 2024, donc avec une prévisibilité plus forte, je me permets d'ajouter une question supplémentaire peut être la seule qui vaille. Si les collectivités avaient été seul décisionnaire. Que elle soit seule en maîtrise du point d'indice. Quelle décision aurait-elle prise avec une année où nous revivons à nouveau 6% d'inflation, avec une année où l'inflation alimentaire est importante. Quelle décision a-t-elle prise je crois très sincèrement, madame la sénatrice qu'elles auraient pris précisément la même décision que nous avons annoncé. Madame Ract-Madoux. Bien, nous en avons terminé avec les questions au gouvernement. Merci madame, la Première ministre. Mesdames, et messieurs les Ministres nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mercredi 21 juin à 15h je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Bonjour monsieur le Ministre, mes chers collègues par lettre en tête. De ce jour, le gouvernement demande en application de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution que la suite éventuelle de l'examen en 2ème lecture de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite soit inscrite à l'ordre du jour à l'issue du présent espace réservé éventuellement ce soir acte est donné de cette demande. Par lettre en date de ce jour, la commission de la culture de l'éducation et de la communication et la commission des Lois demandent au Sénat en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires de leur conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour une durée de 6 mois pour mener une mission conjointe de contrôle afin d'examiner la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes. La conférence des présidents examinera sa demande lors de sa réunion de ce jour. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie présenté par Monsieur François Patriat et plusieurs de ses collègues demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans la discussion générale. La parole est à monsieur François Patriat, auteur de la proposition de loi. Monsieur le président vous avez 10 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure mes, mes chers collègues. Nous savons combien à être maire est une mission difficile, exigeante, parfois ingrate et combien exaltante, mission accomplie avec humanisme par des femmes et des hommes qui oeuvre avec passion dans leur territoire et dévouement pour leurs concitoyens. Dans l'ombre de ses élus oeuvre avec tout autant d'engagement une garde rapprochée entièrement dévouée au maire et qui les emploie, ces hommes mais surtout ces femmes à 94% ce sont les secrétaires de mairie maillon incontournable de la vie commune. Juristes urbanistes comptable, informaticienne les secrétaire de mairie en fonction dans les communes de moins de 3500 habitants sont essentiels à la fois pour les habitants pour qu'ils représentent le 1er service public de proximité et pour le maire pour qui sont le principal et parfois l'unique collaborateur. Très polyvalent avec un sens aigu du service public, ils exercent une fonction d'appuyer administratifs techniques et juridiques auprès du maire et des élus dans tous les domaines d'intervention municipale, accueil du public et de démarches administratives médiation entre les citoyens et l'administration conseille aux maires et aux élus municipaux avec l'élaboration du budget en charge de comptabilité, de la commande publique dossiers de subvention de l'urbanisme, du droit funéraire de l'état civil de l'organisation des élections du fonctionnement de la commune et les instances d'ici les agents techniques et de travaux et véritable cheville ouvrière de la vie communale garant du respect des règles légales et réglementaires dans tous les domaines de compétence des municipalités. Ces agents doivent en outre se tenir informé de toutes les évolutions normatives concernant les collectivités territoriales. En plus d'être les piliers administratifs de nos municipalités leur rôle va bien au-delà car ils sont garants de la bonne gestion des affaires publiques, municipales. Ils sont aussi les gardiens de la démocratie locale. Facilitateur du dialogue entre les élus, les citoyens qu'il joue un rôle crucial dans la diffusion de l'information municipale dans la mise en place des dispositifs de participation citoyenne et de la résolution des problèmes rencontrés par les habitants de nos communes. Leur disponibilité et leur sens de l'écoute, contribue à renforcer la confiance entre l'administration et les citoyens. Ces agents joue incontestablement un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de nos collectivités locales et leur contribution ne doivent pas être sous-estimé. Pourtant. Derrière la gratitude unanime de leurs élus. Les secrétaires de mairie sont confrontés à des conditions de travail difficiles à l'isolement et une reconnaissance insuffisante les rémunérations sont plus attractive ne reflétant pas la complexité et la diversité de leurs missions. Les possibilités de formation sont limités et surtout les perspectives de carrière sont quasi existant Aujourd'hui. Près de 2000 postes restent vacants et ce ne sont pas moins et ce ne sont pas moins que 8000 à 10.000 postes qui devrait être renouvelée d'ici 2030. Les secrétaires de mairie mérite donc une plus grande reconnaissance de leur contribution précieuse à la gouvernance locale au Sénat. Cette impérieuse nécessité de valoriser ce métier a fait l'objet d'un large consensus politique comme l'a montré le 6 avril dernier l'adoption à l'unanimité par le Sénat d'une proposition de loi initiée par notre collègue 6 Céline Brulin, il connaissait les collègues du groupe communiste républicain et citoyen écologiste visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Naturellement je ne manquerai pas aussi de saluer ici le travail approfondi de la délégation aux collectivités territoriales et le rapport de nos collègues, Catherine Di Folco, Cédric Vial et Jérôme Durain sur l'attractivité du métier et leurs propositions pour faire de la fonction de secrétaire de mairie un véritable métier nous travaillons ensemble à, à renforcer leur statut et à leur fournir des outils pour monter en compétences afin d'accomplir des missions avec succès. C'est l'objet du texte que nous vous proposons la présente, proposition de loi vise d'une part à répondre à ce besoin de renforcement des compétences tout en veillant à conserver un large vivier de candidats et d'autre part à reconnaître l'expérience des agents de catégorie C exerçant d'ores et déjà c'est fonction. À cet égard l'Arctique le 1er permet de créer une voie de promotion interne dérogatoire en dehors des quotas pour les agents de catégorie C, qui exerce la fonction de secrétaire de mairie afin de leur permettent par le biais d'un processus de reconnaissance des acquis de l'expérience simplifiée d'être nommé à la catégorie B, il s'agit d'ici d'une forme de robes de plan de requalification qui s'adresse au secrétaire de mairie actuellement en fonction. L'article 2 s'intéresse quant à lui au futur secrétaire de mairie en prévoyant une formation qualifiante initiale de façon à permettre aux à un agent de catégorie C, quel que soit son Cadre d'emplois au sa filière ce qui permettra d'élargir le vivier faisant fonction secrétariat de mairie ou occupant d'autres fonctions mais souhaitant accéder à celle-ci d'exercer ses fonctions et à ce titre d'être promu en catégorie B en ayant validé des compétences spécifiques et enfin l'article 3, reconnaît la spécificité du métier de secrétaire de mairie en offrant aux agents qui l'exerce le bénéfice d'avancement de carrière accéléré au profit de la poursuite de leur parcours professionnel au sein de la commune qui les emploie et dans d'autres collectivités par exemple sur des postes de directeur général des services dans les communes de plus de 1000 habitants. Cette proposition de loi se veut être une réponse à la problématique des secrétaires de mairie qui devrait être complétée, à la fois par des actes réglementaires. Monsieur le Ministre, mais aussi par des échanges de bonnes pratiques en matière de partage de fonction entre différentes communes d'utilisation de logiciels d'accès de contenus à la formation continue de remplacement en cas d'absence de recours au régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel en leur offrant la garantie d'une rémunération juste. Et équitable par rapport à la réalité de leur travail en soutenant leur développement professionnel nous renforçons leur compétence et leur capacité à servir efficacement les maires et leurs concitoyens en leur accordant une meilleure reconnaissance des conditions de travail améliorées et les perspectives d'évolution professionnelle. Nous investissons dans la qualité des services publics locaux reconnaître leur expérience et récompenser leur expertise permettront de maintenir une motivation élevée et d'attirer de nouveaux talents dans ce secteur crucial mais attention c'est un enjeu d'avenir pour la ruralité. Je vous appelle donc mes chers collègues à soutenir ces ces mesures et à oeuvrer ensemble pour une véritable valorisation des secrétaires de mairie. Je vous remercie. Merci. Collègue, la parole est à présent à Madame, Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois et vous avez 10 minutes Madame la rapporteure. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues. 10 semaines après l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi de Céline Brulin, et ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Nous examinons un nouveau texte visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie déposer cette fois-ci par monsieur François Patriat, ses collègues du groupe. Rassemblement démocrates, progressistes et indépendants et des collègues d'autres groupes. Les textes se suivent et ne se ressemblent pas. Toutefois, et contrairement à la proposition de loi précédente. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée, le 1er juin. Nous pouvons sans aucun doute y voir le signe de sa volonté que ce texte aboutisse, bien évidemment, nous saluons ce volontarisme, même si nous déplorons également qui ne soit pas allé de même sur la proposition de loi du groupe CRCE que je remercie une fois encore d'avoir initié le processus de réflexion et d'action sur cette problématique. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est que des mesures concrètes soient rapidement prises pour répondre aux besoins légitimes de reconnaissance des agents qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie et remédier au manque d'attractivité dans ce métier souffre aujourd'hui sans quoi la pénurie de secrétaire de mairie à laquelle font face aujourd'hui la quasi-totalité des maires des communes de moins de 1000 habitants ne pourra que s'aggraver et une fine et ce sera le bon fonctionnement de ces communes qui sera compromis et la qualité des services publics qui en pâtira. La commission des lois partage donc pleinement la visée de la propre la présente, proposition de loi de revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Elle souscrit en particulier, l'objectif de favoriser l'accès à la catégorie B. Pour des agents qui, parmi les secrétaires de mairie relèvent de la catégorie C, la proposition de loi entend favoriser cet accès par le biais de de nouvelles voies de promotion interne. La première dérogeant à la règle des quotas expirait au 31 décembre 2028, tandis que la 2ème reposant sur la validité d'une formation qualifiante serait pérenne. C'est une évidence, il est grand temps de mettre en adéquation les compétences multiples et exigeante qui sont attendus des secrétaires de mairie et les responsabilités importantes qui leur sont confiées avec le niveau de catégorie hiérarchique reconnu en conséquence, il convient de consacrer l'emploi de secrétaire de mairie comme un emploi de catégorie B au moins j'insiste vraiment, Monsieur le Ministre, sur ce sujet. Pour ce faire, la priorité est de mettre de permettre aux agents de catégorie C qui sont aujourd'hui en poste d'accéder à la catégorie B qui sera déterminé par décret en pratique ce réviser les secrétaires de mairie de catégorie C qui ont tant qu'ils sont 20 ou 25 ans qui n'ont pas la possibilité de passer les concours et à qui les règles de la promotion interne de droit commun ne permettent pas non plus de passer en catégorie B un délai d'environ 5 ans leur serait offert pour bénéficier de cette voie dérogatoire de promotion interne. C'est donc l'objectif de l'article 1er dans sa rédaction issue des travaux de la commission. La 2ème étape et de permettre aux agents de catégorie C, en poste depuis une durée moindre d'accéder également à la catégorie B à la condition, cette fois-ci d'avoir validé une formation qualifiante. Cette nouvelle moi de promotion interne est proposée par l'article de telle que modifiée par la commission. En commission, nous avions jugé nécessaire de lever l'ambiguïté qui affectait la rédaction de l'article 2 et avions donc réservé au secrétaire mérite déjà en poste. La voie de la promotion interne par la formation qualifiante. Notre objectif était de ne pas accroître pour l'avenir. Le nombre de secrétaires de mairie de catégorie C cela nous semblait en contradiction avec la conviction selon laquelle l'emploi de secrétaire de mairie doit être réservé aux catégories B et à. La rédaction proposée par le gouvernement à l'article de nous sans toutefois adéquate en permettant aux agents qui serait nommés à un emploi de secrétaire de mairie entre la promulgation de la loi et le 31 décembre 2028, de bénéficier de la promotion interne via la formation qualifiante. Cette date du 31 décembre 2028 est importante, elle doit marquer, selon nous, la fin de la possibilité pour les maires de nommer aux employes de secrétaire de mairie. Un agent de catégorie C débutera ainsi une nouvelle dynamique de recrutement et pour les secrétaires de mairie la consécration pleine et entière de leur emploi que mon emploi de catégorie B. Bien évidemment ce tournant fondamental nécessitera une mesure réglementaire, à savoir la modification du statut particulier du Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Nous serons par conséquent particulièrement attentif à ce que le gouvernement procède à cette modification sans elle la présente, proposition de loi manquera son objectif essentiel. Par ailleurs, la commission a souhaité renforcer l'identification des fonctions de secrétaire de mairie et pour cela, consacré de manière innovante, l'exercice de telles fonction dans le code général des collectivités territoriales, ces dispositions pourra, je le crois, contribué à la meilleure reconnaissance de ses agents en levant les ambiguïtés qui peuvent exister aujourd'hui. enfin nous devons tirer parti de la succession, à quelques semaines d'intervalle de 2 textes pourtant sur le même sujet. Pour enrichir le texte que nous dont nous discutons aujourd'hui par les dispositions votées à l'unanimité en avril. Afin d'accroître l'ambition de la présente, proposition de loi, la commission a donc repris les mesures relatives à la formation à la promotion interne et à l'emploi de contractuels. Tout d'abord, la Commission a souhaité conforter la formation des secrétaires de mairie qui est essentielle au regard de la variété des missions exercées de la technicité des compétences requises. L'article 2 bis introduit ainsi une formation initiale obligatoire propre à ses agents. L'objectif est que chaque secrétaire de mairie dispose dès sa prise de poste, des outils adaptés pour exercer ses missions. Nous savons en effet combien une fois en poste, il devient difficile au secrétaire de mairie de suivre des formations, même de quelques jours seulement par manque de temps éloignement géographique du lieu de formation et surtout en raison de la quasi-impossibilité à se faire remplacer en leur absence. Ensuite parce qu'il est nécessaire d'améliorer les perspectives d'évolution de carrière de l'ensemble des secrétaires de mairie, quelle que soit leur Cadre d'emploi l'article de terre vise à favoriser de façon pérenne, aussi bien à la promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie C pour leur accès la catégorie B que celle des secrétaires de mairie de catégorie B pour leur accès à la catégorie A, il nous semble en effet important de ne pas oublier des agents de catégorie B qui exerce aussi depuis de nombreuses années et qui n'ont pas la possibilité de passer un concours pour accéder à la catégorie A. Enfin, la commission a jugé nécessaire de compléter les dispositions visant à renforcer l'attractivité de l'emploi de secrétaire de mairie par une mesure visant à donner aux employeurs locaux davantage de souplesse ainsi l'article IV permet aux communes comptant. Entre 1000 et 2000 habitants. Le recruter des agents contractuels à temps complet aux employes de secrétaire de mairie, sachant qu'aujourd'hui, elles peuvent déjà le faire pour des emplois à temps non complet. Donc, la commission des lois vous propose d'adopter cette proposition de loi ainsi modifiée. Alors nous reconnaissons tous qu'elle ne pourra pas remédier à elle seule au manque d'attractivité dont souffrent ce métier ni répondre aux besoins criants de reconnaissance de milieu d'agents Je suis néanmoins convaincu qu'en faisant de l'emploi de secrétaire de mairie un emploi de catégorie B, nous enverrons un signal fort à la fois aux agents et aux maires et que nous amorceront une véritable revalorisation de ce métier indispensable à nos communes et nos concitoyens. Chers collègues, à deux mois d'écart, le Sénat a pris ce sujet à bras le corps. J'espère qu'il s'exprimera tout à l'heure avec la même belle unanimité que le 6 avril dernier. Il revient désormais au gouvernement, non seulement de veiller à ce que ce texte acquiert force de loi, mais également de travailler sans plus attendre à ces évolutions concrètes. Pour ce faire, il pourra s'appuyer sur le travail réalisé par les rapporteurs de la mission d'information sur l'attractivité du métier de secrétaire de mairie initiée par la délégation aux collectivités territoriales. Avec mes collègues Cédric Vial Jérôme Durain. Nous avons formulé un certain nombre de propositions très précises qui relèvent du domaine réglementaire, certaines pouvant être mises en application sans trop tarder, d'autres de nature législative seront présentées par amendement tout à l'heure. Au-delà de la question relative à la catégorie hiérarchique à la formation, ce sont les règles relatives, la rémunération des secrétaires de mairie qui doivent être revus. Plus largement, c'est l'ensemble des grilles indiciaires de la fonction publique territoriale qui doit être réformé. La récente revalorisation de l'indice minimum de traitement Poursuivre, l'augmentation du SMIC a en effet accru encore un peu plus ce tassement des grilles indiciaires. Un tiers des agents des collectivités et désormais payés au SMIC. De même la refonte générale des règles d'avancement pour l'ensemble des fonctionnaires mériterait d'être menés à bien au plus vite. Alors Monsieur le Ministre, je vous le disais déjà le 6 avril, la balle est dans votre camp. Et merci de ne pas attendre un 3ème texte pour agir. Je vous remercie de votre attention. Merci cher collègue. La parole est à présent monsieur Stanislas Guerini Ministre de la Transformation et de la fonction publique. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure. Monsieur le président du groupe RDPI Monsieur Président Patriat mesdames et messieurs les sénatrice, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous y voilà. Nous avions pris date. Il y a 2 mois, lors du débat sur la proposition là que vous aviez porté madame la sénatrice Boulin avec votre groupe CRCE. Nous avions pris date pour avancer et je crois qu'on peut dire que nous honorons aujourd'hui un rendez-vous essentiel parce que c'est de ça dont il s'agit. Être au rendez vous d'un métier. Vous l'avez à nouveau rappelé qui est la Pierre angulaire de nos communes, celui de secrétaire de mairie rendez-vous de reconnaissance a rendez-vous de valorisation a rendez vous de promotion. Que nous avons pris avec les secrétaires de mairie. Nous avions partagé le 6 avril dernier, un constat clair. Ce constat. Je résume à grands traits, nous le connaissons un métier exercé à 94% par des femmes. Majoritairement à temps non complet. Majoritairement en catégorie C. Nous avions eu en avril dernier des débats. Je veux dire de grande qualité convergents je crois pour mieux reconnaître celles et ceux qui exerce ses fonctions primordiales auprès de nos concitoyens d'avions partager ensemble. Des pistes intéressantes pour renforcer l'attractivité de ce métier reconnaître la poly-compétence requise pour exercer ses tâches complexes qui relève réellement de la catégorie B, c'était je crois un point de consensus très clair de nos débats sa nécessité d'agir sur plusieurs directions d'abord une meilleure reconnaissance du métier. Des perspectives de constructions de carrière d'évolution de carrière qui soient renforcées et surtout. Aussi des rémunérations étoffer. Ces enjeux sont primordiaux. Je crois qu'il y a pas de débat et si. Nous devons valoriser les secrétaires de mairie, actuellement en poste. C'est une question de fidélisation mais aussi attirer attirer des profils pour ce métier, quand on sait qu'un tiers des secrétaires de mairie partiront à la retraite d'ici 2030. Alors après l'adoption à l'unanimité de la proposition de loi de madame la sénatrice brûle hein, je veux également saluer le travail précieux que la délégation aux collectivités territoriales a pu mener ces dernières semaines et ces derniers mois sous l'égide sous votre égide madame la présidente Gatel. Dans le cas du rapport d'information que vous avez porté avec madame la rapporteure de la messagerie. Folco Monsieur le sénateur Vial dont je veux saluer également les travaux et Monsieur le Sénateur, hein, vous avez je crois mener un travail précieux je veux à cet instant aussi salué l'initiative du président Patriat du groupe RDPI d'avoir porté ce texte ce qui nous rassemble aujourd'hui et je crois qu'il peut susciter une convergence de vues. Je veux saluer le travail que vous avez mené en commission, madame la rapporteure di Falco afin d'intégrer des. La commission des propositions qui étaient portés dans la PPL de la sénatrice brûle hein. Vous avez l'art de la synthèse madame la rapporteur, et je vous en remercie. En ce sens, le texte qui nous occupe aujourd'hui me semble faire consensus, vous l'avez compris, je suis favorable et je vous proposerai d'y apporter quelques dispositions complémentaires lors de nos débats. Je suis certain qu'on va pouvoir travailler dans le même esprit transpartisan. Que nous avions eu le 6 avril et je le dis sans détour, je souhaite que ce texte puisse cheminer être adopté le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la responsabilité d'engager au nom du gouvernement, la procédure accélérée. Au fond, cette proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. Elle me semble extrêmement importante. Tant pour les secrétaires de mairie pour ce qu'elle peut traduire de ce que nous voulons faire du statut de la fonction publique. Un formidable outil au bénéfice du développement des compétences des agents de la reconnaissance de leur engagement. La proposition de loi que vous avez déposé. Monsieur le Président Patriat. D'abord elle permet de mieux reconnaître les secrétaires de mairie. Je crois que c'est une priorité que nous partageons tous ceux passe, vous l'avez dit madame la rapporteure par l'inscription cette fonction dans le code général des collectivités territoriales et je vous remercie d'avoir porté cette disposition en commission, je la soutiens à tout point de vue cela passe également par la reconnaissance du niveau de ses fonctions. Je l'ai dit-elle correspondent à minima à la catégorie B, cela relève du domaine réglementaire, mais j'en prends l'engagement ici, vous m'avez appelé dans l'hémicycle de la traduire dans les textes correspondants et de le faire Cela passe également peut-être par une nouvelle dénomination avait été l'objet de nos débats. Moi j'ai pris un engagement de méthode qui était de respecter la parole d'abord des secrétaires de mairie. Toutes les parties prenantes, associations d'élus, le travail que vous avez menée également sur cette question pour pouvoir porter ce changement de dénomination. Il me semble qu'il y a une forme de consensus qui est en train de se dégager de jamais parfait mais il émerge en faveur du nom de secrétaire général de mairie. Moi je suis favorable au au terme et au nom de ce consensus que nous puissions inscrire dans la loi. Cette nouvelle. Dénomination donc d'abord la reconnaissance puis ensuite c'est faciliter l'accès. Au plus grand nombre. Lorsque les compétences sont au rendez-vous. Je me réjouis à ce type que vous aviez repris la disposition du texte de la sénatrice brûle hein pour permettre aux communes entre 1000 et 2000 habitants de pouvoir recruter directement des contractuels. J'ajoute un engagement, vous m'aviez appelé à cet engagement, je prends l'engagement avec ma collègue, Sylvie Retailleau. Ministre de l'enseignement supérieur de la recherche de travailler en lien avec les universités pour favoriser l'émergence de formation initiale de secrétaire de mairie, comme vous le proposez mesdames et messieurs les sénateurs dans la mission d'information de façon à démultiplier les candidats potentiels au concours de la catégorie B ou à ou en tant que contractuel. 3ème élément. Reconnaissance accès. Valorisation de la formation, je viens d'en parler pour la formation initiale. Je vais en parler pour la formation continue aujourd'hui bien souvent le fait de se former. Je le dis très directement. On n'a pas assez d'impact dans le parcours d'un agent public c'est à ça que nous devons répondre et je crois que cette proposition de loi pour les secrétaires de mairie nous apporte des leviers d'abord pour exercer les missions propres au métier de secrétaire de mairie et là encore je salue la réintégration que vous avez fait en commission de la disposition de la proposition de loi brûle hein pour imposer une formation obligatoire à la prise de fonction. Ensuite pour faciliter et encourager la promotion. Et c'est une nouveauté que propose ce texte de prévoir que les secrétaires de mairie qui exercent déjà ses fonctions qui auront suivi une formation de qualification puissent bénéficier d'une promotion hors quota de promotion pour passer en catégorie B, je crois que c'est une excellente disposition je veux aller plus loin. J'ai la conviction, je vous l'ai dit qu'il faut surtout pas fermer les viviers de recrutement. C'est la raison pour la cage présenterait un amendement pour offrir la possibilité dès la promulgation de la loi. Un agent de catégorie C. Qui serait par exemple, agent d'accueil dans un département qui souhaiteraient devenir secrétaire de mairie d'accéder à ces fonctions et de ce fait à la catégorie B grâce à la formation qualifiante dont je ne veux pas l'exclure. Ça va nous permettre dans les 5 prochaines années de constituer un vivier qui répond à la nécessaire qualification en baie de ce métier. Si vous adoptez cette proposition de loi. Ça sera la première fois que la formation permettra par la reconnaissance des compétences d'être une nouvelle voie de promotion un accélérateur dans une carrière et c'est la philosophie que j'entends porter pour réformer transformer notre fonction publique dans son ensemble. J'ai parlé de formation. Je veux aussi parler de promotion parce que ce texte porte des dispositions très importantes. J'ai pris l'engagement auprès des collectivités les employeurs territoriaux d'assouplir les dispositifs de promotion pour mieux reconnaître les agents et une fois encore nous retrouvons ici les grands principes pour les secrétaires dans ce texte de loi par les 2 dispositions de promotion qu'il propose. Par la formation. J'en ai parlé et par la mise en place sur ces prochaines années, d'un plan de requalification d'une VAE d'une validation des acquis de l'expérience dédié à nos secrétaires de mairie qui sera adapté au secrétaire de mairie et que nous définirons en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes. J'ai eu l'occasion d'en parler, d'en parler que le sénateur Vial notamment j'ai. Une réserve par rapport à un des dispositifs qui avait été discuté de prévoir un dispositif de même nature pour une promotion interne des secrétaires de mairie de catégorie B en catégorie A également hors quota, je trouve qu'elle est moins justifiée puisque ça correspondrait moins une logique de requalification ses missions pouvant correspondre soit à la catégorie B, soit la catégorie A. Comme j'avais pu vous l'indiquez, aussi je suis réservé sur un article celui qui était dans la PPL de Céline Brulin sur l'Arctique qui prévoirait un pourcentage de places dédiées au secrétaire mêlé à l'intérieur des quotas eux-mêmes au moment même et je l'ai dit, c'est mon objectif ou nous visons plutôt à assouplir les quotas de promotion. Enfin, il faut le dire clairement, la reconnaissance des secrétaires de mairie, ça passe aussi par leur rémunération. Le calibrage en catégorie B, c'est une voix pour apporter une rémunération supplémentaire un gain immédiat mais je souhaite que nous allions plus loin et je soutiens à ce titre l'amendement du président Patriat qui vise, oh la la promotion facilité à offrir des accélérateurs de carrière au sein de chaque grade. de chaque grade. Je crois qu'il faut consacrer la particularité de ce métier. Le niveau de responsabilité particulière mais je sais que c'est une philosophie que nous partageons. Au-delà de l'indiciaire. Je sais également ce qui peut être fait en matière indemnitaire je sais mesdames et messieurs les rapporteurs que vous étiez favorable à la création d'une prime de responsabilité dédié au secrétaire de mairie. Je partage le sens de cette demande. Ce métier, c'est un métier de responsabilité. Je crois et je l'ai dit que le dispositif juridique actuel permet déjà cela via le Rifseep dans la catégorie il est fait ce du Rifseep et je crois que si il est trop peu utilisé par les maires. Je propose que nous puissions y travailler ensemble avec les employeurs territoriaux pour prévoir le cadre d'une future charte d'engagement par exemple sur les critères les montants qui pourraient être utilisés afin de faire de cette. Il est fait ce secrétaire de mairie une véritable prime de responsabilité pour le secrétaire de mairie. Je veux pas être trop long, nous allons avoir des débats je veux conclure quand même en en en disant évidemment que nous allons continuer à agir ensemble de chacun dans ses responsabilités par la loi. Par le règlement, mais également par la mobilisation de l'ensemble des acteurs et j'assumerai là aussi mon rôle de ministre de la fonction publique demandé de prendre des engagements en matière indiciaire. C'est ce que je fais en soutenant ou en introduisant ces différents articles, les décrets je les travaillera avec les employeurs territoriaux et j'ai associerai évidemment les parlementaires on devra mobiliser l'ensemble des associations d'élus sur tous les leviers. Vous avez mentionné quelques-uns de formation notamment. Je crois qu'il faut développer des agents mentionne de la mutualisation, c'est une dimension extrêmement importante et un cadre juridique qui permet d'ores et déjà de faire beaucoup de choses avec des centres de gestion avec les intercommunalités. Mais il faut accompagner les différents acteurs pour permettre une meilleure mutualisation. Pour le secrétaire de mairie et puis la mise en réseau. Je crois que c'était un des éléments un des apports essentiels de votre travail, vous plaidez pour le développement des immersions du tutorat. J'ai su pleinement favorable je crois moi aussi à la force des rencontres au partage de pratique en proximité les secrétaires de mairie d'ailleurs Samson elles-mêmes saisie mais ce doit maintenant ça doit passer à l'échelle au fond grâce à l'animation des de gestion des interco et je m'engage. De mon côté a renforcé aussi des Liens avec le réseau France service alors Mesdames et messieurs les sénateurs, nous étions donnés rendez-vous ici, d'ici l'été, c'est l'engagement que j'avais pris en séance nous y sommes. Soyons à la hauteur de nos engagements et de ce texte ambitieux qui, je le crois, servira à l'attractivité et au fond l'efficacité de nos services publics. Merci Monsieur le Ministre, dans la suite de la discussion générale. La parole est à monsieur Guy Bénard Roche du groupe des écologistes et vous avez quatre minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure collègue. Alors où le fait politique n'est plus compris l'élue de proximité demeure les l'élu préféré des Français, nous le disons tous. Action concrète du maire au plus proche du quotidien de nos concitoyens à l'écoute permanente auprès des administrés qu'les plus solides qui perdure, alors que beaucoup. Trop de Français sont perdus dans le, comment ça marche d'un mille-feuille territorial dont ils se demandent la fonction et parfois la légitimité. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui porte sur des rouages clés du fonctionnement de cet échelon local si essentiel le poste de secrétaire de mairie. Aussi sérieux essentiel que soit le sujet dans le groupe regrette toutefois un peu la manoeuvre ayant conduit à cette nouvelle PPL le Sénat dans son ensemble et dans la diversité de ces groupes est très attentif à la question du bon fonctionnement de l'échelon local. Cette préoccupation est telle que nous avons pu sur ces morts il y a à peine plus d'un mois, le 6 avril déjà débattent du sujet préoccupant de la revalorisation des secrétaires de mairie grâce à un texte de nos collègues communistes adopté à l'unanimité. Nous paraît un peu dommage que la majorité présidentielle, qu'elle soit parlementaire ou gouvernementale n'est pas trouvé utile d'exprimer ses positions et de proposer ses solutions sous forme d'amendement à ce moment opportun qui était un réel temps de débat parlementaire et démocratique. Vouloir espérer à juste titre, arriver à un compromis bénéfique pour l'ensemble du pays devrait être le seul moteur de notre action. Refusé en quelque sorte que ceci passe par une loi soutenue par quelqu'un d'autre que sa majorité ne nous paraît pas être forcément. Gage de bonnes intentions. Toujours est-il que du Chablais. Avec ce nouveau texte et une nouvelle chance de répondre aux attentes légitimes de nos territoires. Je salue le sérieux de notre commission qui a donc réintroduit les dispositions déjà voté en avril dans le texte que nous étudions aujourd'hui pour ce poste de secrétaire de mairie. Je profite du temps de cette discussion générale pour saluer le dévouement de ces personnes véritable clé de voûte de l'échelon local dans l'appui juridique, administratif, technique particulièrement lors de la préparation du budget permet le bon fonctionnement de nos communes de leurs actions et le déroulement de leurs actions et des politiques locales. Véritable outil d'interface entre les élus et l'administration et les citoyens. Ce poste remplis par des femmes en très grande majorité ne bénéficient pas d'un cadre ou statut à la hauteur d'une mission qui lui sont dévolus. Ce manque de reconnaissance de ce métier pourrait amener à des difficultés de recrutement dans les prochaines années qui existe déjà d'ailleurs au vu des 2000 postes vacants. L'urgence d'agir en faveur de la revalorisation de ses fonctions, hé bien la la contractualisation à plus grande échelle, nous pose toujours un problème vous le savez. Comme les 2 tiers de ses personnels exercent à temps partiel et que près Dakar travaille sur plusieurs communes, nous aurions préféré voir une réflexion de mutualisation éventuelle au niveau intercommunal pour partager le personnel entre les communes. Pour autant, notant le constat pas fraisiers la volonté commune de sécuriser au mieux le fonctionnement des maires des mairies, pardon, il y a la pérennisation et la valorisation de secrétaire de mairie la pérennisation la visibilité dans les perspectives de carrière dans le de formation de ces postes particuliers sans la clé de voûte de la consolidation et de la reconnaissance de leur travail. Je salue également les travaux de la délégation aux collectivités territoriales qui a émis des recommandations très pertinente sur le sujet. Dans une réelle démarche transpartisane. Notre groupe a cosigné ses amendements en espérant voir concrétiser dans ce texte. Les travaux de la délégation aux collectivités territoriales. Notre groupe votera donc ce texte et à son tour appelle le gouvernement à se saisir en fait pleinement et rapidement de ces questions majeures des agents à qui nous devrions permettent plus que jamais de travailler dans des conditions dignes et convenables afin d'assurer un service public de qualité accessible pour tous. J'ai bien noté les engagements pris aujourd'hui par le ministre. Tout comme la commission l'avait fait il y a un mois nous encourageons le gouvernement a bien prendre en compte les rémunérations et parcours professionnel de ces personnes, dans le cas des travaux portant sur l'accès, les rémunérations et les parcours professionnels dans la fonction publique lancée le 1er février dernier par le ministre de notre formation et de la fonction plus. Merci la parole est à présent monsieur Alain Richard du groupe RDPI monsieur le président vous avez quatre minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues. À notre tour, nous souhaitons nous engager pour remédier. À un point faible de notre dispositif public que nous avons tous identifiés. Il nous a été largement présentée dans nos départements, nous avons voulu travailler sur la base de la première tentative de la première réflexion menée à l'initiative de nos amis communistes et Jacques un feu rappelle que lorsque nous avions voté ensemble. Pour cette proposition. C'était dans le contexte nous considérions qu'il y avait un certain nombre de perfectionnement ou de rectification aille faire c'est donc ce que nous souhaitons faire aujourd'hui et en nous inscrivant dans le même esprit transpartisan. Et je suis sûr que ceci sera partagée par tous ceux qui se tiendront ce ce ce travail avons, nous ne sommes pas mal consacré en particulier Didier Rambaud et moi et moi même au sein de notre groupe. Je veux aussi saluer la contribution. Qui va être exploité cet après-midi par de la de la délégation aux collectivités locales qui a également approfondi le dossier je dois tout particulièrement salué l'excellente contribution de notre rapporteur Madame Di Folco. Qui manifestent à nouveau son excellente connaissance de ses sujets d'administration et de fonction publique. Pour aller très vite. Notre souhait est que la loi consacre rapidement le classement général en catégorie B des secrétaires généraux de mairie puisque nous souhaitons que ce terme soit reconnu à l'avenir comme beaucoup de collègues. Nous souhaitons également et ça a été un point de discussion en commission que j'espère nous allons pouvoir. Surmonter. Que cette inculpés Gration en catégorie B bénéficie aussi à de nouveaux entrants. À condition. Venant de la fonction publique, venant de la catégorie C à condition qu'ils aient satisfait à une formation nous souhaitons également c'était un des points importants et nouveaux de notre proposition de loi leur garantir une progression de carrière liées aux contraintes et à la pression particulière que représente cette sanction du fait de la charge de responsabilité. Nous souhaitons enfin que la proposition de loi, la loi que nous allons je pense aider à aboutir. Englobe à la fois une obligation mais des possibilités réelles de formation puisqu'on voit bien que c'est à l'heure actuelle, un des angles morts de la situation des secrétaires de mairie pour lesquels il n'y a pas véritablement de qualification formellement reconnu et qui sont en difficulté. Malgré les efforts qu'il existe du Cnfpt. Et de ses délégations départementales mais pour accomplir les formations qui sont nécessaires dans leurs fonctions. Je voudrais, Monsieur le Ministre ajouté personnellement de sujets complémentaire complémentaire qui relève plutôt du règlement mais qui je crois répondent à des nécessités pour rendre le l'emploi attractif et et durablement attractif. C'est la possibilité pour les communes de consentir une aide au logement. Des secrétaires de mairie car beaucoup connaissent des un déplacement professionnel lors de leur de leur recrutement, qui suppose une aide de ce point de vue là également la possibilité pour les communes de consentir une aide aux transports car certaines de certains ou certaines de ces personnes classées en secrétariat général de de mairies peuvent avoir des déplacements à faire, notamment lorsqu'ils sont en service dans 2 voire 3 communes. Nous aurons besoin et. Vos premières annonces sont encourageantes. Monsieur le Ministre, nous aurons besoin du soutien du gouvernement en Direct. Pour les dispositions. Pour comment dire surmonter l'irrecevabilité financière des dispositions ouvrant à des charges financières pour les collectivités. Je voudrais aussi insister pour que vous prévoyez d'ici à la loi de finances un soutien particulier pour les plus petites de ces communes qui sont souvent avec des niveaux de ressources qui sont 100 ou 200.000 euros par an et pour lesquels cet effort peut être disproportionné. En tout cas, en tenant compte de leurs ressources. Nous avons donc besoin et nous comptons sur votre appui. Monsieur le Ministre, en particulier pour le passage à l'Assemblée nationale qui permettra que ceci devienne vraiment la loi. Merci, cher collègue, la parole est à présent Monsieur Hussein Bourgi du groupe socialiste pour six minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission des lois. Madame la rapporteure, mes chers collègues. Le 6 avril dernier nous débattions ici même de la proposition de loi de notre collègue Céline Brulin, et du groupe CRCE. Au sujet des secrétaires de mairie, de la nécessité de revaloriser ce métier. 2 mois plus tard, nous nous retrouverons à nouveau ici pour débattre de la proposition de loi de notre collègue le président François Patriat de son groupe. Toujours au sujet des secrétaires de mairie. Cela est suffisamment rare pour être relevé, j'y vois 2 options. La première hypothèse traduit l'expression de notre mauvaise conscience à l'égard des secrétaires de mairie dont nous plaisant a salué l'engagement et a embrassé la cause. La 2ème hypothèse traduit le constat d'un travail inachevé lorsque nous votions la proposition de loi de Céline Brulin, le 6 avril dernier. Je rassure tous mes collègues. Car si nous avons parfois mauvaise conscience aussi nous éprouvant le sentiment de travail inachevé. Ce n'est fort heureusement pas de notre responsabilité, c'est la faute de l'article 40 de la Constitution qui nous entrave nous contraint et nous limite dans la marge de manoeuvre budgétaire. Et législatives. C'est aussi la faute du gouvernement. Je m'en excuse. Monsieur le Ministre, car vous n'avez pas fait le choix le 6 avril dernier d'enrichir la proposition de loi de Céline Brulin, et je le regrette. Partant de ce constat, je ne peux que déplorer la position du gouvernement sur le sujet des secrétaires de mairie. Ou on leur témoigne de la sollicitude tout en adoptant une position d'attente ou plutôt une position des petits pas. À partir de votre intervention de ce jour. Alors Monsieur le Ministre, je vous le demande, très simplement. Quand comptez vous présenter un projet de loi transversale, un projet de loi digne de ce nom. Un projet de loi volontariste qui concerne tous les sujets qui intéressent secrétaire de mairie. Un projet de loi qui concerne aussi les moyens budgétaires alloués aux nécessaire évolution de ce métier. Ce 1er juin la délégation aux collectivités territoriales du Sénat a rendu des conclusions d'un rapport sur le métier de secrétaire de mairie. Je souhaite ici saluer le travail remarquable de mes collègues, Catherine Di Folco, Cédric Vial et Jérôme Durain et surtout attirer votre attention Monsieur le Ministre, sur les 17 propositions frappée de bon sens qu'ils ont formulées. Monsieur le ministre, il n'appartient qu'à vous de puiser dans cette boîte à idées que le Sénat verse au débat et met à votre disposition. Je suis certain que parmi ces 17 propositions, vous trouverez matière pour enrichir vos propres réflexions et vos propres travaux. Je forme le voeu que le débat de ce jour ne permettent d'avoir des réponses de votre part sur l'échéance sur le fameux projet de loi sur l'attractivité de la fonction publique que vous nous annoncez depuis tant de mois et je pense que votre réponse intéressera à la fois les sénateurs et sénatrices ici présents, mais les nombreux secrétaire de mairie qui nous suivent en ce moment même. Qui nous suivent à travers le site du Sénat et que je salue en effet il devient urgent de le faire car le métier de secrétaire de mérite un métier sous tension agent polyvalent à la fois rédacteur juristes fiscalistes trésorier urbaniste mais aussi parfois assistant social. Conseiller en informatique et en orientation scolaire. Le secrétaire de mairie représente bien souvent le 1er visage du service public municipal, un service public à visage humain qui n'oblige pas à prendre rendez vous ni à passer par une plateforme dématérialisée. Un service public au sens noble du terme accessible à toutes et à tous au quotidien les secrétaires de mairie permettent à nos villages de fonctionner en tant qu'entité administrative et politique au quotidien, ces dizaines de milliers de femmes et d'hommes concours à la mise en oeuvre des politiques publiques communales et à leur efficience, disons-le sans ambages, sans le secrétaire de mairie. Les communes notamment en milieu rural n'existerait plus. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous le savons tous. Le secrétaire de mairie aiment leur métier mais pour nombre d'entre eux pour nombre d'entre elles, leur métier est aujourd'hui synonyme de manque de reconnaissance de quête de sens d'isolement. Les auditions menées par Madame la rapporteure Catherine Di Folco, à l'occasion des 2 propositions de loi nous ont permis d'écouter et d'entendre des témoignages mettant en exergue un manque d'attractivité pour un métier pourtant indispensable. Les raisons sont nombreuses. Manque de statut propres métier précarité des contrats à temps partiel faible rémunération, cette réalité est en totale inadéquation avec la multiplicité des missions à accomplir et avec la complexité des tâches administratives réglementaires qui pèsent sur les collectivités sur les communes et les intercommunalités. Ce manque d'attractivité, a déjà des conséquences au 10 mars 2023, 1919 postes secrétaire de mairie était vacants en France et les petites communes sont hélas les plus touchés. Le texte que nous, nous les examinons aujourd'hui et qui aide-t-il à la hauteur des enjeux. Assurément non. Cette proposition de loi est nécessairement parcellaire. Ses auteurs ont fait avec les contraintes liées à l'article 40 que j'évoquais il y a quelques instants la rédaction issue des travaux en commission des lois à parmi a permis d'en améliorer dans bonifier la teneur. Je souhaite au nom de mon groupe saluer Catherine Di Folco notre rapporteur car ces apports immanquablement enrichi et la qualité. Les deux textes, celui de Céline Brulin, le 6 avril et celui de François Patriat aujourd'hui la présente, proposition de loi met l'accent tant sur la formation de secrétaire de mairie que sur l'évolution de carrière de levier essentiel pour relancer un peu l'attractivité de ce métier. Ces mesures sont bien nous y sont favorables. La rémunération reste pour l'heure l'angle mort de nos travaux alors que nos collectivités locales peinent à recruter. En effet, ne peuvent proposer des salaires aussi attrayant, qu'elle le souhaiterait. Il semble évident qu'un concours de l'État est nécessaire, particulièrement dans les petites communes du monde rural. Monsieur le Ministre, je me tourne vers vous. Vous avez la maîtrise de l'Ordre du jour à l'Assemblée nationale. J'ai un voeu juste un voeu à formuler. Est-ce que vous pouvez vous engager à ce que ce texte soit voté avant la fin de la session parlementaire afin que ces 2 propositions de loi aussi modeste soit-elle soit pleinement pleinement en vigueur dans les prochains mois qui viennent de secrétaire de mairie le demande et en le faisant vous feriez oeuvre utile. Nous comptons sur vous. Les secrétaires de mairie compte sur vos. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Céline Brulin, du groupe communiste. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il y a quelques mois en effet, notre petit mais efficace groupe CRCE vous présenter une proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie. Avec l'appui de notre rapporteur Catherine Di Folco et de son état d'esprit constructif, nous parvenions unanimement à poser une première Pierre modeste mais nécessaire en faveur de la reconnaissance de ces femmes car je le redis, ce sont à plus de 90% des femmes indispensable à la vie de nos petites communes. Le couple mère secrétaire de mairie et reconnu vécue comme le pilier de la vie de nos communes rurales bien plus sans doute que le couple mère préfet vanté durant la crise sanitaire. Ensemble, ils font vivre ces communes qui sont le premier mais parfois aussi le dernier des services publics dans nombre de nos territoires et qui à ce titre doivent faire face à des attentats, des besoins toujours plus grands, à mesure que l'État abandonne ses territoires lors de l'examen de notre texte. Sollicité par tous les bancs de cet hémicycle, vous. Monsieur le Ministre à poursuivre le le travail de manière transpartisane nous prenions même date pour que le projet de loi de finances 2024 permettent de concrétiser d'indispensables mesures salariales en guise de quoi nous voilà aujourd'hui devant une nouvelle proposition de loi portée par le groupe RDPI la proximité d'élections sénatoriales, il serait-elle pour quelque chose. Alors, nous qui sommes tant attachés à l'initiative parlementaire nous reconnaissons bien évidemment ce droit à chacun des groupes futile d'inspiration gouvernementale, mais nous pensions peut être un peu naïvement que cette nouvelle proposition de loi à laquelle j'imagine vous avez apporté une petite contribution Monsieur le Ministre permettrait d'aller beaucoup plus loin dans la reconnaissance des secrétaires de mairie. Nous pensions que des mesures d'ordre réglementaire, que vous avez le pouvoir de prendre des mesures d'ordre salarial notamment seraient mises à l'ordre du jour beaucoup plus rapidement. Nous pensions que le travail effectué par Cédric Vial Catherine Di Folco et Jérôme Durain au nom de notre délégation aux collectivités territoriales seraient mis à profit car au-delà de la légitime reconnaissance au secrétaire de mairie. Il faut lutter contre la pénurie que nous connaissons et qui risque de s'accroître, compte tenu du départ en retraite prochain même si vous en avait reculé l'âge d'un tiers d'entre elles d'ici 2030. Cette proposition de loi retravailler par la rapporteure va permettre d'accélérer la promotion interne des secrétaires de mairie aujourd'hui majoritairement catégorie C vers la catégorie B. c'est une bonne chose et nous ne mégote rompt pas notre soutien à cette mesure mais on pourrait imaginer si vous n'étiez pas si addict à l'article 40 que cela permette aussi à celles qui sont depuis de longue date en catégorie B de rejoindre la catégorie A, on pourrait imaginer un plan de déprécarisation de la profession la pénurie oblige à recruter des contractaient des contractuels pardon mais rien n'empêche de travailler à leur intégration au statut de la fonction publique territoriale. On pourrait imaginer que l'amélioration du sort des secrétaires de mairie guide l'amélioration globale de la situation des fonctionnaires notamment territoriaux, vous l'avez évoqué fort justement Madame la rapporteure, or vous ne proposez qu'un point et demi de revalorisation pour le point d'indice, ainsi que des primes non renouvelable, qui ne compte pas dans le calcul de la retraite. Mécontent de nouveau l'ensemble des organisations syndicales comme les associations d'élus pas associé à la démarche. Alors que les collectivités et leurs budget serré doivent concrétiser ces mesures, on pourrait imaginer par exemple lors de la présentation du programme francs sur ruralité. Des mesures de compensation à l'égard de ces communes qui leur permettrait précisément de faire oeuvre utile en en matière de salaire pour les secrétaires de mairie on est malheureusement encore loin de tout cela. Alors je ne doute pas que nous allons améliorer encore un peu les choses ici au Sénat mais ne considérez pas Monsieur le Ministre, que cela vaudra pour solde de tout compte. Bref, avec les pouvoirs dont vous disposez. Vous pouvez faire beaucoup mieux, je vous remercie. Si cher collègue, la parole est à présent à Madame. Françoise Gatel du groupe Union centriste. Vous avez six minutes, chers collègues. Madame madame la présidente. Monsieur le Ministre, monsieur le Président Madame la rapporteure mes, mes chers collègues, alors sans doute que les secrétaires de mairie sont une sorte de tube de l'été puisque nous y sommes depuis avril et que je souhaiterais vraiment comme mes collègues l'ont dit que nous aboutissions. Avant l'été. Si nous sommes aussi nombreux et aussi intéressés par ce sujet. C'est sûrement parce qu'il le veut bien et la paternité de l'ouvrage sera sans doute difficile à définir mais je veux saluer le travail excellent de Céline Brulin, et de ses collègues, le travail remarquable et très sérieux, rigoureux de notre rapporteur Catherine Di Folco et aussi naturellement le travail de mes collègues du trio Catherine Di Folco, Jérôme Durain et Cédric Vial qui ont fait un travail extrêmement intéressant intéressant remarquable et de grande qualité sur les secrétaires de mairie et puis je veux saluer tous les secrétaires ou toutes les secrétaires de mairie nous on connaît son beaucoup. Nous savons ce qu'est leur vie au quotidien et nous savons combien ils sont ou elles sont un peu plus que la cheville ouvrière de de l'action publique. Monsieur le ministre, il y a que vous que je n'ai pas salués. Donc je vais le faire mais très très franchement sans arrière-pensée mais un peu comme Madame brûle la fête sous la forme d'une notation de fin d'année. À un élève. Alors l'élève et bon il a appliqué. Peut mieux faire et doit accélérer. Il doit nous permettre de conclure en tout cas nous avons aujourd'hui dans notre pays 23.000 secrétaire de mairie, 1900 postes vacants et plus de 30% de ces personnes qui partiront en retraite à la fin de de de la décennie ce poste il est unique par sa responsabilité et j'ai eu l'occasion dans mon département de connaître la douleur d'une secrétaire de mairie et de son maire, quand le plan local d'urbanisme juste. On va dire, en voie de finition a été l'objet d'un recours qui a été positif parce que la secrétaire de mairie n'avait pas pu envoyer le fameux document officiel à la date prévue, il y avait un retard de 24h. Donc la responsabilité, elle est énorme et les secrétaires de mairie quelqu'un l'a dit parmi nous. Sont des frappes Drycan de possible quand les maires sont des inventeurs de possible et si nous n'avons pas de secrétaire de mairie monsieur Ministre nous n'aurons plus de mer. Et donc il faut effectivement pour ses secrétaires de mairie savoir les attirer les former les accompagner parce qu'elle travaille souvent dans une grande solitude. Il faut savoir les reconnaître quand nous parlons des secrétaires de mairie, nous parlons des communes et des mères. Alors nous ne cessons ici comme partout et j'en suis heureuse de déplorer d'être attristé par le désenchantement des mères alors nous compatissons nous saluons nous rendons hommage. Mais ça ne suffit pas et ce désenchantement des mères, il est dû à plusieurs causes dont je crois le fait de se retrouver trop souvent devant une complexité énorme sans l'appui d'une secrétaire de mairie qui est une sorte de de couteau suisse ce métier, on doit le considérer dans sa particularité et alors moi je suis déconcerté. J'ai un billet d'humeur si je puis dire sur l'Arctique 40. L'article 40, c'est un principe de précaution qui conduit au fait que nous n'allons pas encourager les maires. À faire des dépenses et que nous essayons d'être vertueux seulement l'Arctique 40 norme une norme une norme de précaution et aujourd'hui nous la transformons en objectif et à cause de l'article 40. Nous ne pouvons pas offrir un maire la possibilité de faire évoluer. Sa secrétaire de mairie du Cadre B et encadrera ça coûte pour un emploi à temps complet, 1800 euros par mois. Il y a d'autres verrous qui existe. Le principe de libre administration des collectivités et le principe. d'équilibre du budget de fonctionnement. Donc sincèrement je pense que si nous ne sommes pas capables tous ensemble de surmonter des carcans comme celui de la norme qui devient contreproductive. Je pense que nous ne servons pas. L'intérêt public et l'efficacité de de l'action publique c'est inexplicable auprès des des élus locaux. Donc Monsieur le Ministre, vous avez entendu ce soutien unanime et cette polyphonie extrêmement positive ce travail rigoureux qui a été fait moi je ne. Sous-estime pas eu je reconnais votre bonne foi et votre volonté mais là il faut vraiment conclure, il faut avancer, il faut savoir parfois, Monsieur le Ministre disruptif et se dégager des carcans normatifs. Et je pense que celui du statut de la fonction publique et trop normatif pour être équitable je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Stéphane Ravier du groupe des non inscrits.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le sens des responsabilités. Le service de proximité, la souplesse la fidélité. Voilà des qualités que tout employeur ça renchérit. Ce sont celles de la plupart des secrétaires. Riposte très poste en très grande majorité occupés par des femmes. Et pourtant à ce jour, cette fonction n'attire pas car sursollicité peu rémunérés et peu valorisé. Leur humilité silencieuse et les a trop longtemps confiné dans l'oubli du législateur, il est temps que ça change. Si les communes rurales sont la clé de l'équilibre des territoires. Les secrétaires de mairie sont la clé des communes rurales, plus la commune et rural, plus elles sont polyvalente est primordial bon fonctionnement local. Souvent seules, elles occupent notamment une fonction stratégique pour la gestion des opérations électorales. Elles sont les garantes de la vitalité démocratique de la France périphérique et donc le lien de confiance entre le peuple et le pouvoir entre les administrés et l'administration. Elles ont aussi la charge du bon déroulement des moments les plus importants de la vie des habitants puisqu'elles assistent l'officier d'état civil qui est le maire. Pour cela elle sacrifie de leur temps les samedis et dimanches, l'élargissement de leurs compétences, de manière générale. Des journées à rallonge qu'elles acceptent avec abnégation. Ces couteaux suisses à la française après leur métier sur le tas et s'adapte à la multiplication et à la complexification des normes. Ce sont les premières victimes à subir le harcèlement textuel évoquée par un récent rapport sénatorial et les injonctions contradictoires des différents codes. Elles ont aussi un rôle d'appui auprès du maire de son conseil municipal et des services qu'elle coordonne, sans le soutien des uns et le pivot entre les interlocuteurs. D'ailleurs les élus changent plus souvent que les secrétaire de mairie. Elles ont aussi un rôle de mémoire et de continuité des institutions communales. Ce guichet humain cette oreille désintéressé il y à l'écoute, ni le numérique, ni l'Intelligence artificielle ne pourront les remplacer. Aujourd'hui pourtant, il y a une pénurie de secrétaire de mairie et nous sommes appelés à trouver des réponses à la hauteur de l'enjeu. Il y a 2000 postes à pourvoir, c'est-à-dire 2000 communes en urgence vitale, plus la commune est petite, plus l'importance de la fonction est cruciale, là où tous les services publics ont disparu. Le secrétaire de mairie maintient une présence au service du public. Il y a ainsi un véritable enjeu d'avenir spécialement pour la ruralité. C'est pourquoi je soutiendrai ce texte et les amendements qui iront dans le sens d'une meilleure formation et d'une revalorisation salariale et statutaire. Je pense aussi qu'il est plus que temps que la loi s'adapte à l'évolution de leur fonction en requalifiant les agents de catégorie C, en catégorie B, je serai heureux de pouvoir voter avec vous une meilleure reconnaissance des secrétaires de mairie qui tienne notre nation debout en cimentant son socle communal de leur présence bienveillante. Merci la parole est à présent un autre collègue monsieur Éric. Du groupe RDSE. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, madame la rapporteure, chers collègues. Les problématiques de recrutement des secrétaires de mairie sans ça symptomatique des mutations de la fonction publique territoriale et du fonctionnement des collectivités. Le métier concentre à lui seul les difficultés de la territoriale disait d'ailleurs ma collègue Maryse Carrère lors de l'examen de la procédure de propositions de loi sur le sujet, en avril, le manque de formation. L'inflation normative. Les transferts de compétences aux intercommunalités la frustration des administrés face et des services publics dégradés. Tout cela participe à la fois aux 1300, démission de maire et aux 1900 postes de secrétaire de mairie vacants. Les deux étant naturellement lié car maire et secrétaire de mairie forme dans les plus petites communes, un binôme indissociable. Cette proposition de loi s'intéresse aux de difficultés principales de ce métier. Le manque de formation et le manque de reconnaissance. Là où le secrétaire de mairie est souvent décrit comme le couteau suisse qui est Paul Lemaire, malgré l'implantation des maison France Services, le secrétaire de mairie demeure une ressource indispensable la mairie étant le seul service public présent dans l'intégralité des communes au plus près des populations les plus fragiles. Cette polyvalence nécessite une formation plus musclée régulièrement actualisé, poursuivent les évolutions réglementaires. Pour l'heure les intercommunalités prennent le relais, notamment grâce au réseau des secrétaires de mairie qui permettent une constante une concertation entre agents d'un même territoire et une mise en commun des compétences. Cette proposition de loi vise donc à renforcer leur formation à la fois pour leur donner des clés supplémentaires dans l'exercice de leur métier mais aussi pour leur permettre d'évoluer plus vite. Pour la secrétaire de mairie de catégorie C des gens en poste. La proposition de loi prévoit de nouvelles voies de promotion interne pour un accès facilité à la catégorie B. Jusqu'à 2028 par un processus de reconnaissance des acquis de l'expérience simplifiée une dérogation de la règle des quotas. À compter de 2029 grâce à la validation d'une formation qualifiante. Nous proposerons sur ce point de revenir à la version initiale qui prévoyait une entrée en vigueur de cette mesure sans délai. Je solliciterai pour ma part un rapport au gouvernement sur l'opportunité de créer un BTS secrétaire de mairie une formation initiale et nationale axée sur la professionnalisation ce qu'une formation universitaire ne permet pas toujours. Des mesures qui nécessiteront toutefois de créer des conditions favorables à ces formations. Les pénuries de personnel et la multiplicité des employeurs peuvent en effet freiner les départs en formation avec la crainte d'une accumulation du travail difficile à rattraper. Lors du retour en poste mais la relance de l'attractivité de ce métier doit se faire car elle répond à un besoin impérieux sur nos territoires. Afin de soutenir les secrétaires de mairie exerçant dans plusieurs communes. Notre groupe avait déposé un amendement malheureusement déclaré recevables visant à mieux valoriser les agents multi-employeurs en zone rurale. Le cas est fréquent, est à l'origine de nombreuses désaffection du fait de la surcharge de travail, de la fatigue et des coûts supplémentaires liés aux transports. On l'a dit, 1900 postes sont aujourd'hui vacants et un tiers des secrétaires en poste cesseront leur activité dans les 8 prochaines années. En comptant les agents qui travaillent dans plusieurs mairies, ce sont des milliers de communes dont l'attractivité sera directement impacté. Nous devons donc envisager des mesures plus fortes de revalorisation spécifique. Pour conclure, le groupe RDSE soutiendra bien entendu cette proposition de loi qui traite d'un vrai sujet de préoccupation de nos élus locaux pour garantir le bon fonctionnement des communes mais aussi la qualité du service public, il est urgent de revaloriser ce métier en mutation et en tension. Cette initiative ne pourra toutefois pas exemptés. Le gouvernement d'un travail sur la revalorisation salariale et d'autres mesures non législative très attendu je vous. Merci, Merci, cher collègue, la parole est à présent hein Monsieur Cédric Vial du groupe Les Républicains et vous avez six minutes. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre. Monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues. Les secrétaires de mairie exerce des fonctions essentielles au bon fonctionnement des mairies de moins de 3500 habitants. Ils sont près de 23.000 à exercer ce beau métier en formant un binôme avec leur mère qu'ils assistent, conseille et accompagne. Ils sont également les garants de la continuité du service public sur les territoires où ils exercent. Il s'agit d'un métier complet, polyvalent et par dessus tout d'un métier qui a du sens. Pourtant il est depuis 2022, considéré comme le métier le plus en tension de la fonction publique territoriale. Près de 1000 postes sont actuellement vacants entre 8 et 10.000 postes devront être renouvelés d'ici 2030. Cette situation exceptionnelle nécessite un plan d'action rapide afin de répondre à cet enjeu majeur pour notre organisation territoriale, mais aussi pour répondre aux attentes légitimes des secrétaires de mairie et des mères de notre pays. C'est dans cet esprit que nous avons conduit une mission d'information avec mes collègues Jérôme Durain et Catherine Di Folco. Nous avons consulté les principaux acteurs nationaux et locaux concernés par cette profession nous avons étudié des initiatives innovantes mises en oeuvre localement et nous avons enfin proposer une vision d'avenir de ce métier, déclinées en 17 propositions pour le rendre plus lisibles, plus accessibles et plus attractif. Ce plan d'action forment un tout qui peut se présenter sous la forme de 5 axes, la formation en premier lieu. Deuxièmement, une meilleure reconnaissance du métier et des responsabilités afférentes. Troisièmement, des perspectives de carrière et d'évolution professionnelle. Quatrièmement un accompagnement durant l'exercice de leurs fonctions et cinquièmement par une communication pour plus d'attractivité de ce métier. Ce travail a été réalisé par le Sénat. Comme le Sénat, on a l'habitude dans un état d'esprit. De construction transpartisan. Il a par ailleurs il a d'ailleurs été approuvé à l'unanimité par les membres de la délégation aux collectivités présidé par Françoise Gatel, que je remercie sincèrement de son soutien précieux. La logique aurait voulu que ces propositions face ensuite l'objet d'une transcription législative. Mais Monsieur le Ministre. Première alerte, l'annonce d'une PPL préparée par vos services sans attendent le résultat de nos travaux est venue bouleverser cette logique et les bons usages plutôt que de s'en formaliser et bercé par vos affirmations de vouloir conduire également un travail collectif et transpartisan. Nous vous avons fait confiance et nous nous sommes adaptés. Pourtant 2ème, alerte le dépôt de cette PPL par notre collègue Patriat sans aucun échange préalable n'a pas permis qu'elle soit réellement pluraliste. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, nous jugeons tellement important d'aboutir que nous modifierons le texte en commission grâce au travail de de nos collègue Catherine Di Folco notre rapporteur. Le reste, fera l'objet de discussions avec vous Monsieur le Ministre, dans la perspective d'aboutir aujourd'hui en séance. Pourquoi se méfier. Vous nous avez tellement rassurée sur vos intentions d'aboutir à un résultat qui soit le fruit d'un travail collectif. Troisième Alerte lors de votre audition par les membres de notre délégation vous avez par exemple affirmé au sujet de la création de la prime de responsabilité qui est un élément majeur est central du nouveau système que nous vous proposons. Je suis favorable à ce que. Vous. Vous. Proposé mais il faudra étudier les modalités. Dont acte. Poursuivons donc et étudions ces modalités pour avancer. Pour nous, le plus important reste d'aboutir car l'attente est forte parmi les secrétaires de mairie et nous ne voulons pas décevoir. Alors voyons nous échangeons. L'échéance approche et seul le gouvernement détient la possibilité d'inscrire par amendement un certain nombre de dispositions auxquelles nous tenons. Pas de problème de droits d'auteur. Je vous propose de les déposer vous-même avec notre soutien ou d'autoriser leurs discussions lorsque votre seul accord. Suffit travail collectif transpartisan. Nous décidons de nous voir Monsieur le Ministre. Mon objectif est clair, comme la plupart de mes collègues je veux transposer le résultat de notre travail dans la loi pour que son examen ne devienne pas le rendez-vous désespoir déçu. Mais quel est le vôtre. Monsieur le ministre. L'objectif de cet échange informel et de traiter le sénateur Vial en lui confirmant votre intérêt pour son rapport d'information. Et tout en tenant une position globalement défavorable sur ces amendements C'est ainsi, Monsieur le Ministre, que sont décrites vos intentions dans le dossier préparé par vos collaborateurs que vous avez malencontreusement oubliés après votre départ. Plus loin, bien sûr, il est précisé mesure par mesure pourquoi ou comment vous vous y opposerait vous les éviterez. Sachant que nous nous enverrions aujourd'hui, je ne voulais pas renvoyer par la Poste mais évidemment je vous le rendrai à l'issue de mon intervention. En tous les cas, il ne reste aujourd'hui pas grand-chose de nos propositions. J'ai attendu jusqu'au dernier moment un geste de votre part sur certaines dispositions de nature législative et il n'est pas venu. Et maintenant je sais aussi par anticipation le sort que vous souhaitez réserver aux autres dispositions de nature réglementaire. Pour valoriser les secrétaires de mairie ou leur offrir des perspectives de carrière. Monsieur le Ministre, je regrette mais affirme à l'avance que cette PPL sera un nouveau rendez-vous manqué. La promesse d'un travail collaboratif et collectif s'est dissoute dans de petites sournoiserie. Comme le chantait Diane Tell. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours c'est chacun pour soi. Nous ne pouvions pas nous entendent, Monsieur le Ministre, nous avions des objectifs trop différents, nous voulions quelles que soient les conditions et la paternité des mesures faire aboutir un système d'organisation qui reconnaît mieux le métier de secrétaire de mairie Laurent plus attractif et permet d'anticiper le défi majeur du recrutement dans les prochaines années. Vous vouliez un texte avec le logo de la majorité sur ce sujet avant les élections sénatoriales pour faire semblant de l'avoir traité. Si vous étiez un homme d'État, vous sauriez qu'au Sénat ces choses-là ne se font pas. Je vous remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur. Pourquoi un texte spécifique pour les secrétaires de mairie avant tout parce que c'est un métier pas comme les autres. Vous devez savoir gérer un budget monter des dossiers, tu vention. Maîtriser le droit de l'urbanisme connaître. Un bon nombre de démarches administratives. Vous former aux nouveaux logiciels organiser des élections et bien souvent travaillé sur plusieurs mairies. Bref, les secrétaires de mairie sont de véritables couteaux suisses des agents tout-terrain de la fonction publique. Vous êtes avec le maire. La première porte à laquelle l'habitant vient frapper. Parfois pour des demandes très concrètes. Parfois pour recevoir des engueulades. Mais aussi pour gérer des situations personnelles compliqué. Et cela nécessite un vrai savoir-faire dans les relations humaines. Ce métier, il est passionnant ce qui le font le font avec coeur. Mais nous devons le constater il y a une réelle crise des vocations. Les maires, ça a été dit-on de plus en plus de mal à recruter. La pyramide des âges nous indique une secrétaire sur 3 cessera son activité au cours des 8 prochaines années. Nous oblige donc à proposer des solutions concrètes et c'est tout l'objet de ce texte. Cette proposition de loi, elle ne résout pas tout, mais en partie elle vise juste. Elle permet de déroger à la règle des quotas elle simplifie les parcours de carrière dans la fonction publique qui, on le sait sont tellement complexes et rigides. Ce texte permettra une meilleure reconnaissance des acquis et l'accession avec plus de souplesse à des grades supérieurs notamment je pense de la catégorie C à la catégorie B. Il facilitera le recrutement et permettra l'embauche de contractuels dans les communes jusqu'à 2000 habitants. Au sujet des formations. Il est nécessaire d'en proposer à celles et à ceux qui vont rentrer dans le métier. Néanmoins, soyons vigilants à ne pas les rendre obligatoire pour tout le monde. Et notamment pour ceux qui ont déjà plusieurs années d'expérience. La progression des carrières c'est une chose mais il faut également que ça se voit et que ça se traduise dans le salaire. Le gouvernement vient d'annoncer une hausse du point d'indice. Mais il faut d'urgence comme annoncé s'attaquer à la révision des grilles indiciaires de la fonction publique, nous le savons, à l'heure actuelle. Passer de la catégorie C au 1er échelon de la catégorie B ne change quasiment rien sur la fiche de paye. Il est également nécessaire d'accompagner les communes qui n'auraient pas la capacité d'organiser des formations de recruter et d'assumer des augmentations des progressions de carrière. Nous souhaitons qu'après le vote d'aujourd'hui le texte soit rapidement repris à l'Assemblée nationale et que la loi soit promulguée dans les délais les plus brefs. Au-delà du sujet de la carrière. Il y a aussi un découragement des secrétaires de mairie et des mères aussi d'ailleurs liés à la lourdeur. À la rigidité et parfois la nature des relations avec les services de l'État. Je pense notamment aux services de contrôle de légalité aux trésorerie au service de la DDT. L'État doit opérer une révolution en interne pour que ces services soient perçus comme un partenaire et non comme un adversaire des communes. Tous les élus du groupe cosignataires voteront ce texte important et salue cette initiative, je vous remercie de votre attention. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure l'a très bien décrit demain les secrétaires de mairie se feront plus rares. Ce qui est un comble pour nos mairies. Car parmi les nombreuses tâches qu'elles ont entre leurs mains. Nombre d'entre elles ne cesse de gagner en complexité. Je pense notamment à l'urbanisme ou aux marchés publics. Nous évoquons souvent sur ces bancs, l'importance du couple mère préfet pour appuyer de l'extérieur, nos communes. Mais le binôme mère secrétaire de mairie l'est tout autant constituant la colonne vertébrale des petites municipalités. Les auteurs de l'excellent rapport publié par la délégation aux collectivités territoriales ont souligné ce que nous observons dans nos départements. Compétence polyvalence et disponibilité à des agents nécessite de leur offrir en contrepartie un horizon professionnel des évolutions dans leur carrière, assorti d'une rémunération dynamique accompagnant leur implication. La lassitude et des professionnels d'aujourd'hui annonce la désaffection des candidats de demain. Il n'y a donc pas d'autre alternative que de rendre son attractivité à ce beau métier qui personnifie la première richesse de nos petites communes la proximité. aussi les dispositions que Madame la rapporteure a fait adopter pour tenir compte des compétences acquises dans la promotion des agents à la catégorie supérieure. Bé ou ah constitue une avancée salutaire. La rémunération est un facteur fondamental d'attractivité. Monsieur le Ministre et elle dépend de votre pouvoir réglementaire. Le salaire des secrétaires de mairie étant versée par les communes. L'État dans sa politique de dotation aux collectivités doit intégrer le fait que ces agents principalement des femmes incarnent souvent à elle seule le 1er échelon de l'administration. Et pour mener à bien leur mission, elle nécessite un effort de formation là aussi n'oublions pas que les problématiques inhérente à l'et ruralité demeure l'éloignement géographique complique également la participation physique aux enseignements. Pourquoi ne pas délivrer ses contenus à distance. Ceux-ci réglerait tant la question du déplacement que celle du nombre de places disponibles souvent trop réduit. Cette plus grande capacité, doit aller de Pair avec une augmentation du nombre de sessions proposées tout au long de l'année. Et pour permettre à l'indispensable tuilage, pourquoi ne pas proposer à certaines secrétaire. De consacrer entièrement leurs dernières années avant la retraite, à la formation. En plus de diffuser leur connaissance intime de la fonction. Elle pourrait également assurer un tutorat. Auprès de nouvelles recrues. Enfin, madame la rapporteure l'a rappelé lors de l'examen de ce texte en commission, la question de l'intitulé du poste fait encore débat principalement chez les premières concernées. L'idée de renommer le métier leur métier en secrétaire général de mairie, me paraît mieux correspondre aux réalités qu'ils recouvrent. Il participe aussi de l'attractivité de ce poste qui s'effectue d'une manne d'une manière transversale en oeuvrant autant à la préparation du budget qui a la gestion du personnel communal. Mais la défiance exprimée par certaines représentante syndicale se comprend sans amélioration substantielle des perspectives de carrière et de salaire. Les secrétaires de mairie ne prendront guère au sérieux nos belles formules de législateur. En se penchant sur cette question le Sénat rempli sa mission. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement qui doit montrer s'il est prêt à encourager et promouvoir des agents compétents et dévoués, en permettant l'adoption de certaines mesures concrètes, je vous remercie. Merci la discussion générale est Close. Madame Dominique Estrosi Sassone vous demandez la parole. Oui madame la présidente. Notre groupe demande 5 minutes de suspension de séance. Merci beaucoup. Monsieur le président de la commission des lois. Vous vouliez. Très bien. Je suis cependant que la séance pour cinq minutes. Merci.

Séance est reprise nous passons donc à la discussion du texte de la commission. D'abord des prises de parole à l'article 1er à. Cédric Vial. Vous avez demandé la parole, ne voit pas. Si Monsieur Vial.

on a besoin d'un toilettage de des textes réglementaires qui peuvent exister, qui concerne les secrétaires de mairie puisque on a de différences d'appréciation, on l'a vu notamment en auditionnant soit la direction de la fonction publique de votre ministère Monsieur le Ministre soit la fédération des centres de gestion. Qui ont des lectures différentes de ce qu'est un secrétaire de mairie de quelle strate ils interviennent et donc. C'est l'empilement des textes au fur et à mesure des années qui fait qu'aujourd'hui il y a des des des des difficultés de lecture et réglementaire. Le secrétaire de mairie, c'est le décret de 87, c'est moins de 3500 habitants. On parle souvent de moins de 2000. Pourquoi, parce qu'au sud de 1000 on peut avoir des DGS mais on peut c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, il y a donc un flou par exemple sur ce qui se passe entre 2000 et 3500 habitants sur le, sur sur les secrétaires de mairie on vous on on souhaiterait donc rappeler à c'est à cette occasion, alors qu'on va parler de ce qu'il a un secrétaire de mairie de ce qu'est un secrétaire général de mairie, de la nécessité de faire un texte probablement une circulaire Monsieur le Ministre qui puisse rappeler à la fois l'émission les fonctions les différentes strates les suggestions afférentes à chaque à chacune de de ses fonctions en renvoyant vers des textes réglementaires et en l'étoile autant un petit peu puisqu'on va créer peu probablement tout à l'heure un type de secrétaire général qui existe déjà dans un des textes qui est, qui a été pris à mon avis de, de manière, de manière maladroite. Donc, cette intervention était pour rappeler les choses pour dire on va on va voir un certain nombre de discussions tout à l'heure sur des questions de strates de noms de statut. Je pense que on doit faire ce travail de de toilettage des textes et probablement d'une circulaire cadre qui permettre d'expliquer vraiment toutes les toutes les différentes fonctions et de renvoyer vers les textes Ferrand, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-François Longeot. Merci madame la présidente, monsieur le ministre. Merci de m'accorder cette ce moment pour. Rappeler le rôle des secrétaires de mairie dans nos collectivités rôle qui est fondamental. Ce sont les bras droit des mères et les compétences dont elle doit faire preuve au quotidien sont nombreuses. Pourtant, d'ici à 2030 un tiers des effectifs des secrétaires de mairie seront à la retraite et les maires essentiellement en milieu rural se trouveront démunis. Si les fonctions de secrétaire de mairie ni nécessite une polyvalence accrue et ça a été dit et des compétences plurielle cela demeure pas moins une fonction invisible qui Aspire au petit à obtenir une réelle reconnaissance tout d'abord, il est évident que la dénomination doit être changé pour que la fonction soit mieux reconnue, secrétaire général de mairie. Conviendrait très certainement mieux. Mais le plus important demeure la. La revalorisation de ce métier puisque 60,5% occupent actuellement des postes d'agents de catégorie C ce qui ne respond correspond aucunement à la réalité du métier. Il serait donc important d'obtenir une validation des acquis pour que ces agents puissent passer de la catégorie C à la catégorie B sans passer de concours et que les différences de traitement entre titulaires et non titulaires, soit éviter. Des grilles un indiciaire d'indemnisation propre pourraient être mises en place en adéquation avec leurs responsabilités et les multiples savoir-faire nécessaires en effet la mise en place du Rifseep. As certainement combler une partie des lacunes de la grille indiciaire de la fonction publique avec l'augmentation du SMIG, mais ça ne suffit pas. La formation doit être davantage accompagner pour permettre au secrétaire de se former tout au long de leur carrière en effet que la forte évolution normatives induit inévitablement une technicité accrue des secrétaires impliqués, qui ne comptent pas leur temps qui effectue le plus souvent. Plus de 35 heures hebdomadaires ayant droit à de travailler 40 heures 25 mai ces heures ne sont actuellement pas pris en compte et c'est important vient débat sur les retraites pour le calcul de la retraite, tout comme 80% du Rif cette. Il est donc important de répondent aujourd'hui aux attentes de nos secrétaires de mairie ne les. Décevons pas une nouvelle fois merci. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci ma madame a présenter je je le ferai pas à chaque article mais puisqu'il y a eu des prises de parole sur l'article un mot à mon tour, en réponse au fond à ce que le sénateur Vial a pu indiquer. Vous indiquez à juste titre que nous avons besoin d'un toilettage réglementaire. Vous appelez à ce qu'on puisse avoir une circulaire cadre on aura le débat d'intitulés de fonction nature de grade. Je crois en effet que beaucoup de sujets sont d'ordre réglementaire et donc je voulais dire, Au démarrage de nos débats que je prends cet engagement-là de traduire effectivement dans les textes réglementaires et de formuler cette circulaire cadre à l'issue de l'adoption de cette proposition de loi et donc je voulais poser, ceci pour fixer un cadre à nos débats. Merci. Nous allons commencer par l'amendement numéro 10. Monsieur Vial. Oui merci madame la présidente. Merci d'abord Monsieur le Ministre pour votre réponse sur la circulaire. Cet amendement 10 est relativement important puisqu'il il parle effectivement de la question de la dénomination c'est un vieux sujet. Il a 40 ans il y a, on a souvent tergiversé. On n'a jamais trouvé vraiment de solution notamment la la seule fois où on avait tranché pour créer un cadre d'emploi commun au secrétaire de mairie. difficiles, très très différentes dans un derrière une seule dénomination ce qui finalement a posé un certain nombre de problèmes et a abouti à l'extinction de ce cas d'emploi. La proposition que, que l'on fait par cet amendement. C'est de considérer. Hein comme ça a été dit aussi par la rapporteure tout à l'heure que les fonctions de secrétaire de mairie relève de du catégorie B.

c'est pour les B et Léa laisser aujourd'hui reste secrétaire de mairie, ils sont 60% aujourd'hui, c'est la majorité. Par contre, effectivement dans le dispositif qui est prévu, on va tout faire pour essayer d'accompagner ses secrétaires de mairie par de la formation par la promotion interne qui reconnaît l'expérience, on va les accompagner vers la fonction de secrétaire général de mairie, c'est là aussi cette volonté d'une d'une de leur proposer une évolution professionnelle de secrétaire de mairie à secrétaire général de mairie qui devient la norme. Quelle que soit la strate. Mais par rapport au grade de l'agent et par rapport aux compétences de l'agent peut être secrétaire général de mairie dans une commune de 50 habitants d'une commune de 3500 habitants. Donc cet amendement rappelle ça avec cette distinction de dire on parle bien de secrétaire général de mairie à partir du du grade B ou ah dans toutes les communes de moins 3500 habitants. Entre nous par rapport à cette appellation. Je suis complètement d'accord avec vous pour dire qu'il faut changer l'appellation et secrétaire général de mairie me convient tout à fait, mais j'allais dire me convient tout à fait quel que soit le grade. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure et vous l'avez repris pour moi. In fine, Une secrétaire de mairie devra être de catégorie B alors inscrire maintenant dans la loi que les catégories C s'appelle secrétaire de mairie, ça me chagrine un petit peu voilà je suis sur la réserve. Et d'autre part faire une distinction d'appellation entre deux collègues. Qui exerce les mêmes fonctions mais qui n'ont pas le même grade. Voilà je suis réservé aussi mais toutefois je vais mettre un avis de sagesse. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la présidente est exactement le même avis que la rapporteure pour être très clair dans le débat de points de convergence absolue avec votre argumentaire. La nécessité de changer l'intitulé de la fonction, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, secrétaire général de mairie, il me semble qu'un consensus et donc je soutiendrai d'ailleurs des amendements qui prévoient cet intitulé de la fonction et l'inscrire dans la loi 2ème point de convergence que à partir de 2029 l'ensemble des secrétaires de mairie soit de catégorie B le point divergence est le même que celui de la rapporteure elle a très bien exprimé j'j'ai ajoute le point que la traduction la correspondance. Entre la fonction et la catégorie et de nature réglementaire et j'ai indiqué que je prends les engagements de données traduction réglementaire à la correspondance catégorie B ou ah. Pour le secrétaire général de mairie si c'est le choix qui est fait par la Haute Assemblée. Monsieur Bourgi non très bien. Si ce qu'. Papa. On a vite demande de retrait au profit des amendements qui porteront le changement d'intitulé simplement. Monsieur Vial. Vous avez demandé la parole. Ah monsieur Rhissa pardon. Oui madame la présidente, moi je voudrais sur le fond, soutenir la proposition de monsieur Vial, parce que je je crois que, en effet, cette reconnaissance du terme de secrétaire général de mairie est est en même temps l'expression de la reconnaissance d'un niveau de qualification qui sera validé lorsque les personnes seront élevé à la catégorie B, en application de l'article 1er, ceci dit si c'est du domaine réglementaire, je suppose que notre collègue acceptera de retirer son amendement. Mais ce que je souhaiterais, c'est que la position du ministre compte le décret sortira, soit bien que ce terme de secrétaire général de mairie soit réservé aux agents qui ont franchi le cap de formation et de qualification qui justifie la catégorie mais les autres restant catégorie étant en situation transitoire avant la période de 2029. c'est un sujet de fond parce que je pense que ça peut déterminer effectivement tout ce qu'on souhaite mettre derrière. C'était une proposition qui est au coeur du rapport de la mission parlementaire qu'on a fait justement, c'est là notre point de désaccord avec Catherine Di Folco. Si vous voulez supprimer les les les catégories c'est bien sûr pas physiquement, si vous voulez supprimer les catégories C donnait pas de ne ne leur donnait pas le titre que de secrétaire général de mairie le le l'objectif justement c'est de dire demain dans les mairies, on a besoin de secrétaires généraux, ce qui ne le sont pas, peuvent le devenir. Mais sinon pour le devenir, il faut être B ou C si vous leur donnez le titre aux agents de catégorie C de secrétaire général de mairie vous les incitez pas à passer à passer mais toute la logique de du rapport c'est dire maintenant on doit mettre en place des filières de formation, formation, elles doivent conduire vers le vers le B vers des types de secrétaires généraux de mairie laissée. Ils sont 60% il faut non pas les transformer en bé non pas les supprimer, il faut les accompagner pour devenir bé en reconnaissant leur expérience parce qu'ils exercent déjà des missions de B et donc on les, on va aller passer B ou en les pas par une formation ils vont ils vont passer. Bé ils sont 60% aujourd'hui. Les procédures qu'on va étudier tout à l'heure avec les règles de droit commun. C'est 25 à 30% qui vont passer de C à B.. Il en restera encore 40 ou 45%. Notre objectif, c'est quoi, c'est que c'est 40 et 45% ils ils ont les continue à les inciter à passer B et et donc pour ça qu'on les incite à faire la formation avec un examen professionnel, passé la promotion interne un peu plus tard pour passer mais c'est ça l'objectif. Et donc justement parce qu'on ne concourent au même objectif. Il faut faire cette distinction. C'est une manière de, de, de leur proposer à ses agents une évolution de leur dire c'est pas la même chose. Par contre, vous pouvez devenir ça et et on souhaite que vous que son reconnaissent vos, vos compétences, soit vous le deviendrez, je pense que c'est c'est c'est vertueux et c'est c'est là probablement la clé de tout ce qu'on veut mettre en place ensemble je la, je diffère avec vous monsieur Ministre madame la rapporteure. Je pense que c'est aux maires, de décider qui veulent embaucher, c'est pas au ministère de leur dire vous avez le droit ou pas le droit d'embaucher un tel. Ou pas a-t-elle ils embaucheront qui volent. Par contre ils embauchent hein catégorie il ne sera pas secrétaire général de mairie. Merci cher collègue Madame brûle hein pour. Explication de vote. Merci madame la présidente. J'ai plutôt tendance à être d'accord avec la rapporteure. D'abord parce que effectivement il s'agit d'accompagner. 60% des secrétaires de mairie qui sont aujourd'hui en catégorie C vers la catégorie B. ça va quand même prendre un petit peu de temps, il me semble même si on veut tous accélérer les choses. Et donc. Des. Femmes en l'occurrence puisque ce sont essentiellement des femmes vont continuer de s'appeler secrétaire de mairie quand d'autres de leurs collègues exerçant exactement la même profession s'appelleront, secrétaire général de mairie. Donc je crois que leur demande de reconnaissance. Ne sera pas exaucé, au sens où certaines peuvent qu'on se sentir un peu rabaissé, j'aime pas bien le terme mais par le le fait de conserver l'appellation actuelle qui deviendrait finalement un peu désuète. Et en plus il me semble que dans tous nos débats. Nous avions aussi intégrer la dimension rendons lisibles. La particularité de ce métier et qui exercent une profession particulière qu'on veut faire reconnaître portent des noms différents, on va ajouter de la confusion, alors qu'on veut au contraire essayer de clarifier les choses et de mieux dire ce que recouvre cette profession. Donc moi je serais plutôt pour ne pas faire la distinction hormis. Mais ça je pense que ça tombe un peu sous le sens entre secrétaire général de mairie et DGS puisque, effectivement, ça n'est pas du tout la même catégorie. Merci. Cher collègue, Monsieur Bourgi pour explication de vote. Oui madame la présidente, mes chers collègues. Exactement les mêmes arguments que Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre et ma collègue Céline Brulin, mais je vais en apporter un autre à nos réflexions, vous le savez très bien les métiers de secrétaire de mairie, ce sont souvent des métiers à temps partiel des contrats à temps partiel. Mettons-nous à la place d'une secrétaire ou d'un secrétaire de mairie qui travailleraient dans 2 ou 3 communes en fonction de la strate de la commune là il serait secrétaire de mairie et dans l'autre commune, secrétaire général. Il me semble qu'il serait souhaitable et qu'il puisse y avoir et une cohérence d'ensemble et qu'on appelle tout le monde secrétaire général par ailleurs dans l'amendement qui est proposé, je vois une référence à la catégorie C or tous nos travaux ont consisté à dire, il faut en finir avec les catégories C lorsqu'ils sont recrutés sur les métiers de secrétaire de mairie. Donc si jamais on dit qu'on veut résorber la catégorie C, c'est pas pour l'inscrire dans la loi et pour donner l'occasion à des mères de continuer à recruter des catégories C, sinon on n'aura jamais fini avec la déprécarisation des secrétaire de mairie. Merci. Je mets donc on voit cet amendement avec un avis de sagesse de la Commission défavorable du gouvernement. À noter que si nous votons cette à moment il fait tomber les 2 autres amendements. Qui vote pour.

Qui vote contre. Qui vote contre. On fait un assis debout, ce sera plus clair. Qui vote pour. Qui vote contre.

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord saluer bien sûr les avancées contenues dans cette proposition de loi sur l'été rappelé visant à revaloriser le métier des secrétaires de mairie. Qui est essentiel au fonctionnement des mairies à la fois pour les habitants en tant que 1er service public de proximité, mais aussi pour le maire en tant que principal. Et parfois. Collaborateurs les différentes mesures prévues pour renforcer l'attractivité de ce métier sont satisfaisantes, mais comme cela a été dit malheureusement insuffisante face à la forte tension de recrutement dans la fonction publique territoriale où plus de 1970 postes sont vacants. Aujourd'hui, le recours aux contractuels pour les emplois de secrétaire de mairie, et de plus en plus nécessaire notamment dans les communes rurales. Les personnes qui exercent ce métier connaissent de nombreuses contraintes sociales, familiales et professionnelles. Il ne dispose pas bien souvent des conditions pour préparer et réussir les concours internes. Pour cette raison, j'avais proposé un amendement ouvrant une possibilité de titularisation pour les agents contractuels. Cette solution permettrait de conserver les contractuels en poste qui sont tentés d'arrêter et d'attirer de nouveaux profils dans cet amendement j'avais pris toutes les précautions nécessaires. pour mettre en place une une expérimentation cependant cet amendement a été déclarée irrecevable en application de l'article 40. Alors que les personnes visées par le ou positif proposés sont déjà des agents contractuels. Il ne s'agissait donc pas de créer ou d'aggraver une charge publique, je ne peux que déplorer que l'initiative législative dont nous disposons en tant que parlementaire soit de plus en plus limitées et contrainte par une interprétation visiblement excessive des articles 40 et 45 de la Constitution. Je vous remercie. monsieur Billac juste pour explication pourquoi non non non non, je vous donne pas la parole. Non, je ne vous donne pas la parole. Non, c'est simplement pour vous dire que votre amendement. Est tomber parce qu'il est satisfait. C'est-à-dire qu'il mettait ou à temps non complet

Merci madame la présidente, mes chers collègues. Les agents sur le terrain sont mis face à des paradoxes d'or or guide organisationnel qui freine très largement l'amélioration de l'attractivité du métier de secrétaire de mairie suite au partage des travaux de la délégation aux collectivités et de sa présidente Françoise Gatel je cite une réaction du secrétaire de mairie avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger. Certains agents ont passé les examens et nous ne monte pas en catégorie d'autres changent de catégorie sans avoir obtenu d'examen s'secrétaire de mairie vendéenne a passé et obtenu en 2005 l'examen pour devenir rédactrice territoriale pourtant en 2023, soit près de 20 ans plus tard, elle est toujours considérée adjointe administrative de première classe. J'imagine qu'elle n'est pas la seule dans cette situation, une situation qui crée de la frustration chez les agents, que nous pouvons aisément concevoir sur l'ensemble de la Vendée. Il n'y a que 6 postes de rédacteur, ce qui est loin d'être suffisant, le peu de postes ouverts limite les perspectives d'évolution des agents et freine le renforcement de l'attractivité du métier. Il est urgent donc de remédier à cette carence de reconnaissance les de nouvelles voies de promotion interne sont les bienvenues, évidemment. Merci.

qui sont pas au fait de de toutes les règlements de la fonction publique territoriale, pour passer de CMB avec ce dispositif de promotion interne hors quota qui est une très bonne chose. Le droit commun prévoit qu'il faut avoir il faut être fonctionnaire depuis territoriales depuis 8 ans minimum et en poste depuis 4 ans. Ça représente 25 à 30%. Ce que je disais un sondage que j'ai fait je ne sais pas, c'est une féministe. Si vous avez des chiffres plus précis des statistiques à nous donner. Donc ça va représenter 25 ou 30% c'est bien mais ça ne fait pas la rue Michel comme comme on dit, il y aura, il faudra encore mettre d'autres d'autres dispositifs. Deuxièmement. dans dans cette dans la mission si on veut vraiment. Revaloriser les secrétaires de mairie. Ce qu'il faut c'est pas uniquement gérer le stock des secrétaires de mairie c'est leur offrir des perspectives d'évolution, c'est-à-dire que oui, celles qui sont catégorisés il faut leur permettent de pouvoir évoluer en catégorie B et en le faisant avec des procédures qui soit plus simple et plus adaptés à leurs responsabilités dans leurs fonctions, mais il faut qu'elles aient un parcours celles qui sont bé aussi devrait pouvoir passer bé veut passer. Ah devrait passer non pas plus mais au moins attachée principale. On a une règle, Monsieur le Ministre qui interdit, interdit d'avoir d'embaucher un attaché principale dans une commune de moins de 1000 habitants interdit, il faut changer de strates si si vous êtes à et que vous voulez évoluer sur votre poste. Il faut quand il faut changer de collectivité. Moi je vous invite. Dans, dans, dans ma commune, ça m'est arrivé 3 fois un devoir changer de secrétaire de mairie parce que elle avait réussi justement l'examen professionnel pour progresser à la plus le droit de rester travailler dans ma commune je vous invite à voir des des communes touristiques qui ont 10.000 lits touristiques qui ont 500 800 habitants, ils ont pas le droit d'avoir des catégories des attachés principaux et pourtant ils gèrent des équipements beaucoup de suite beaucoup plus gros que des des communes des fois de 3 ou 4000 habitants. Il faut permettre aux agents d'avoir des évolutions de carrière des perspectives de carrière, malheureusement le dispositif aujourd'hui il est important, il est très incomplet. Si madame Céline Brulin. Merci madame la présidente, je voudrais abonder les arguments que vient de développer notre collègue Cédric Vial parce que il y a en effet. Déjà des, des tâches de secrétaire de mairie qui peuvent tout à fait relever. De la conception, voire de l'encadrement et qui justifierait pleinement. Qu'on puisse recruter davantage de catégorie A dans les mairies, y compris les petites. Chacun a son exemple, moi j'ai un exemple d'une commune qui est sur une zone industrielle. Industrie allô portuaire et qui a des enjeux d'aménagement industriel considérable et qui a besoin de compétences en la matière et puis effectivement je pense que il y a beaucoup de secrétaires de mairie qui sont aujourd'hui en catégorie B et qui doivent elles aussi pouvoir continuer d'évoluer de progresser dans leur carrière pour atteindre la catégorie A, voire plus. Et Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger très clairement pourquoi refusez-vous qu'on aille vers cela. J'ai ajoute une inquiétude parce que dans les mesures si j'ai bien compris que vous avez annoncé ces jours derniers. Vous envisagez. Outre la la revalorisation d'un point et demi du point d'indice que tout le monde trouve insuffisante des. Primes, que vous jugez ciblés essentiellement sur les catégories C et B. Mais tout ça Boutabout fait qu'on va aller vers un espèce d'écrasement de la grille ou peut être que les catégories C pourront progresser Amber peut-être qu'il y aura quelques modestes améliorations salariales pour les catégories C et B mais pas pour les ah, c'est-à-dire que c'est un genre de cadeau empoisonné pour demain. Puisque, une fois arrivé aux catégories B avec y compris des rebelles. L'organisation salariale même modeste. Eh bien la progression en terme salarial ne pourra plus se poursuivent pour les catégories A, c'est-à-dire que le problème de pouvoir d'achat que vous entendez ou prétendait régler aujourd'hui il se reposera avec force demain. À cause de l'écrasement de cette grille et donc nous voulons savoir quelle est la raison qui vous conduit à proposer ce genre de mesure. Merci. Merci la parole est à présent un autre collègue monsieur Arnaud. Oui madame la présidente. À l'occasion de de la discussion de cet article 1 et 2. Je souhaiterais avoir quelques précisions. Je me suis évidemment rapproché de mon sang de gestion de la fonction publique territoriale du département des Hautes-Alpes. Et je constate que les secrétaires de mairie exerçant. Avant tout leur fonction dans les départements ruraux, le faible nombre d'argent d'agents limite l'ouverture des postes par votre promotion interne pour les catégories B rédacteur. En application de l'article. 9 du décret du 22 mars 2010 le quota de promotion interne et d'une inscription sur la liste d'aptitude pour trois recrutement intervenu par d'autres voies. Recrutement de lauréats de concours inscription sur liste d'aptitude ou encore recrutements effectués par les voies de détachement ou de mutation une intégration directe. Si on applique cette règle dans mon département a-t-il illustration en 2023 dans le département des Hautes-Alpes un poste seraient ouverte de rédacteur catégorie B pour 37 candidats, un poste ouvert d'attacher catégorie A donc pour 23 candidats de. Or, ce que le projet semble pas dire précisément et qu'il est primordial de mon point de vue de connaître ce sont les modalités permettant de définir le nombre de postes ouverts pour les secrétaires de mairie par votre promotion interne l'exposé des motifs. Indique qu'il s'agit d'une voie dérogatoire en dehors des quotas, ce qui signifierait de mon point de vue que tous les agents remplissant les fonctions de secrétaire de mairie avec les critères d'ancienneté de promotion interne seraient automatiquement promus à l'instar des agents de maîtrise, je vous demande si c'est bien le cas de bien vouloir me le confirmer pour que les choses soient bien claires et que l'on puisse vis-à-vis de nos collaborateurs qui sont dans cette dynamique-là dans des départements où il y a très peu de promotion, compte tenu du du quota que j'ai d'évoquer que les choses soient effectivement précise, c'est la seule façon de rassurer et surtout de maintenir une dynamique de promotion et d'évolution pour nos collaborateurs qui non à défaut que d'autres choix de partir le département là où il y a plus d'offres de quotas ouvert je vous remercie de bien vouloir m'apporter ces précisions. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il se trouve que le Sénat a rendu hier un rapport sur l'impact des normes sur la gestion de nos collectivités locales. Et dans ce rapport que souligne-t-on je vais présider cette. Mission d'information. Yann Pantel en était le rapporteur au titre du groupe RDSE. C'était une initiative. Du RDSE. C'est qu'il faut libérer un peu la gestion administrative de nos collectivités. Alors évidemment cette PPL ne veut pas embrassé aussi largement ce qui relève bien souvent du pouvoir réglementaire. Monsieur le Ministre, mais entendu cet appel. Ce que vient de vous dire Jean Michel à ce que vient de vous dire Cédric Vial. Et un peu partout sur tous les bancs. C'est que vous le ministère central la fonction publique. Est encore au ministère. Or il s'agit de fonction publique territoriale et il faut aussi laisser dans la libre administration des collectivités, beaucoup plus, beaucoup plus de souplesse sans introduit cette PPL on introduit un peu doivent reconnaître les choses mais enfin il y a loin de la coupe aux lèvres. On ne va pas aller loin, on va faire beaucoup de frustration et on va encore venir beaucoup de choses et à avoir en vérité, peu de résultats. Et les gens beaucoup plus frustré. Je vous invite monsieur le ministre à aller beaucoup plus loin. Qu'il est possible, c'est une possibilité. C'est pas une obligation. De passer de catégorie C, en catégorie B sans quota. Bon, encore faut-il que la collectivité présente le dossier de l'agent à la promotion interne. Et si cet agent. Figure sur la liste d'aptitude. Encore faut-il que la collectivité ouvre le poste en catégorie B pour nommer son agent, on est d'accord. C'est le principe même d'une promotion interne. Mais là ce qu'on facilite ce passage en enlevant le quota en réalité celui dont vous avez parlé d'un pour trois. Pendant cette période dérogatoire des 5 ans. Il n'y aura pas de quotas. Mais c'est pas automatique, c'est pas systématique c'est peuvent il y a le mot peut dans le dans le texte de. Du projet de loi, donc ça veut dire que le maire. Peut présenter le dossier de son agent. Et si l'agent est sur la liste d'aptitude après il pourra ouvrir le poste il n'en a pas l'obligation. Mais c'est une facilité qui est accordée. C'est un assouplissement temporaire. Très bien. Nous passons à l'étude des amendements. Trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 3 Monsieur Bourgi. L'amendement numéro 13 Monsieur Oui merci madame la présidente. On passe à l'amendement 13, que malheureusement l'amendement 12. Qui a été frappée d'irrecevabilité pour l'Arctique 40 il aurait suffi. Monsieur le Ministre que dans votre discussion générale, vous disiez que vous étiez favorable au moins ce qu'on est à la discussion pour que cet amendement ne tombe pas, ça faisait partie des des des demandes que que j'avais pu formuler malheureusement. On on en restera donc. Au simple catégorie C qui pourront passer en bé je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure là. L'amendement numéro 13 lui-prévoit de. Demander au secrétaire de mairie qui deviendront, secrétaire général de mairie par la promotion interne de un engagement d'au moins 3 ans dans le poste. Notre objectif, il est bien clair. 10.000 postes à recruter d'ici. D'ici 2030. Si on ne met pas tout en oeuvre pour essayer de garder les secrétaires de mairie qui sont en place, de les promouvoir pour les garder et que cette promotion interne ne soit pas uniquement un moyen d'accéder à la catégorie B sans sans passer le concours mais que ça soit bien un moyen pour reconnaître les les secrétaires généraux de mairie et de les conserver dans leur poste. Alors c'est une mesure qui pourrait être de bon sens. compliqué des fois à mettre en oeuvre. Mais ça se fait déjà pour des formations de médecin ou dans, dans d'autres dans d'autres professions, il y a ce type d'obligations qui est mis en place, ça nous permettrait en tous les cas de d'améliorer nos chances de de réussir le défi qui est le le recrutement je rappelle de 10.000 agents d'ici 2030. Merci. L'amendement numéro 19 monsieur Billac. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Dans cet article 1er acheteur une voie de promotion interne dérogatoire et temporaire pour permettre aux agents il exerça les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre emplois dans la catégorie c'est. D'être nommée dans un carton d'emploi de la catégorie B. L'alinéa 2 précise que les modalités d'application de certains veulent voir de promotion interne serait précisée par un décret en Conseil d'État. Et là je rejoins la remarque que même de faire mon collègue Bocher.

Les modalités de fixer les modalités. Pourquoi. Renvoyer un décret madame la rapporteur j'ai siégé 12h alors conseil national des valeurs chaude d'énormes. Et je prends le pari aujourd'hui ici que ce décret il va mettre tellement de conditions Thalmann d'Arkan Thelma de complications qui sera applicable nulle part. Voilà je crois votre bonne foi mais je connais trop l'administration pardonnez-moi. Merci madame le rapporteur, votre avis sur les trois amendements, s'il vous plaît. Merci madame la présidente. Alors Monsieur Bourgi, je, je suis désolé mais du coup. Avec l'adoption de l'amendement de monsieur Vial précédemment. donc fait la distinction entre les catégories C les catégories B et donc une appellation différente. Il n'y a plus de coordination par rapport à votre. À votre amendement. Donc je vous demanderai un retrait ça sera plus, plus logique. Voilà, la coordination est tombé.

ou de directeur général des services. Alors j'ai j'ai juste de petits soucis. En réalité c'est pas opérants parce que quand vous parlez de directeurs généraux des services, on est d'accord, c'est un emploi fonctionnel et si c'est un emploi fonctionnel. On ne peut pas obliger à rester 3 ans puisque cet emploi dépend de la volonté de la collectivité du maire précisément de garder ou pas garder. Le l'agent. Donc c'est pas opérationnel par rapport à ça de plus. Je comprends votre idée de fidéliser mais l'idée de fidéliser c'est quand même de fidéliser dans la commune qui a fait la promotion de cet agent. Or, comme ses rédiger c'est marqué un poste de secrétaire général. Donc le poste de secrétaire général. Après tout, il pourrait bien exercer dans une autre commune et auquel cas on aurait perdu cette fidélisation. Dans la commune qui a vu elles-mêmes. Enfin qui a pu promettre qu'il a pu promouvoir l'agent pardonnez-moi donc ça me semble inopérant donc. si possible. Un retrait ou un avis. Défavorable. Alors Monsieur Biya. Je vais vous expliquer pourquoi j'émets un avis défavorable par rapport à votre demande. Pourquoi, parce que, en réalité, les centres de gestion. Ils peuvent édicter des lignes directrices de gestion. Et six édictent des lignes directrices de gestion, ce n'est pas au niveau de la C. A. P. qu'elles sont admises. C'est au niveau du comité social territorial Votre rédaction n'est pas opérante. Donc on ne peut pas s'en satisfaire. Et deuxièmement, si on confie au Centre de gestion. Les modalités il y a 90 centres de gestion. Il peut y avoir 80 10 modalités différentes. Or, si c'est un, un décret en Conseil d'État c'est une uniformisation des modalités pour l'ensemble de. Des agents de l'ensemble du territoire et donc c'est quand même plus avantageux. Voilà donc c'était une demande de retrait ou un avis défavorable. oui madame la présidente, j'ai, j'ai exactement les les mêmes avis je veux juste préciser que sur le le première. Amendement qui a été présenté de Monsieur Bourgi. J'y suis favorable de principe je je l'ai défendu ici je dirais sagesse pour des raisons de coordination est retiré monsieur les retirer mais vous connaîtrez donc ma position principe ciel et je trouve que la rapporteure a extrêmement bien préciser les choses, sur les 2 autres amendements dont j'ai exactement le même avis. Merci monsieur Billac pour explication de vote. Oui madame la rapporteure taille à 88 chantre de gestion, j'entends. Je vous informe qu'il y a aussi la Fédération nationale des de projection qui coordonne l'action du Centre. Et puis on ne peut pas répéter ici à longueur de faire que la France est diverse que la France est différente que les territoires ne sont pas tous les mêmes que ça pose un problème de sclérose dans notre pays d'avoir des règlements identique et puis bah je qu'il faut un règlement identique. Pour des secrétaires de mairie. Les communes rurales Grand-Am mais je ne comprends pas tout, pardonnez-moi. Donc je maintiens mon amendement.

puisque, au sud de 1000 habitants. On peut être directeur général des services sur un emploi fonctionnel on peut. Il faut une délibération du conseil municipal et il faut l'accord de l'agent. Sinon qu'est-ce qui se passe au de 2000 habitants. Un agent de catégorie A. qui est en poste peut avoir le titre de de directeur général des services. Aujourd'hui, c'est prévu dans les textes sans vous être emploi fonctionnel, c'est pour ça que je l'avais précisé comme ça part et c'est pour ça que je vous Monsieur le Ministre vous demandais qu'il faut clarifier sa parce qu'aujourd'hui les, les, les choses sont plus claires. Donc ça c'était le, le premier point après effectivement vous avez raison, moi, mon objectif, c'était que la les agents qu'on promeuve reste secrétaire général s'change de communes peu importe au moins qu'on affaiblisse pas le viviez voilà donc si je voulais juste apporter ces éléments d'éclaircissements mais je je je comprends les les autres aux arguments du rapporteur, et je retire cet amendement. Très bien je mets donc aux voix l'amendement numéro 19 avec 2 avis défavorables qui vote pour. Monsieur Biya, je suppose que vous votez pour votre amendement. Très bien, qui votent contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté.

Cinq amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 33 présenté par Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente. Cet amendement il part d'un principe qui, me semble-t-il fait consensus. Elle a été rappelée par Madame la rapporteure c'est qu'à compter de 2029. L'ensemble des recrutements de secrétaire de mairie puisse se faire en catégorie B. Ceci étant posé, pour la clarté des débats. Moi mon. Obsession d'une certaine façon et je crois qu'elle est partagée, c'est de pas fermer les viviers de recrutement d'ici là et donc de garder la possibilité d'ici 2029 que dans le vivier de la fonction publique. L'éditorial qui est aujourd'hui composé à trois quarts d'agents de catégorie C, on puisse continuer à faire des recrutements en catégorie C dans la secrétaire de mairie Qu'on permette aux agents de catégorie C mais qui ne seront pas dans les conditions requises, d'un certain nombre d'années d'expérience par exemple pour bénéficier du quota de promotion qu'on nous allons créer par cette PPL à travers la validation des acquis de l'expérience de pouvoir accéder à cette formation, de qualification et ainsi accéder à la catégorie B et à cette fonction de secrétaire général de mairie et donc je viens modifier le dispositif pour dans la période transitoire. De ne pas restreint des quotas de promotion et de donner à mon sens la pleine effectivité à cet article de créée par cette proposition de loi. Merci l'amendement numéro IV Monsieur

Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. L'article de tend à créer une voie de promotion interne pour les fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et relevant d'un cadre d'emploi de catégorie C qui ont validé une formation qualifiante. La commission a toutefois souhaité différer au 1er janvier 2029, l'entrée en vigueur de cette disposition afin de rang de plus opérationnel, l'articulation entre les dispositifs dérogatoires temporaires de l'article 1 et la disposition pérenne de l'article 2, secrétaire de mairie sont les piliers sur lesquels repose la gestion quotidienne des affaires municipales. Ils sont les gardiens des procédures administratives des dossiers, les décisions prises par nos élus, leur polyvalence et leur adaptabilité sont des qualités indispensables pour faire face aux exigences d'un poste aussi diversifiée. Mais d'ici 2030, un tiers des secrétaires de mairie partiront à la retraite. Les candidats ne se pressent pas pour prendre leur poste aussi il me semble nécessaire que ce dispositif qui vise à favoriser des vocations. Les candidatures pour un métier particulièrement en tension puissent entrer rapidement en vigueur. Je vous remercie. Merci Monsieur Patriat l'amendement de mais en Je vais aller très très vite puisqu'il vient d'être très bien défendu par mon collègue monsieur Gold simplement. Travaux il est défendu. Parce que je vous dis positive, visant à encourager les vocations des candidatures aussi il importe qu'il puisse entrer en vigueur très rapidement

S'interroge et ça a été expliqué tout à l'heure par Madame la rapporteure à une réponse à notre collègue Bihac. C'est de savoir pourquoi une. De mode de promotion successifs et pourquoi on n'ouvre pas tout des de 2024 donc c'est ça que propose de faire cet amendement, passer de 2029 pour le. Second la seconde voie à 2024. On fidélise, on y va, on fait on fait masse de tout ça nous paraissait de bon sens. Merci. Madame le rapporteur vous avis s'il vous plaît. Merci madame la présidente, alors. En ce qui concerne le l'amendement numéro 33 présenté par le gouvernement. Je l'ai dit dans mon propos introductif, ce sera un avis favorable. Ensuite les amendements suivants. En réalité, ce seront des avis de sagesse et je crains fort que si l'amendement du Gouvernement est adopté, il ne tombe.

l'amendement numéro 33 donc demande de retrait. Si le principe qu'il ait convergence. Je crois qu'on l'a exprimé comme test c'est-à-dire de pas fermer la possibilité de donner accès à cette formation, de qualification aux aux agents de catégorie C dès l'adoption du texte. Le principe est le même et donc je vous propose de retirer les amendements au profit de de l'amendement numéro 33. vote. Oui pour pour une petite et je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur ce dispositif. Le dispositif qu'on a voté tout à l'heure sur la promotion interne hors quota va permettre probablement assez rapidement de régler le cas de 30% des agents 60% catégorie c'est 20% de catégorie B si le dispositif fonctionne à plein régime on va on va arriver à peu près à 40 40 40 % de ces 40% de B. Si votre objectif, c'est qu'en 2029, il est plus que des Mais comment faites-vous, si vous ne mettez pas un accélérateur sur la formation des c'est pour passer mais ça veut dire que cette formation qualifiante. Il faut qu'elle soit en place effectivement en parallèle pour tous ceux qui ne répondent pas aux critères les premiers critères, je rappelle 8 ans de fonction publique 4 ans d'ancienneté. Pour cela, pour les autres, il faut qu'ils puissent faire leur formation.

Je ne pense pas qu'on puisse interdire le recrutement de de de catégorie C cette, ce sera une voie de recrutement, même si derrière on va les accompagner vers le bé c'est ça l'objectif. On ne peut pas effacer et on n'effacera pas d'un trait de plume des agents de catégorie C, d'autant qu'on a vu plein d'exemples, ou bien accompagné dans des petites collectivités des agents. Faut faut font font très bien le travail il faut il ne faut pas non plus vouloir tout effacer, il faut vouloir faire différemment, faire mieux. Oui mais il faut être réaliste de d'ici 2029 si on accélère pas sur la formation et et. On n'y arrivera pas et l'interdiction complète me semble une fausse bonne idée. Madame la rapporteur. le gouvernement propose de le supprimer. Donc, il propose de supprimer l'entrée en vigueur de la disposition au 1er janvier 2029, donc c'est pour ça que les autres amendements sont satisfaits et vous aussi. Je mets donc aux voix l'amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui vote pour. Contre, abstention il est adopté les s'amendements suivants tombe.

Merci madame la présidente, Jean. C'est un amendement de notre collègue Alexandra banlieue au fond de type. Qui propose d'ouvrir l'accès à un emploi fonctionnel qui disposant d'une. Patrick Oury indiciaire propre à l'instar de suite désespère de haut niveau uniquement aux agents de catégorie B et A exerçant des fonctions de secrétaire de mairie. La création de ce statut d'emploi demeurerait à la main de sa commère libre par délibération de l'ouvrir ou non ou non pardon. Cependant, cela permettrait surtout une rémunération majorée en pleine considération des fonctions et responsabilités exercées de fait grâce à cette avancée cet emploi seraient mieux identifier et ne sera plus assimilé à un simple poste de secrétariat. Ce qui n'est pas le cas au regard de la technicité et polyvalence de plus en plus demandé toujours dans l'objectif de valorisation défendue par le texte. Cet amendement faciliterait leur parcours professionnel en introduisant de réelles perspectives d'évolution et en rétablissant éventuellement une représentativité plus égalitaire entre les femmes et les hommes à la Star de ce que l'on retrouve sur les strates supérieures. Merci madame la présidente, J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer lors de l'examen de la proposition de de Madame brûlant. Il y a des contraintes à l'emploi fonctionnel. Vous savez que c'est un emploi précaire. Et je ne suis pas certaine que les secrétaires de mairie et besoin d'un emploi précaire. Donc c'est une demande de retrait ou un avis défavorable. Même avis que le rapporteur en précisant que nous avons eue avec les associations d'élus, de nombreux débats sur cette question, je crois pouvoir dire je le dis haut dans l'hémicycle du Sénat que la position des associations d'élus a également évolué sur cette question. Se ralliant à la position à mon sens très sage que vient d'exprimer la rapporteure donc j'ai exactement le même avis que Madame la rapporteure. Merci. Monsieur vous retirer. Il est retiré. Nous passons à l'amendement numéro 14 de monsieur Vial. Merci madame la présidente. Ça y est, on, on rentre là maintenant dans des mesures d'accompagnement. Cet amendement prévoit d'inscrire dans les compétences obligatoires descendent de gestion. L'animation du réseau départemental des secrétaires et secrétaires généraux de de mairie. Pourquoi. Parmi les les difficultés et les contraintes des postes de de secrétaire de mairie et de secrétaires généraux de mairie désormais. Il y a l'isolement. Une étude a été faite par le le Centre de gestion de la Lozère. des des secrétaires de mairie disent ne faire partie d'aucun réseau professionnel et 84% d'entre eux disait qu'souhaiteraient faire partie d'un réseau professionnel. Ça existe déjà un certain nombre de de gestion par avec des partenaires parfois avec le l'AMF ou l'AMRF ou d'autres partenaires ont mis en place ces ces réseaux. L'estimation c'est une estimation qui qui est très empirique, c'est qu'à peu près 40, 30 à 40% des sortes de gestion de France ont mis en place ce type de réseau, c'est une demande je pense forte des des des secrétaires de mairie de pouvoir animer ce réseau, on laisse les cendres de gestion ensuite les organiser comme bon leur semble, avec les partenaires qu'ils voudront se sous sous la forme qui qui qui qui le voudront et c'est une compétence obligatoire. Ça veut dire qu'elle sera Cette prestation intégrée dans ce qu'on appelle les les zéro huit, ça veut dire, financés par la cotisation qui existe déjà sur les salaires que que les communes payent. On a l'accord. Lors de nos auditions de la Fédération nationale des centres de gestion pour cette mesure qu'ils jugent utile et de la plupart des des directeurs de son de gestion qu'on a consulté je pense que c'est une mesure de bon sens. Et et qui peut faire beaucoup pour faire progresser lutter conte l'isolement professionnel des secrétaire de mairie. Merci madame le rapporteur. Je vous laisse présenter le sous-amendement. Alors en réalité je le retire le sous-amendement madame la présidente d'accord n'a plus lieu d'être, compte tenu de, du vote sur le premier article. Fabien, vous pouvez nous donner votre avis sur l'amendement. c'est un avis favorable. Parce que je pense qu'effectivement ce ce réseau de professionnels me paraît indispensable et un bon nombre de Centre de gestion l'assurant déjà ça ne posera pas de problème à ce qu'il devienne obligatoire, donc avis favorable. Très bien. Monsieur le Ministre. J'aimais également un avis favorable à cet amendement qui part du terrain de la pratique et qui vient consacrer. Le rôle essentiel des centres de gestion. Donc, avis favorable du gouvernement. Madame Céline Brulin pour explication de vote. Cette organisation et cette évolution qui est entre autres le fruit du travail. De nos rapporteurs sur le sujet dans la délégation aux collectivités me paraît en effet nécessaire. Il se trouve que. Les secrétaires de mairie qui veulent effectivement rompre l'isolement, essayer de bénéficier les unes des autres. De de pratiques de bonnes pratiques de conseils etc. Ce sont organisées, notamment à travers un réseau social assez connu. Qui regroupe désormais plus de 9000 d'entre elles sur lequel elles échangent ce type de conseil et pour pas allonger nos débats. Je voudrais juste dire que il me semble effectivement que c'est plus au centre de gestion d'organiser. Ce réseau qu'Mark Zuckerberg. Alors juste. Nous avons jusqu'à 20h 35. Pour ce texte. Je crois que nous avons tous la volonté qu'il passe, il reste 17 amendements donc si vous voulez qu'on arrive à voter ce texte. À 20h 35. Je pense que je vous demanderai d'accélérer un peu merci je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis favorable qui votent pour. Contre, abstention. Il être adopté. Nous passons à l'amendement numéro 9 au monsieur Cabanel. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues maillon indispensable au bon fonctionnement des petites communes, le secrétaire de mairie met en oeuvre les décisions du conseil municipal, j'ai gère les ressources humaines, participe à l'élaboration du budget. Les documents administratifs et sont les interlocuteurs privilégiés des usagers. Malgré ses responsabilités de secrétaire de mairie sentent parfois peu reconnue et peu valorisé les entretiens professionnels jouent un rôle essentiel dans leur développement de carrière au froid une occasion précieuse de d'évaluer leurs compétences et leurs besoins d'formation et leurs perspectives d'évolution afin de garantir un processus d'évaluation juste et équilibré, il serait opportun que les secrétaires de mairie puisse être assisté d'un représentant syndical lors de ses entretiens où elles se retrouvent souvent seuls face au maire et ses adjoints ou devant le conseil municipal. C'est l'objet de la main demain par notre collègue aujourd'hui présidente madame n'Atari Merci cher collègue madame le rapporteur, votre avis. Je comprends l'intention mais je pense que cette mesure n'est pas n'est pas opérationnel et surtout elle est pas justifiée. Pourquoi, parce que dans une petite collectivité, on parle bien des petites collectivités, un secrétaire de mairie. Il y a pas de représentants syndicaux. La plupart du temps, donc il faudrait faire venir un représentant syndical d'une d'une d'une fédération. Départementale, régionale ou le bon qui, qui n'a pas vraiment intérêt à venir dans une petite collectivité qui ne connaît pas l'agent qui ne connaît pas la structure qui ne connaît pas le maire et etc. De plus, je me permets de radio. Tu sais que si l'agent conteste son évaluation conteste son entretien il il a le loisir de le faire auprès de la que le la commission administrative paritaire du Centre de gestion et là c'est une commission paritaire, donc il y a des élus syndicaux et des élus. Des élus qui peuvent statuer sur sa demande donc à mon avis demande de retrait chers collègues ou avis défavorable. Monsieur le Ministre même avec la rapporte. Monsieur Cabanel. Avec votre autorisation je le retire. Merci très chers collègues. Nous passons à l'article 2 bis Madame Billon pour prendre la parole sur cet article. Merci madame la présidente. Cette prise de parole résulte d'un échange avec madame Lemaire depuis tu sers l'article 2 bis vient renforcer la formation des secrétaires de mairie en créant une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées qui doit être dispensé dans un délai d'un an à compter de la prise de poste, ce dispositif est le bienvenu, compte tenu de l'offre de formation actuelle trop courte trop fragmenté comme cela et a été soulignée par la rapporteure. Ces formations sont dispensées par le Centre national de la fonction publique territoriale, en l'occurrence en Vendée, les agents doivent se rendre à la maison des communes de la Vendée à la Roche-sur-Yon poursuivent cette formation pour un grand nombre d'agents. Cela représente un temps de trajet conséquents et des difficultés de mobilité, la secrétaire de mairie depuis tu sers une commune à environ une heure de route de la préfecture a pris l'initiative de devenir référent Cnfpt afin de proposer une offre de formation locale la mairie de plus de serre au croisement de 3 communautés de communes est ainsi devenue un centre de formation pour les agents du sud Vendée les avantages de ces centres délocalisés sont multiples, ils offrent notamment la possibilité de renforcer le maillage territorial et de développer un réseau entre agent. Donc il serait donc nécessaire de tout mettre en oeuvre pour valoriser et soutenir ce type d'initiative pour qu'elle se multiplient mais aussi pour garantir leur pérennité c'est l'objet de cette intervention. Je vous remercie. Merci l'amendement numéro 5 retiré, Monsieur Durand ou oui parfait. L'amendement numéro 15 monsieur C'est un amendement de coordination la main fait madame la rapporteure votre avis. C'est un avis favorable. Monsieur le Ministre

Oui merci. Dans la présidente, là on revient sur la question de, de la formation et plus particulièrement de la formation initiale. De quelques instants sur le constat, on a lors de de de notre mission pu. Étudier un certain nombre de dispositifs qui a été mis en place en fait Monsieur il n'existe pas de formation de secrétaire de mairie. C'est un métier pour lequel il n'existe pas de formation on se forme sur le tas, on se forme à l'expérience sur le terrain depuis quelques années, certaines initiatives ont vu le jour quand même. Ici ou là une licence professionnelle. Ici ou là et c'est le le plus fréquent des diplômes universitaires des DU qui dépendent de l'université et on a eu la surprise de constater que certains de ses diplômes. Peuvent être intégrées au niveau bac, d'autres un niveau bac plus deux, je crois même en avoir vu le niveau infra-bac. Ils forment tous au même titre c'est DU secrétaire de mairie, certains comportent 100 heures de formation, d'autres 500 heures certains en apprentissage. On, on a une disparité de la formation. si on veut revaloriser le métier, il faut flécher ces formations sur un grade de catégorie B de secrétaire général de mairie, ce qu'on a vu tout à l'heure et donc que le niveau de qualification, soit a minima équivalent au au poste de B et que s'il porte le même titre si on a la même formation avec le même nom. Il faut qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans les formations que qu'on dispense et je pense, si on veut atteint notre objectif d'ici 2030 de recrutement qu'il faut même aller plus loin et qu'il faut mettre en place une filière diplômante soit de BTS soit de licences professionnelles liées aux métiers de secrétaire général de mairie, c'est un très beau métier il faut former à ce métier et ça répondra aussi une question qu'on se posera plus tard comment on communique on donne envie aux gens de venir sur ces métiers-là on met en place ces formations, on sera sur les forums des métiers, on sera présent auprès des étudiants, on fera connaître ce métier donc non seulement on a besoin d'harmoniser les choses et de le mettre en place ça c'est, ça relève de la responsabilité, notamment du ministère de l'Éducation nationale, c'est pour ça qu'on demande un rapport pour se pencher précisément. Surtout collègue madame le rapporteur. Votre avis. Alors écoutez madame la présidente, chose n'est pas courante mais pour une fois j'accepte. Un rapport parce qu'il me semble effectivement que le sujet en vaut la chandelle et qu'il s'agit de de préparer les futures formations donc pour ça il faut avoir une vue d'ensemble et par un rapport. Ça me paraît important et si vous me permettez madame la présidente. Et pour aller un peu plus vite. Le le l'amendement suivant de monsieur Gold en fait vise le même objet. Si chaque là vous aviez l'amabilité de le rendre conforme à celui de monsieur

aux décisions qu'on doit prendre. Et en l'occurrence à la formation à la mise en place de diplômes universitaire je je précise simplement que il y a aussi l'autonomie des établissements, qu'il faut respecter établissements universitaires. C'est exactement le sens du travail qu'on a initié avec ma collègue j'ai mentionné dans mon discours en discussion en général. Sylvie Retailleau, de pouvoir effectivement mettre en place ce diplôme universitaire, ce sera un élément fort d'attractivité de communication aussi autour de ce métier et donc si cela passe par un travail préalable autour d'un rapport pour faire l'état des lieux des différentes filières existantes et initiatives prises bien ça sera un avis de sagesse la part du gouvernement. Monsieur Gold vous rendez conforme et je vous laisse un temps pour. Explications de vote. Non. Très rapidement oui je rends conforme et puis je pense que ça suffit de ne pas. Très bien, parfait, je mets donc aux voix ces deux amendements identiques. Avec un avis favorable de la commission sagesse du gouvernement qui votent pour. Contre, abstention. Il est ils sont adoptés. Les amendements à l'article de terre le numéro 34 sera présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui madame la présidente, je je le présenterai rapidement parce qu'on a, on avait déjà eu ces débats à l'occasion de de l'examen de la la proposition de loi de Céline Brulin, et donc c'est une position au fond de cohérence que je vous présente là moi je suis favorable, vous l'avez compris, à tous les dispositifs qui vont nous permettre d'assouplir les quotas de promotion, on en a amplement. Débattus à l'occasion de l'examen cette PPL et donc je trouve un peu contradictoire. L'idée qu'on vienne créer. Un quota dans le quota d'une certaine façon, au moment où on vienne assouplir de façon générale, les quotas de promotion bénéfice de secrétaire de mairie donc je garde c'est un amendement de suppression de cette disposition là qui est au fond cohérente avec la position d'ensemble que j'ai pu vous présenter. Je suis désolé, c'est quand même un point de divergence entre nous. Monsieur le ministre, et moi je pense qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route les catégories B, je le rappelle dans ces catégories B il y a des personnes qui exercent depuis de fort longues années, qui ne peuvent pas prétendre facilement à cette promotion interne qui est dans le droit commun hein on est bien sur les quotas. Donc avoir un oeil un peu plus bienveillant sur sur eux me paraît indispensable. D'autant plus que l'amendement qui avait été présenté par notre collègue Vial a subi les foudres de l'article 40, je pense que cette mesure est encore plus. Importante, donc ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la commission qui vote pour. Non, vous votez contre madame le rapporteur oui qui votre Qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je retire numéro 6. Madame, Monsieur Durand, il est retiré l'amendement numéro 16 monsieur Vial. Madame le rapporteur votre avis favorable. Favorable. Favorable. Très bien, parfait. J'aimais. Donc on voit cet amendement avec 2 avis favorable qui votent pour, contre, abstention

Très brièvement. Cet amendement il est il est défendu et vise simplement à rétablir la petite sur l'Avantage spécifique de l'ancienneté. Madame le rapporteur. Alors ça, ça va être le 2ème point de divergence, je suis désolée mais ce sera un avis défavorable, parce que moi je considère que. Il y a lieu de réformer et je l'ai dit dans mon propos liminaire Des des des échelons pour l'ensemble des agents et pas faire une spécificité du métier de secrétaire de mairie dans une petite collectivité, il y a des secrétaires de mairie et des agents techniques et etc. Une secrétaire de mairie verra sa carrière avancer plus vite elle est en catégorie c'est toujours. Par exemple un agent un agent technique est aussi en catégorie C qui travaille dans la même commune qui peut avoir des suggestions importantes ne verra pas son avancement d'échelon aussi rapide et je pense que ça fera une. Des divergences dans au sein des mêmes collègues donc je trouve ça. Pas très favorable, donc pour moi, tant qu'il n'y a pas une révision générale, ce sera un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Oui madame la présidente, moi ça sera un avis favorable à cet. Amendement. Que je défends et c'est peut être l'occasion d'avoir quelques instants la discussion sur la reconnaissance en matière de rémunération. Pour la secrétaire de mairie avant tout ceux mentionnés. C'est un élément important qui doit trouver traduction dans la loi, c'est des débats que nous avions eu sur, au fond, la forme de reconnaissance que nous pourrions apporter et d'ailleurs nous avions eu ces débats en séance. Le 6 avril à l'occasion de l'examen. La première proposition de loi, vous en souvenez peut-être, j'avais l'occasion de vous donner les dispositif indemnitaire plafond Rifseep qui était à disposition des communes et de vous indiquer qu'ils étaient aujourd'hui assez largement sous-utilisés par les communes et vous m'aviez répondu certainement à juste titre, mais au fond, Monsieur le Ministre, prenez vos responsabilités et se proposer une valorisation indiciaire dans la rémunération fixe de nos secrétaire de mairie. Et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui en réalité et que les dispositifs ne viennent pas en opposition les uns avec les autres qu'est ce que propose l'amendement du président Patriat de dire qu'exercer le métier. La fonction de secrétaire de mairie, effectivement, c'est une responsabilité particulière. C'est une responsabilité distinctive quelqu'un qui est de catégorie B rédacteur qui n'exerce pas la fonction de secrétaire de mairie et un rédacteur une rédactrice qui exerce la fonction de secrétaire mais ça n'est pas la même chose, vous l'avez dit les uns les autres en matière de prise de responsabilité de complexité parfois la présente Gatel le rappeler aussi de prise de risque aussi d'une certaine façon et donc je crois que la philosophie qui consiste à dire au fond dans une logique d'affectation fonctionnelle qu'exercer ce métier là ça vaut une forme de prime en matière de responsabilité, je crois que c'est une logique que nous devrions reconnaître et donc je propose effectivement que nous soutenions cette proposition du présent Patriat pour dire que le temps on exerce ce métier de secrétaire de mairie. Alors on aura une accélération sur ces grilles d'ancienneté, j'avais remarqué que c'est un dispositif qui a inspiré de, de dispositifs qui existent déjà, celui des fonctions qu'on exerce parfois dans des quartiers prioritaires de la ville, c'est d'une certaine façon son inspiration et celui que nous avons créé dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique avec le fait d'acc proposer des accélérateurs de carrière pour des emplois fonctionnels. De façon assez légitime reconnaître la responsabilité particulière de la secrétaire de mairie en adoptant cette possibilité d'accélération indiciaire en matière d'ancienneté et d'un mot, je dis que cette disposition n'est pas antinomique avec notamment le dispositif que vous portez monsieur Vial d'avoir au fond une prime de responsabilité. Je sais, je ne veux pas le débat sur l'article 40, j'en suis pas ici responsable mais je prends mes responsabilités. C'est pour ça que dans mon discours. J'ai évoqué cette question là pour dire que je prenais l'engagement. Dans ce qui est lié FSE aujourd'hui, c'est-à-dire la reconnaissance dans le Rifseep de la fonction de secrétaire de mairie, qu'on puisse accompagner les maires et donc qu'on mène ce travail avec les employeurs. Dans le cadre d'une charte qui viendrait donner les conditions qu'on pourrait. Mettre autour de les fesses en fonction des différentes caractéristiques. Justement particulière à telle ou telle commune pour encadrer et créé par le règlement au fond. Cette disposition indemnitaire qui viendrait, je crois bien compléter le processus d'accélération indiciaire qui est proposé ici par l'amendement de François Patriat. Monsieur Richard, monsieur le président vous aviez demandé la parole. Je souhaiterais tout de même reprendre la discussion. Pour. Différencier de l'argument de Madame la rapporteure parce que. Bien entendu, il peut y avoir d'autres situations à issue au sud d'une d'une analyse transversale d'une négociation sociale dans lesquels on puisse introduire. de de promotion d'échelon en fonction de circonstances particulières mais je crois vraiment que nous ne devrions pas avoir de doute. Sur la nécessité de le faire pour la fonction propres de secrétaire de mairie parce que. je prends évident en plus la comparaison avec la situation du travail en quartiers prioritaires. Il y a un stress. Il y a une pression. Il y a. Le fait qu'il a été mentionné par plusieurs collègues dans le débat que le secrétaire de mairie la secrétaire de mairie porte la responsabilité de la bonne fin de toute une série d'opérations. Dont dépendent. Dont dépend la la vie de la commune et ses intérêts. Donc il me semble vraiment que. La nature de cette mission, la charge mentale qu'elle représente justifie cette accélération d'ailleurs mesuré. De. De d'ancienneté et de promotion comme contrepartie d'une charge mentale particulière donc il me semble que nous devrions voter cet amendement. Merci Monsieur le Président Patriat pour explication de vote. Du débat, tout le monde s'est exprimé en vantant les vertus secrétaire de mairie le caractère exceptionnel de leurs fonctions la multifonctionnalité qu'ils expliquent le fait que c'était des couteaux suisses qu'elles avaient des tatouages. Alors si on veut de notre activité. Il faut quand même au-delà du d'une justice apparente que Madame la rapporteure voudrait rétablir. Il y a une question d'attractivité si on traite de la même façon, secrétaire général de mairie, secrétaire de mairie compterait un agent de service par ailleurs en disant ben il pourrait le faire la même chose, là je comprend plus très bien parce que c'est cette volonté de revenir un peu tiré vers le bas. Ce que nous voulons promouvoir ce n'est pas une façon de reconnaître effectivement dû donner la secrétaire de mairie la reconnaissance qu'elle mérite donc je tiens absolument à essayer de convaincre mes collègues de de voter mon amendement. Madame le rapporteur. Je voulais juste un petit mot pour dire que ça cette mesure là finalement elle est contraire elle elle vient en contradiction avec la mesure qui a été prise il y a quelques années de supprimer les différentes mesures d'avancement d'échelons. Vous savez qu'il avait l'avancement. Normal l'avancement accéléré l'avancement au choix. On a dit on a décidé à un moment de faire un avancement. Unique de droit. Donc en fait on revient en arrière en en faisant un accélérateur. bon c'était tout ce que je voulais dire mais je maintiens. Madame var alias pour explication de vote. Oui, je partage l'avis de Madame. je connais bien ce métier mais je je je me dis franchement qu'est ce qui est plus intéressant pour la secrétaire de mairie pour la elle prend le grade de secrétaire général. Mais elle garde son échelle indiciaire de catégorie. C'est plus que le Reset qui excusez-moi ne n'a ne lui apporte pas grand chose pour la retraite cet avancement d'échelons qui va créer un régime particulier par rapport aux autres catégories professionnelles. Moi je préférerais que vous lui attribuez une échelle indiciaire qui correspondent à ce nouveau grade de secrétaire général. Ça me paraîtrait plus logique. Monsieur le ministre. Simplement précisé pour qui aucune ambiguïté. Ce que nous ferions là si nous adoptions cet amendement, ce serait une double accélération. Secrétaire de mairie qui viendrait promu. Catégorie B elle verrait une progression indiciaire du fait de sa promotion catégorie B et donc l'amendement proposé il y a pas annihiler déjà cette progression indiciaire et à cette progression indiciaire du fait de passer en catégorie B on y ajouterait le fait de franchir des échelons. Plus rapidement parce que je crois que ça a été extrêmement bien rappelé par Alain Richard et François Patriat au fond ça viendra reconnaître que en termes d'expérience une année passée entre homme de secrétaire de mairie ça vaut parfois 2 années passées quand on exerce pas cette fonction-là et donc on viendrait effectivement leur proposer en plus un accélérateur de carrière indiciaire dans la rémunération fixe donc je crois que ça serait à mon sens une occasion manquée de revalorisation en matière de rémunération. Encore une fois sans exclusive de ce que nous pourrions faire comme travail sur le dispositif indemnitaire c'était en partie les débats que d'adopter cet amendement. Donc je me permets d'insister mais je pense que c'est un amendement qui vraiment irait dans le sens de nos secrétaires de mairie et de revalorisation de rémunération. Merci je mets donc on voit cet amendement avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui vote pour. Qui vote contre. 10, absent il n'est pas adopté. à l'article 4 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le sept si les retirer. C'est toujours dans la suite des coordinations le 17 Monsieur Vial. Coordination. Madame le rapporteur favorable. Parfait. Favorable pour le gouvernement je mets donc aux voix cet amendement numéro 17 avec 2 avis favorable qui vote pour. Contre, abstention il était adopté l'amendement 25 monsieur Arnaud. Et madame la présidente. Depuis la loi de du 12 mars 2012, les employes de secrétaire de mairie de communes de moins de 1000 habitants peuvent être occupé de manière permanente par les contractuels. Si l'amendement qui a été proposé par la Commission permet aux communes comptant entre 1000 et 2000 habitants de recruter des agents contractuels pour leur emploi de secrétaire de mairie à temps complet. Le présent amendement vise à élargir la mesure aux communes jusqu'à 3500 habitants. Je constate notamment dans les départements comme le mien, les Hautes-Alpes, des difficultés de recrutement de secrétaire de mairie qui concerne majorité territoire notamment les plus ruraux et ceux de montagne, la possibilité de recruter par la voie contractuelle s'avère être un, un recours salvateur pour un grand nombre de nos communes. Donc cet amendement permettrait à un plus grand nombre de municipalités d'avoir la faculté d'embaucher une secrétaire de mairie, secrétaire général de mairie en tant qu'agent contractuel. En élargissant le seuil à 3500 habitants 4ème groupe démographique au sens de l'article correspondant du code général des collectivités territoriales, ce sont 2300 communes supplémentaires qui seraient visés par cette mesure, dont un certain nombre de chef-, lieu de canton mais aussi de communes de stations de sports d'hiver qui ont souvent une population permanente faible mais qui sont surclassé ont des difficultés de pouvoir recruter dans de bonnes conditions des secrétaires de mairie et donc ont souvent recours à des contractuels, donc d'où ma proposition. Merci. Merci madame la présidente. vient en complément de ce qui a déjà été fait dans la loi, transformation de la fonction publique, puisque dans la loi de transformation de la fonction publique, on était allé que jusqu'à 50%. Bon là on fait un pas supplémentaire pour aller à temps Je ne pense pas que ce soit bien pertinent d'aller au-delà de du seuil de 2000 habitants. Pourquoi, parce que, en réalité il y a relativement peu de communes de plus de 2000 habitants qui embauche une. Attends mairie on est plutôt sur le volet DGS et puis j'allais dire votre amendement peut être satisfait. Parce qu'à partir de 2000 habitants, il est pas interdit à une commune de recruter un contractuel, si il n'a pas d'agents, fonctionnaires qui postule ils peuvent recruter un contractuel déjà donc j'allais dire votre amendement réalité les satisfait. Donc demande de retrait ou avec des fleurs. Monsieur le Ministre, et même avis que le rapporteur, madame la présidente. Vous retirez ou je mets aux voix monsieur Arnaud. Non par principe je le maintiens parce que je considère que ce ce 3500 habitants a d'ailleurs été référente pris comme référence telle heure par Cédric Vial, rappelant que la fonction que DGS commence à partir de 3500 habitants. Je pense que je maintiens cet amendement et l'Assemblée votera ou votera pas. Merci je mets donc aux voix avec 2 avis défavorable qui vote pour.

Oui merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues. Cet cet amendement vise à instituer dans chaque centre de gestion de la fonction publique. Conseil représentatif des agents administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de mairie. Ce conseil sera constitué pour moitié d'élus et pour moitié de représentants donc des agents administratifs. Représentant il émet des avis simple sur toutes les questions d'ordre général qui concerne ce cadre d'emploi. Tout à l'heure nous avons échangé et certainement de collègues ont exprimé une réalité de la situation au regard de l'isolement d'un certain nombre de secrétaire de mairie et que par rapport à cela le fait qu'il puisse y avoir en liaison et un accord avec. Donc les centres de gestion, une instance qui soit une instance de dialogue. Au moment où on parle beaucoup de cette nécessité d'avoir un dialogue social appuyé et et un important je veux dire dans toutes les strates de la société. Eh bien ça pourrait être un élément, un Somme toute. Souvent le dialogue il existe, il existe tous les jours. Entre la secrétaire de mairie et et son élu, mais là il s'agit de sortir de ce cadre cadre hein pour avoir un schéma plus général et avoir cette capacité, cette possibilité donc de d'instaurer un dialogue et qui permet ensuite de pouvoir envisager un certain nombre de pistes, notamment par rapport à des enjeux qui sont des enjeux essentiels, c'est celui de la formation et celui du recrutement et que si les secrétaires de mairie dans le cas de cette instance en accord avec les élus puissent réfléchir sur ces enjeux. Je crois que ce serait une avancée qu'il serait éminemment positive. Même le rapporteur, votre avis. Au sein des. Centre de gestion, il existe déjà des instances paritaires. La la la CRP. La commission administrative paritaire et le comité social territorial, donc il y a déjà des instances qui traite des des caps individuels et des cas collectif. si on fait une instance spécifique pour les secrétaires de mairie, pourquoi on créerait pas une instance spécifique pour les ingénieurs territoriaux par exemple mais si on commence à faire des spécificités dans les dans les cadres d'emplois il faut il faut les justifier ses spécificités. En revanche, il existe. Une instance qui qui embrasse toutes les professions et qui est de niveau national. C'est le sens c'est le Conseil supérieur de la fonction publique. Si on veut, c'est plutôt à cette instance là

Contre, abstention il n'est pas adopté. L'amendement 31. Héritier. Merci madame la présidente. Aujourd'hui les les secrétaires de mairie appartiennent essentiellement à la catégorie C pour plus de 60% avec des salaires globalement insuffisant au regard de leur niveau de responsabilité et des compétences multiples qu'qu'exige leur fonction. Pourtant il existe un large consensus pour considérer que le niveau de responsabilités exercées par un un secrétaire de mairie relève a minima de la catégorie B. Certes, le plan de requalification que propose d'instaurer l'article 1er de la proposition de loi permettra. Des agents de catégorie C exerce exerçant les fonctions de secrétaire de mairie d'actes d'accéder un cas d'emploi de catégorie B, mais cette option ne constitue pas une solution pérenne puisqu'il est prévu que ce plan de requalification expirera au 31 décembre 2028, il paraît aujourd'hui opportun de faire évoluer le cadre légal et réglementaire pour en prévoir que la nomination aux aux emplois secrétaire de mairie relève a minima d'agents de catégorie B, sans que cela empêche pour autant le recrutement d'agents de catégorie C qui accéderait alors à la catégorie B sous réserve d'accomplir une formation qualifiante. Contraint par l'article 40 de la Constitution, le Parlement ne peut mettre en oeuvre cette réforme, sans le concours du gouvernement. C'est le sens de cet amendement qui prévoit la remise d'un rapport dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, je vous remercie. Madame le rapporteur. Alors on va vraiment être disruptif aujourd'hui parce que ça sera le 2ème rapport que je vais accepter. Ce n'est pas courant, mais je pense que cela effectivement est nécessaire. Donc, avis favorable. Monsieur le Ministre. sur un plan de requalification qui est prévu sur 5 ans ce qu'en 2028. Ça me semble un calendrier qui. Sincèrement, n'est pas très opérants et donc même sur cette demande de rapport contrairement à la vie que j'ai tout à l'heure je suis obligé d'avoir un avis défavorable, madame la sénatrice. Merci j'aimais. Donc on voit cet amendement avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui vote pour. Abstention il être adopté. Des amendements sur l'intitulé de la proposition de loi 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune monsieur Arnault.

Sur la dénomination pour Me, secrétaire général de mairie dans l'intitulé de la proposition de loi. Quel est votre avis. C'est l'amendement numéro 8. Oui j'entends. Je je. Je je dirais plutôt un avis. Défavorable puisque le quand on a voté le premier amendement de monsieur Vial, il fait partie il fait part de secrétaire et de secrétaire général. Donc. Ça me paraît pas. Ça me paraît pas être une bonne coordination. On en sers pas le mouvement général dans le dans le. La proposition de loi, Monsieur le Ministre, votre avis. Si si mais je crois que Madame la rapporteure a malheureusement raison. Ça veut dire que nous avions le même avis avec madame la rapporteure de défendre le changement d'intitulé pour adopter celui de secrétaire général de mairie point acquis, nous avions indifférent pour. Avoir une différenciation entre des secrétaires de mairie, catégorie C, D, secrétaire général de mairie catégorie A et B vous avez. Décidé que ça serait secrétaire j'secrétaire général de mairie avec différenciation ce dernier amendement propose d'adopter juste secrétaire général de mairie et donc je comprends la position cohérente de la rapporteure cet amendement me semble maintenant hein cohérent avec ce que vous avez adoptée et donc plutôt un avis défavorable, par cohérence avec ce que vous avez vous même adoptée j'essaie. Il est retiré. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il y a-t-il de demandes d'explications de vote. Donc ça, de nouveau. madame la présidente, monsieur le ministre. Même les rapporteurs, mes chers collègues, nous on et ont pu être aujourd'hui dans une CMP conclusive. Si le travail que nous avions effectué au mois d'avril avait été repris avec cette célérité à l'Assemblée nationale compléter le texte serait donc revenu ici en ayant été une collaboration parfaite entre l'Assemblée et le Sénat. C'est pas le choix qui a qui a été fait et je le regrette un peu, néanmoins. L'apport du Sénat est majeur dans le texte. Déposé par notre collègue Patriat avec nous votons aujourd'hui. Nous avons bien noté Monsieur le Ministre, vos engagements sur la procédure accélérée pour une fois je crois qu'elle est vraiment nécessaire et bienvenu. Nous avons aussi noté l'accord sur les. Le rapport qui avait, qui a été demandé et je pense que nous nous retrouverons. l'espère, au moment du projet de loi de finances pour voir la réalité des engagements qui ont été pris aujourd'hui en tous les cas, c'est un texte utile et je remercie vraiment nos collègues du groupe communiste d'avoir et, et de la délégation aux collectivités territoriales d'avoir initié. Ces travaux Et j'espère que ce texte ne reviendra très rapidement et sera suivie par des dispositions adéquates lors du projet de loi de finances, je vous remercie. Merci. Il y a eu plusieurs demandes de prise de parole. Je voulais simplement vous signaler que nous avons une demande de scrutin public pour vous préparer. Monsieur Vial pour explication de vote. Merci madame la présidente. Je une explication de vote avec un petit goût amer parce que effectivement on aurait pu aujourd'hui voter un texte en étant en sortant la tête haute et en étant content de ce que l'on, que Il y a certaines mesures qui sont intéressantes et je pense qu'on a fait progresser en on a fait progresser la cause et. Je salue. Le le le travail qui a été fait par par nos collègues qui ont travaillé sur ce texte. Néanmoins, il nous manque. Il nous manque quand même un certain nombre de choses et ça aura des conséquences. Monsieur le Ministre, pourquoi il manque des choses parce que justement la procédure qui fait que la PPL aient été déposée avant les travaux de la mission parlementaire fait qu'on n'a pas pu intégrer dans la PPL les les les les mesures que l'on souhaitait et qui n'était plus un peu à cause de, d'un certain nombre d'articles comme l'Arctique 40 par voie d'amendement, sauf bien sûr, Monsieur le Ministre, si vous aviez levez le gage ou ou défendu certains de ses amendements. Ce que vous n'avez pas souhaité faire donc le fait qu'on n'ait pas pu l'intégrer dans la PPL parce que vous avez choisi une procédure parlementaire spécifique qu'on n'ait pas pu les introduire par amendement fait que on sera peut-être probablement obligé de déposer une nouvelle proposition de loi et qu'on en reparlera encore pour pouvoir intégrer les mesures qui manquent à l'appel et dont on a besoin pour que l'édifice d'organisation de ce que l'on souhaite faire. Pour les secrétaire de mairie encore une fois, pour revaloriser leur métier pour leur offrir des perspectives de carrière et pour pouvoir rendent leur métier plus attractif et tout simplement pour pas être en manque de secrétaire de mairie et donc en manque de mer dans quelques années. C'est ça l'enjeu, ne l'oublions pas, mes chers collègues, malheureusement un certain nombre de choix donc j'estime que vous êtes principalement responsable ne nous ont pas permis de conclure définitivement ce sujet, prenons ce qui ce qui a été votée ce soit aujourd'hui et c'est tant mieux, mais malheureusement, nous serons probablement obligé d'y revenir on se reverra Monsieur le Ministre, et en tous les cas, j'en profite pour saluer toutes les secrétaires de mairie qui nous regarde et qu'on salue. Merci madame la présidente. Je crois que nous venons d'apporter une nouvelle Pierre. À l'édifice qu'il convient de constituer pour revaloriser à la fois le métier et même les salaires des secrétaires de mairie. Je ne reviens pas. Les collègues l'ont fait. À maintes reprises et dans des termes. Particulièrement parlant sur la manière dont cette PPL est arrivé jusqu'ici le goût amer qu'on peut avoir les uns ou les autres qu'un gouvernement qui passe son temps à nous dire qu'il veut transcender les courants politiques finalement on n'arrive qu'à une chose, c'est à rassembler tout le Sénat pour lui dire que il y avait meilleure façon de s'y prendre pour avancer ensemble. Il reste du chemin à parcourir. Vous n'avez pas répondu monsieur le ministre, il me semble sur pourquoi votre refus qu'on accélère aussi le passage des secrétaires de mairie, c'est qu'ils sont en catégorie B vers la catégorie. Ah ça me semble important. La formation initiale. Nous venons de voter un rapport et je pense que c'est véritablement un chantier qui doit nous mobiliser tous parce que une des clés de l'attractivité tiendra à ça. Je pense qu'il y a aussi un travail de déprécarisation à faire parce qu'autant et dans notre proposition de loi en accord avec la rapporteure nous avions permis des recrutements de contractuels pour les. Mais en même temps pour pour pallier à la pénurie, il faut faire ça mais il faut en parallèle travailler un plan de déprécarisation et puis je crois qu'il faut aussi et certains l'ont dit très bien aujourd'hui qu'on est en tête la difficulté que financières que peut représenter ce type d'emploi pour des communes qui sont de petites communes et qui ont bien d'autres dépenses qui pèse aussi sur leurs épaules en ce moment et qu'il faut prendre en compte des mesures de compensation pour que tout ça puisse se concrétiser dans la vraie vie dans nos villages. Derrière tout ça il y a l'existence même de nos communes. Il y a la reconnaissance légitime du au secrétaire de nos mairies, mais il y a la reconnaissance et l'existence de nos communes. Je vois que certains sont prompts à se tourner vers les communes à chaque nouvelle crise qui surgit. Il faut aussi. Acté et concrétiser que ces communes doivent avoir les moyens de fonctionner. J'ai coutume de dire qu'elles sont le premier mais souvent aussi malheureusement le dernier service public dans un certain nombre de territoires et il faut les aider à assumer ce service public, merci. Merci. Si Monsieur Billac pour explication de vote. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame le rapporteur, chers collègues. Comme les membres du groupe RDSE. Je vais voter la proposition de loi mais. Je crois qu'on ne va pas assez loin et qu'on réglera. Un peu le problème, c'est un petit pas sur la rémunération pour ceux qui vont débuter la catégorie B c'est le SMIC. C'est le SMIC, la catégorie B, il faut le savoir et encore démarre maintenant au 4ème 5ème ou 6ème échelon de la guérilla.

Quant à leur activité sur la rémunération. Je me pose quelques questions. Et puis, le gros problème c'est la formation, comment faites secrétaire ou une secrétaire de mairie dans une commune rurale où il est tout seul pour suivre à la formation initiale, c'est déjà difficile, là on va mettre une formation complémentaire. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que la réalité du terrain c'est qu'une personne seul ça va hé bien quelle est obligée de fermer le secrétariat. Et. Et c'est ça la réalité dans les communes rurales. Alors moi j'avais des projets amendement sur la formation, mais évidemment on ne mord opposé l'article 40. Au jeu proposé et j'en avais déjà parlé à la Première PPL des contrats aidés. Financés à 80% où il aurait pu se former à autant avant d'accéder. Des aspects de contrats d'apprentissage mieux rémunérés où là il y aurait eu une formation théorique. Dispatchés par adapter ou par l'université et à côté une formation pratique auprès d'un ancien ou d'une ancienne secrétaire de mairie on m'opposer leur quelque 40 hamdoulillah qui avait contrat aidé, mais le niveau de rémunération du le pas est beaucoup trop faible et la durée de ces contrats aidés et beaucoup trop courte pour arriver à former un secrétaire de mairie. Alors je change de bol ça va ça va on a parlé de la mise en place d'une formation universitaire. C'est certainement quelque chose qu'il faut faire mais voilà nous voterons pour, mais avait quand même quelques inquiétudes quant à la revalorisation de ce beau métier. Merci monsieur Richard pour explication de vote. Oui madame la présidente. Monsieur le Ministre, ce sera très court même si ce texte n'est pas parfait, même si. Comme l'a dit tout à l'heure Cédric Vial, certains ont un goût amer dans la bouche. Il faut quand même relever que le vert et et à moitié plein plutôt que de relever qu'il est à moitié vide et moi je voudrais véritablement. Saluer le travail qui a été fait à cet égard lui particulièrement naturellement. Le les les les auteurs de de la PPL, travail de la de de la rapporteure bien sûr au sein de la commission des lois et de façon globale le travail qui est fait ici. Je voudrais aussi. Dire que naturellement, Monsieur le Ministre, nous comptons vraiment sur vous pour trouver les moyens de financement des collectivités locales qui seront amenés naturellement à prendre en charge. Ces revalorisations, même si elles sont naturellement insuffisantes. Et et les intéressés vont nous le dire, cela va encore coûter de l'argent aux collectivités locales et il serait naturellement indispensable que vu les difficultés qu'elles connaissent à l'heure actuelle ne soit pas découragés par des mesures qui, le cas échéant ne serait pas compensée. Monsieur le Ministre, je vous en remercie par avance. Merci Monsieur Durand pour explication de vote. Merci madame la présidente. L'explication de vote que je. Formulerai au nom de de mon groupe ce soir exprimera. Une satisfaction des regrets et des attentes. La satisfaction, c'est qu'on ait pu. Avancer sur un certain nombre de sujets dont nous avons constaté et je le dis en regardant Catherine Di Folco et Cédric Vial. À la faveur de la mission que nous avons conduit pour la délégation aux collectivités territoriales. Beaucoup d'attentes sur le terrain et. Autour. De sujets qui sont extrêmement concret pour les employeurs territoriaux pour les mères. Que sont l'isolement. Des secrétaires de mairie. Le multi-employeurs. La difficulté d'assurer une polyvalence sur des sujets extrêmement variés. La difficulté à assumer des responsabilités qui engage. Le maire, le conseil municipal et on, c'est la pression qui est faite sur les élus en ce moment. La question de la formation initiale. La question de l'accompagnement dans l'emploi, la question de l'animation d'un réseau où les secrétaires de mairie peuvent trouver à la fois. Du soutien parfois psychologique du soutien par les pairs par leurs collègues et puis de l'apport de compétences. La question en fin de la rémunération qui n'est pas. La moindre des questions qui est posée aux secrétaire de mairie, nous avons avancé sur tout cela. Le regret, c'est qu'il ait fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Une première PPL présenté par Céline Brulin, et son groupe. Une mission de la délégation aux collectivités territoriales, une 2ème PPL présenté par le RDPI et on voit qu'on n'est pas encore allé au bout du chemin, donc. Les attentes pour terminer ses vis-à-vis du gouvernement, Monsieur le Ministre que que vous puissiez nous aider puisque c'est vous maintenant à qui nous transmettons la balle que vous nous puis nous aider. Aller au bout de ce travail. Le Sénat a fait son travail. Le Sénat essayé d'apporter le plus, qu'il pouvait apporter. Nous comptons maintenant sur le gouvernement pour transformer l'essai. Monsieur Patriat. La présidente. Et mes chers collègues. D'abord je voudrais remercier tous les collègues qui, qui voteront ce texte. En le remerciant de leur soutien. J'entends bien que ce texte n'est sans doute pas le texte idéal. Auquel chacun d'entre vous d'autres vous aurez Qu'il apporte néanmoins des avancées importantes qu'aucun texte n'avait apporté avant madame brûle hein j'entends vos remarques ne brûle hein mais lorsque nous avons voté à l'unanimité votre texte. Nous n'avons pas émis des réserves sur le texte, nous avons trouvé qu'il était bien qu'il avançait et nous l'avons voté.

Des textes que vous auriez préparé, alors là les amis je me tourne vers la majorité des de la Assemblée du Sénat. Combien de textes présentés par la majorité du Sénat préempte des textes qui sont proposés par le gouvernement. Ensuite, combien de fois et j'ai le sentiment, souvent, combien de fois, combien de fois je le dis comme telle. Donc de grâce passe pas ce procès là nous et même parfois on vous entendant même si on est d'accord sur ce texte et je vous remercie de de le voter. Je remercie les propos d'André Reichardt en particulier de faire la part des choses et de ce que vient de dire Jérôme Durain en disant qu'il y a des avancées mais qu'il y a des autres j'ai parfois le sentiment que lorsque nous déposons un texte, il y aurait une forme d'illégitimité de la part de l'autre groupe à poser que vous auriez des droits supplémentaires à le faire avant nous, mieux que nous. Bah, écoutez, je vous le disais, quand même, à l'instant, je vous en remercie tous et puis j'espère que ce texte obtenir une illimité à tous, merci. Merci, monsieur le Ministre. Je vous remercie madame la présidence, mesdames, messieurs les sénateurs. D'abord au vu des prises de parole qui ont été les vôtres. Je crois que nous nous dirigeons vers un vote à l'unanimité de cette proposition de loi et je ne peux que m'en réjouir Non pas pour le gouvernement, non pas pour le Sénat, mais pour le secrétaire mérite parce que je crois que votre vote ce soir et le travail que vous avez effectué depuis des semaines, depuis des mois. Madame la rapporteur je veux vous en remercier madame brûle hein c'est le président patrie à vous tous ici ça a été un travail utile et qui fait vraiment, je crois, avancer les choses. Pour le secrétaire de mairie, j'ai pris un engagement qui était celui d'engager la procédure accélérée. C'est dire la volonté du gouvernement d'aboutir. D'aboutir rapidement. Je partage le souhait que la Première ministre a émis que nous puissions trouver la niche parlementaire susceptible de l'adopter d'ici l'été et donc nous travaillons à cette à ce dessin là pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et donner une traduction dans la loi définitive et nous nous reverrons peut être au travail que vous ferez autour de la commission mixte paritaire. Je voudrais vous dire de ne pas être trop dur avec le travail que vous avez vous même effectué. Bien sûr que peut être ici ou là on peut avoir des regrets, j'exprime moi-même le regret que nous n'ayons pas adopté cette procédure d'accélération en matière de grilles d'ancienneté qui aurait je crois apporter une rétribution supplémentaire à une reconnaissance supplémentaire en matière de rémunération. Mais ça veut dire qu'il nous reste peut-être encore un peu de travail à effectuer. Bien sûr nous nous heurtons là aux limites de la différence entre le travail législatif travail réglementaire et puis le travail dans la vraie vie, dans la pratique que nous devrons mener en matière de formation de filières universitaires de mutualisation des moyens de travail que nous devrons mener avec les cendres de gestion avec le Cnfpt aussi avec les collectivités avec les collectifs de secrétaire de secrétaire de mairie elles-mêmes parce qu'elle mène un travail sur le terrain utile et donc. Entre les droits formels que nous votons ici et les droits réels. Je crois qu'il doit y avoir notre engagement collectif. Vous avez en tout cas, celui du ministre de la transformation et de la fonction publique que nous puissions dans les actes continuer à améliorer l'attractivité de ce métier essentiel qui fait tenir debout nos communes, celui de secrétaire de mairie et je vous remercie vraiment pour le travail qui a été effectué. Merci. Comme je vous le disais tout à l'heure j'ai été donc saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDPI sur l'ensemble de la proposition de voix, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

et notifié à la présidence. Nombre de votants, 343 Nombre de suffrages exprimés, 342 pour l'adoption, 342 contre 0. Le Sénat a donc adopté. Très bien. Nous allons passer au plateau suivant. Merci Monsieur le Ministre. Après avis de toutes les parties prenantes, nous suspendrons à 20h. Un minima, nous aurons les trois premières interventions. Très bien. L'ordre du jour appelle la discussion en 2ème lecture de la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en 2ème lecture visant à protéger les logements contre l'occupation illicite demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Dans la discussion générale. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti Garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le Ministre. Madame

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, cher Olivier. Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs. Je suis heureux de vous retrouver pour examiner en 2ème lecture la proposition de loi du président Kasbarian donc je veux bien sûr saluer le travail. Travail qui vise à protéger les logements de nos concitoyens contre toute forme d'occupation illicite. Les choses sont claires, la lutte contre le squat est indispensable. C'est d'ailleurs bien sûr, une de mes priorités car, oui, la loi doit d'abord protéger les honnêtes gens. Le texte qui est soumis aujourd'hui à votre approbation je l'espère définitif comporte des avancées majeures en matière pénale administrative et civile. Au pénal, d'abord je tiens à souligner la qualité des travaux parlementaires qui ont permis de préciser le Champ du délit d'introduction ou de maintien dans un local autre que le domicile. Par ailleurs, après la deuxième lecture à l'Assemblée la notion de local à usage économique a été précisé ainsi que l'avait souhaité le président Patriat que je veux ici chaleureusement remercié. Les débats ont également conduit à instaurer une gradation dans l'échelle des peines qui me semble tout à fait bienvenue. Ainsi le squad d'un domicile lieu particulièrement protégés en tant que lieu de l'intime de la vie privée est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Alors que le squat d'un local autre que le domicile est puni d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. Enfin, je salue le fait que la nouvelle infraction punissant le locataire de mauvaise foi qui se maintient. Sans motif de droit dans un local à usage d'habitation soit désormais punie d'une peine d'amende. Sur le volet pénal. Le texte qui résulte de la navette parlementaire me semble donc tout à fait satisfaisant. Je veux saluer votre travail. Monsieur le rapporteur, écharpe, ainsi que l'engagement connue de longue date de votre collègue la scène, autrice Estrosi Sassone. En ce qui concerne la procédure d'évacuation administrative vous avez convenu avec l'assemblée d'élargir le Champ d'application de cette procédure, issu de la loi Dalo pour la libération des domiciles comme des logements vacants. Le Sénat comme l'Assemblée. Convenu de circonscrire ce dispositif à la situation des squatters. Je m'en félicite car la procédure d'évacuation administrative à l'évidence n'est pas approprié pour régler ce type de litige, le texte aborde également la procédure d'expulsion que l'on pourrait qualifier de droit commun. Ainsi, vous avez souhaité de concert avec les députés l'insertion automatique dans le contrat de bail d'une clause de résiliation de plein droit pour impayés de loyers. Cette généralisation constitue. Une avancée en terme de lisibilité et de simplification procédurale. Parallèlement, un consensus s'est dégagé pour imposer un rythme plus rapide à la procédure d'expulsion, je ne peux qu'approuver. Bien sûr ce nouvel équilibre qui permet de faire passer de 3 à un à un non. La procédure d'expulsion tout en préservant le droit au logement pour lequel le gouvernement et en particulier mon collègue Olivier Klein est particulièrement mobilisée, mesdames, messieurs les sénateurs. Il me semble que vous arrivez au bout de vos travaux car la rédaction qui est soumise aujourd'hui à votre haute assemblée est le fruit de nos travaux communs. Il me semble équilibré parce qu'elle renforce les droits des propriétaires sans remettre en cause la protection des occupants de bonne foi. Je forme donc le voeu. Vous puissiez adopter cette proposition de loi en des termes identiques. Au texte issu de l'Assemblée nationale. Merci. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, cher Éric. Madame la vice-présidente de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Alors que cette proposition de loi arrive au terme de son processus législatif. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail des deux chambres. C'est un texte qui traite de sujets importants et de situation profondément humaine. Grâce au travail des deux chambres. Nous avons maintenant un texte enrichi à l'équilibre renforcée. Je me félicite de ces avancées concrètes nécessaires et précieuse. La navette parlementaire a été gage de protection de clarification et de sécurisation juridique. La situation du squatters qui doit être sanctionné à mesure de sa faute et maintenant clairement distinguer de celle du locataire défaillant. Ce dernier devant pouvoir être accompagnées lorsqu'il est de bonne foi. Le squatteur sera plus durement sanctionnés, alors que leurs locataires restera compte elle lui protéger et accompagner quand sa situation. Le justifie. Mesdames, et messieurs les sénateurs, les parlementaires et le gouvernement ont entendu les alertes, les retours des associations pour parvenir à ce texte mesurer et infiniment utile. Le texte que vous allez examiner ne conduira évidemment pas les locataires en impayés de loyers en prison et je m'en réjouis. Il ne réduira pas l'accompagnement social non plus. Au contraire, il stabilise il ne clarifie et ils le déclenchent plus tôt dans la procédure pour combattre dès que possible la spirale de la pauvreté. Il n'empêche pas le juge bien évidemment d'accorder des délais aux locataires qui peuvent payer leur loyer, mais qui ont été confrontés à une période difficile. Le juge conservera le pouvoir de juger au cas par cas en fonction des demandes qui seront faites par le locataire et par et de sa situation financière. Il renforce le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives les CAPEX pour mieux accompagner les locataires. Grâce aux ajouts du Sénat c'est CAPEX seront désarmés davantage territorialisée avec une place accrue des élus locaux et je veux à mon tour remercier tous ceux qui ont permis, ici au Sénat ces avancées, en particulier monsieur le rapporteur. Et Madame Estrosi Sassone et l'ensemble des parlementaires qui se sont associés à ces travaux. Elles seront aussi davantage décisionnaires par exemple pour le maintien des APL et je les inviterai évidemment dans le contexte actuel, à être ouverte. Face aux difficultés rencontrées par bon nombre de nos concitoyens. Elles pourront débuter plutôt leur travail pour que le diagnostic social et financier soit prêt dès que possible. C'est pour cela que je crois très important de conserver tous les efforts faits dans la prévention des expulsions locatives. Il faut laisser le temps du travail social. Il faut laisser au juge le pouvoir d'analyser chaque situation d'être au plus proche des réalités difficiles d'une expulsion qui est toujours un échec. Enfin, et cela me tenait particulièrement à coeur, ce texte renforce les sanctions contre les marchands de sommeil. En tant qu'ancien maire de Clichy-sous-Bois. J'ai été confronté trop souvent à ce qui indument organise des squats en faisant croire qu'ils sont propriétaires des logements en toute illégalité et au détriment des plus faibles. Cela s'inscrit d'ailleurs dans la lutte du gouvernement contre l'habitat indigne dans les procédures ont été renforcé et simplifié par la loi Elan adopté lors de la précédente législature. Ma mobilisation sur ce sujet est constante, elle se traduit dans ce texte et elle continuera de se traduire avec vous et avec les élus locaux de tous bords dans les prochaines semaines. Mesdames, et messieurs les sénateurs, loin des caricatures et des surenchères. Vous avez aujourd'hui à vous prononcer sur un texte équilibré et proportionné. Bâti dans une logique de compromis grâce au travail, je le redis attentif des parlementaires. Mesdames, et messieurs les sénateurs, je le dis, cette proposition de loi n'a jamais eu pour objectif de résoudre la crise du logement dans notre pays. Mais elle permet de lutter contre les abus, contre ceux qui profitent du système et arnaques les petites gens. Elle permet de résoudre des cas insupportable des situations humaine que vous rencontrez lors de vos rendez-vous en circonscription et dans vos départements qui ont été mis en lumière lors des auditions. Que ça soit des petits propriétaires qui se font abuser par des situations intolérables de squat ou bien de locataires de bonne foi qui se retrouvent temporairement en difficulté pour payer leur loyer. Ce texte, assure la juste conciliation entre le droit à la propriété et celui du droit au logement. De droit essentiel qu'il ne faut pas opposer, il permet de protéger tant les propriétaires que les locataires. Mesdames et messieurs pour ma part je n'oppose pas, lutte contre le squat et l'occupation illicite avec une politique ambitieuse et sociale sur le logement, une politique du logement ne peut pas être une politique du squat, une politique du logement ne peut pas être une politique des impayés de loyers. Une politique du logement doit répondre à toutes les attentes légitimes. Je le redis face au mal-logement. L'objectif, c'est l'accès à un logement pérenne. La politique du logement que nous menons est une politique en faveur des plus modestes et des plus fragiles. Jamais dans l'histoire, l'effort en faveur du Losc de l'hébergement d'urgence a été aussi massif que durant ces 2 quinquennat. En 2017, c'était 120.000 places d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, ce soir c'est encore 205.000 places. 6 millions d'euros sont dépensés chaque soir pour l'hébergement d'urgence et c'est l'honneur de ce pays. L'honneur de ce gouvernement. Le plan logement d'abord de annoncée par la Première ministre lors de la restitution du Conseil national de la refondation du logement et que j'aurai l'honneur de présenter la semaine prochaine permet une hausse des moyens afin de prolonger la dynamique positive du premier plan logement d'abord, l'accès à un logement durable. Pour sortir de la logique de l'hébergement d'urgence et notre priorité. Cela passera par la création de 10.000 nouvelles places de pension de famille et de 35.000 nouvelles places en intermédiation locative d'ici la fin du quinquennat. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Ce texte a été améliorée et équilibré. Grâce à un travail transpartisan des deux chambres, il témoigne de notre capacité à construire des compromis au service de l'intérêt général. En réponse aux attentes concrète et quotidienne des Françaises et des Français. Je suis certain que nos débats de ce soir, permettront de continuer à faire oeuvre utile et ainsi de préserver l'équilibre de cette. Proposition de loi qui va dans le bon sens et que je vous invite bien sûr à adopter. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à présent à Monsieur André Reichardt rapporteur de la commission des lois et vous avez 10 minutes, chers collègues. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes réunis une seconde fois pour débattre en 2ème lecture de la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite pour laquelle fait suffisamment rare pour être souligné. La procédure accélérée, n'a pas été engagé par le gouvernement, il faut s'en féliciter. Ce texte traite de deux sujets auxquelles le Sénat et depuis longtemps attentif. La lutte contre le squat d'une part la sécurisation des rapports locatifs, d'autre part. Il y a plus de 2 ans en janvier 2021. Le Sénat a adopté la proposition de loi de notre collègue Dominique Estrosi Sassone. Visant à mieux protéger la propriété privée contre le squat plusieurs dispositions que le Sénat avait alors soutenu ont été reprises dans ce texte initial de l'Assemblée nationale ou intégrées par nos soins dans le texte de première lecture, nous sommes nombreux à regretter que le gouvernement n'ait pas été plutôt à l'écoute, messieurs les ministres des propositions du Sénat, ce qui nous aurait permis de gagner un temps précieux pour lutter contre le phénomène du squat qui affectent régulièrement des petits propriétaires. Je considère donc que le texte sur lequel nous allons débattre aujourd'hui s'inscrit dans la pleine continuité des travaux sénatoriaux, il faut s'en féliciter. Nous pouvons nous féliciter également d'arriver enfin au terme d'un processus. de presque 3 ans depuis le dépôt de la PPL Estrosi Sassone en 2020. Jean revient désormais au contenu de ce texte. Sur les 15 articles qu'il comptait, à l'issue de la première lecture cinq restent encore en discussion, les autres ayant été adopté au supprimer conforme par l'Assemblée nationale. De façon générale, nous pouvons largement nous satisfaire du texte qui nous a été transmis à l'exception de quelques points a relativement mineures sur lesquelles je reviendrai. Nous pouvons considérer ce texte comme un compromis respectueux respectueux des positions des deux chambres qui préserve très majoritairement nos apports et tient compte de nos lignes rouges. En particulier le chapitre trois cas insérer le Sénat et qui vise à équilibrer le texte en renforçant l'accompagnement social des locataires en difficulté a été adopté conforme par l'Assemblée nationale. Monsieur le Ministre Klein vous nous l'avez rappelé et je tiens à mon tour a insisté à cet égard. Sans revenir sur l'ensemble des dispositions de ce texte puisque 10 articles font déjà l'objet d'une rédaction commune aux deux chambres et que vous nous avons largement pu débattre lors de la première lecture. Je centrerai mes propos sur les articles encore en discussion n'n'a cinq, à savoir les articles 4 article premier, à qui crée un délit d'occupation frauduleuse des locaux à usage d'habitation et des locaux à usage commercial agricole ou professionnel n'a fait l'objet que d'une modification sémantique qui ne pose aucune difficulté. Dans la mesure où conformément à la position exprimée par le Sénat en première lecture, le gouvernement n'a pas maintenu son souhait de limiter ce délit aux seul locaux exploiter. L'article 1er c'est avait été adopté en séance publique au Sénat sur proposition de notre collègue Catherine Procaccia il imposait aux préfets de recourir à la force publique dans un délai de 7 jours suivant la décision du juge pour les quoi. Les cas de squat de domicile, j'avais déjà à l'époque exprimé quelques réserves sur cet amendement, en soulignant les difficultés de nature pratique et juridique qui est soulevé notamment le fait que ce délai de 7 jours était inférieur au délai commun de recours qui s'élève, comme vous le savez, à un mois et qu'il était préférable de maintenir un pouvoir d'appréciation à l'égard du préfet lorsque celui-ci est saisi d'une demande de recours à la force publique. Notamment pour tenir compte des éventuels troubles à l'ordre public que pourrait proposer l'expulsion de force. En se reposant sur les mêmes arguments. L'Assemblée nationale il fallait s'y attendre à supprimer cet article lors de la deuxième lecture mes chers collègues, en cohérence avec les réserves que j'avais exprimée en janvier dernier à cet égard, je vous propose de maintenir cette suppression. J'revient désormais à l'article 2 relatif à la procédure administrative des vues d'évacuation forcée plus connu sous le nom de procédure de l'article 38 de la loi Dalo. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'est revenu que sur une seule et des modifications apportées par le Sénat en supprimant la réduction de 48 à 24h du délai dont disposerait le préfet pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux. Elle a en outre compléter cet article afin de prendre en compte les récentes réserves d'interprétation, formulées par le Conseil constitutionnel à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité qui portait précisément sur cet article 38 de la loi Dalo ces ajouts me semble t'utile. Car ils permettront de garantir la plein la pleine conformité de cette procédure à la constitution est ainsi de réserver son assise juridique C'est pourquoi je vous suggère d'adopter cet article conforme en prenant toutefois acte du désaccord attendu sur la réduction du délai de mise en demeure du squatteur de quitter les lieux. Outre des modifications rédactionnelle mineure portant cette fois sur l'article de terre. L'Assemblée nationale a renforcé à cet article le contrôle de l'application du dispositif de mise à disposition dispositions temporaires de logements vacants. En imposant à l'état de vérifier régulièrement la conformité de la mise en oeuvre de ce dispositif aux dispositions légales et réglementaires applicables lorsque ce dispositif bénéficier à des personnes morales de droit privé. Cette précision va dans le bon sens va dans le sens de la position exprimée par le Sénat en première lecture nous avions appelé le gouvernement à accentuer le suivi de ce dispositif pour l'instant quasi inexistant. C'est pourquoi je vous invite à nouveau à adopter cet article dans la rédaction qui nous avait été qui nous a été transmise. Mes chers collègues. Enfin l'article IV. Concernant les pouvoirs d'office du juge en matière d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets des clauses résolutoire de plein droit qui a fait l'objet d'un désaccord substantiel en première lecture entre les deux chambres a pu oublier aboutir à une rédaction que j'estime représenter un compromis. Pour mémoire, l'Assemblée souhaitait initialement conditionner l'octroi de délais de paiement. La vérification des constitutif de la dette locative le contrôle du caractère descend du logement et surtout la suspension des effets de la clause résolutoire c'est-à-dire le maintien de le logement souhaitait, je le répète conditionné tout cela à une saisine du locataire au lieu de la possibilité pour le juge de se saisir d'office en première lecture. Le Sénat a rétabli les pouvoirs d'office du juge en la matière, jugeant qu'il a été dans l'intérêt aussi bien du locataire que les bailleurs que les relations contractuelles soient maintenus et que la dette locative soit acquitté plutôt qu'une expulsion dite ferme en 2ème lecture, l'Assemblée nationale, c'est en grande partie il faut l'en remercier. Aligné sur la position du Sénat en maintenant les pouvoirs d'office du juge pour l'octroi des délais de paiement pour la vérification des éléments constitutifs de la dette locative et la vérification de la décence du logement. En revanche, la suspension des effets de la clause résolutoire c'est-à-dire le maintien dans le juge dans le logement ne pourra plus être accordée par le juge qu'à la suite d'une saisine en ce sens par le bailleur ou le locataire je vous cache pas que pour moi ça a été une vraie interrogation. Et il s'agit, à mes yeux d'un point de vigilance dont il conviendra de suivre les effets. Une fois la loi entrée en vigueur. À ce stade, nous pouvons néanmoins prendre le pari. Le Parti plutôt excusez-moi de faire confiance aux acteurs judiciaires qui devrait adopter une lecture souple de cet article afin de faire en sorte que les locataires soient vraiment informés de leurs droits. Le Sénat a d'ailleurs adopté et c'est à signaler un amendement en première lecture maintenue par l'Assemblée nationale imposant au préfet d'informer les locataires faisant l'objet d'une assignation en justice, de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, et c'est à noter. Je vous propose donc d'adopter également cet article dans la rédaction qui nous a été transmise en guise de conclusion, mes chers collègues, je pense que nous pouvons nous réjouir de l'aboutissement de ce texte de compromis qui constitue, à mon sens un bel exemple. S'il était besoin de le rappeler. De l'utilité de la procédure ordinaire, messieurs les ministres, qui laisse davantage de temps aux échanges et à la construction d'une position commune entre les deux chambres. Je vous remercie pour votre. Merci, avant de suspendre mes chers collègues, je voudrais vous dire que les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observation. Je considère ces conclusions comme adoptée en application du 5e. Alinéa de l'article 13 de la Constitution ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire prises pour son application. La commission des affaires économiques a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable. 23 voix pour aucune voix contre à la nomination de Madame Laurence Bory Bancel à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. Je vais suspendre la séance elle sera reprise à 21h 30 pour la suite de l'examen de ce texte en application de l'article 48 alinéa 3 de la Constitution. La séance est suspendue, bonne appétit messieurs nos ministres et mes chers collègues.